La séance est ouverte le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 26 octobre a été publié sur le site internet du Sénat : nous n'avons pas reçu d'observation, il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement, je vous rappelle que la séance est retransmise sur Public Sénat en Direct et sur notre site internet, chacun sera attentif à respecter au cours de nos échanges, le respect qu'il s'agisse du respect des uns et des autres, ou celui du temps de parole ceci fait partie des principes du Sénat je donne immédiatement la parole au président Claude Malhuret. Pour le groupe, les indépendants républiques et territoires. Madame la Première ministre, une fois de plus, les agriculteurs ont subi les violences, les intrusions les saccages les destructions Les harcèlement de bandes de casseurs de Black blocks et 2 fiché S, soutenu par les idéologues d'une écologie de la décroissance et par des parlementaires qui se déshonore en participant à des manifestations interdites dont ils connaissent à l'avance les débordements. 61 gendarmes blessés, certains par des boules de pétanque et des cocktails Molotov, des conduites d'eau détruit des champs ravagés, rien de nouveau, c'est la 5ème bassine attaqué en 2 ans, celle de Sainte-, Soline avait donné lieu à un travail de concertation exemplaire, toutes les parties prenantes, y compris France Nature Environnement ont validé le projet, c'est celui d'une Corée impérative, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais ils s'en fichent totalement au moment où Poutine coupe le gaz, on s'aperçoit que par leur faute, on a plus assez d'énergie nucléaire et que les Allemands n'en ont plus du tout au moment où ils bloquent les bateaux qui partent d'Ukraine, les mêmes veut le mettre à genoux, notre agriculture, ils ont détruit, en mars dernier 1500 tonnes d'un train de blé pour dire aux paysans qu'il faut produire moins, alors que l'Afrique attend le blé français, combien de temps va durer le délire anti-système d'une minorité des contestataires gavé qui achètent leur salade en sachet dans les supermarchés, sans même comprendre qu'il faut de l'eau pour la produire Ce vandalisme se déroule dans l'indifférence, sur les 35, destruction des installations de recherche végétale 28 plaintes ont été déposées, si procès ont été engagées, une seule condamnation en 2020 à Perpignan, des juges ont même reconnu l'état de nécessité pour relaxer les casseurs madame la première ministre nos agricultures nos agriculteurs, nos éleveurs nos chercheurs n'en peuvent plus, l'immense majorité des Français, des soutiens, mais on ne parle que de ce qui asperge les chefs-d'oeuvre de soupe et qui bloquent les autoroutes, ils ont l'impression que personne ne les défend, pouvez-vous les rassurer et leur dire que la fin de l'impunité est une priorité pour le gouvernement. Oui, monsieur le président, Mesdames et messieurs, le les sénateurs, monsieur le Président Maluret. Comme vous, comme beaucoup de Français, j'ai été choqué par les violences auxquelles nous avons assisté le week-end dernier à Sainte-, Soline dans les Deux-Sèvres et je veux avant toute chose, rendre hommage à nos forces de l'ordre, chaque jour, policiers et gendarmes nous protège, il préserve l'ordre républicain, aucune violence contre n'est acceptable et le gouvernement sera toujours à leurs côtés. Alors mesdames et messieurs, de quoi parle-t-on à Sainte-Soline, un projet de bassines portée et attendue par les agriculteurs du territoire, a fait l'objet de concertations longue et approfondie grâce à ces discussions, le projet a été fortement modifié et je peux en témoigner en tant qu'ancienne préfète de la région Poitou-Charentes, ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l'eau qui a été approuvée en 2019 à la quasi-unanimité des collectivités, bien sûr, mais aussi des associations de protection de l'environnement, ce projet va permettre de réduire les prélèvements dans les milieux naturels, c'est un projet responsable qui lie la réalisation des réserves à des engagements environnementaux pris par les agriculteurs et c'est un projet qui est également nécessaire pour aider ses agriculteurs à faire face à la sécheresse et pour mieux réguler l'usage de l'eau, donc je le dis clairement, c'est un bon projet, il a passé toutes les étapes des processus d'autorisation dans le respect des règles de l'état de droit, il a pu faire l'objet de recours par les opposants, les opposants qui ont perdu devant la justice, malgré un projet écologiquement vertueux, comme le montrent les études du Bureau des recherches géologiques et minières, malgré un projet concerté et attendue par les agriculteurs, malgré les arrêtés d'interdiction de manifester, pris par la préfecture et confirmée par la justice, des manifestations se sont tenues sur ce site, ce le week-end dernier. Si la majorité des manifestants étaient pacifiques, plusieurs centaines d'individus violents ont pris à partie les gendarmes qui protégeaient le site, le bilan de leur action est lourd tirs de mortiers jets de cocktails Molotov, véhicule de gendarmerie détruits et une soixantaine de militaires blessés, ce sont des scènes inacceptable et profondément choquante. Malgré la grande violence de l'agression, les gendarmes ont tenu et sous l'autorité du ministre de l'intérieur, ils ont maintenu l'ordre républicain et je veux à nouveau les remercier et leur rendre hommage et exprimé également toute la ma solidarité et la solidarité du gouvernement avec tous les gendarmes blessés, donc je le dis clairement l'opposition à un projet ne justifie jamais la violence, la justice est saisie et je peux vous l'assurer, monsieur président il n'y aura aucune impunité pour ces auteurs de violence, je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Philippe mouiller pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame le 1er Ministre Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je reviens et bien entendu sur le sujet de ce week-end à Sainte-Soline où nous avons vécu un week-end terrible dans les 2 Sèvres, dans mon département et je tiens à associer mon collègue Gilbert Favreau ici présent, comme vous l'avez évoqué durant 2 jours, cette commune de 350 habitants a vu déferler près de 4000 personnes participant à une manifestation interdite par la préfecture, contestant la réalisation une réserves de substitution, malheureusement, comme cela était prévisible et ressentie environ 400 extrémistes violents étaient associés à cette manifestation, manifestation également par leur présence, par des élus de la République qui appelle aujourd'hui à la désobéissance civique, nous avons vécu des scènes de violence inouïe et comme vous l'avez fait madame le communiste tiens également à saluer l'engagement des forces de l'ordre à apporter tout le soutien aux personnels blessés et a fait six féliciter la préfète des Deux-Sèvres. Ce projet de de réserve, contesté par les manifestants, comme vous l'avez dit, était finalement validé par l'ensemble des acteurs : l'État, le monde à l'école, les associations environnementales, les élus locaux, ce projet est aujourd'hui financé et légalement autorisé, malgré cela, cette manifestation a été orchestrée au nom de l'écologie, mais ce n'est qu'un prétexte politique voulant instituer un système de violence et d'anarchie depuis 24 heures aujourd'hui Sainte-Soline à retrouver un peu de calme malgré ce qui est évoqué par les médias, il n'y a pas de ZAD mais les agriculteurs et les habitants qui étaient, qui ont été harcelés et qui mérite tout notre soutien, Aspire à de la tranquillité, monsieur le Ministre de l'Intérieur, puisque ces questions était dédiée face à ce type d'événement inquiétant pour notre société, quelle réponse judiciaire qui réponse politique, comment faire pour que demain à San souligne comme partout en France, ou un projet d'aménagement et démocratiquement autorisé, nous puissions le réaliser sereinement. On vous réponde : la parole au ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. les 1000 700 gendarmes qui étaient mobilisés, dont plus de 60, vous l'avez vu, ont été blessés, dont quelques-uns très gravement des mâchoire fracassée, des gens qui sont encore à l'hôpital au moment où nous parlons, il s'agit pas de petits faits de délinquance qui se sont déroulées dans votre département, mais des attaques graves contre les responsables de l'Ordre public alors même que cette manifestation était interdite cette interdiction validé par la justice, je veux moi aussi remercier Madame la préfète de ce département qui a été courageuse présente qui a d'ailleurs, je crois, communiquer à bon escient, sans provocation, mais proche des agriculteurs et je veux ici dire aussi que c'était l'outil de travail des agriculteurs qu'on a voulu casser et tiendront toujours avoir le gouvernement en associant le ministre de l'Agriculture et le ministre à la transition écologique évidemment à leurs côtés, ces manifestations, je mets des guillemets extrêmement violente, ce n'est pas le premier jour que le gouvernement les connaît des gouvernements avant nous les ont eu à les gérer, je pense notamment à Bernard Cazeneuve et je veux rappeler que si aujourd'hui nous pouvons fiché S, un certain nombre de personnes ultraviolentes ultra contestataire ou de l'ultra gauche évoquant effectivement le fait que les services de renseignements suivent ces personnes, c'est bien parce que un gouvernement précédent, celui du président Hollande avait considéré que l'ultra violence de l'ultra-gauche était une menace pour la nation pour l'ordre républicain et donc à la fois les moyens de renseignement qui nous ont permis de mettre les 1000 700 gendarmes, empêchant ainsi la ZAD d'exister en constatant, monsieur le sénateur, qu'il n'y a plus que quelques dizaines de personnes aujourd'hui plus personne n'en parle, mais il n'y a plus que quelques dizaines de personnes près du site que les engins de chantiers vont reprendre leur chemin pour construire cette bassine je veux ici dire que nous suivrons particulièrement cette difficulté nouvelle qui est l'ordre public, nouvelle formule, si j'ose dire, des manifestations spontanées, violente parfois extrêmement radicalisés et je vous remercie d'ailleurs d'avoir voté la loi de probation du ministère de l'Intérieur, parce que vous avez pris en considération cette menace et vous avez donné les moyens, ministère de l'Intérieur, d'y répondre. Quelques secondes. Oui, Monsieur le Ministre, nous avons besoin de l'État dans cette opération, nous ne voulons pas revu Notre-Dame-des-Landes, donc nous souhaitons à moi de le mobilisation de chacun. Mais merci, la parole est à notre collègue Evelyne Perrot pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Becht Ministre du commerce extérieur, aujourd'hui même, en fin de matinée, la Russie a annoncé reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur le retrait militaire du couloir de transport, nous ne pouvons que saluer cette excellente nouvelle, le monde entier retient son souffle car avec la suspension de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, nous ne sommes, nous ne sommes peut-être pas passé loin d'une catastrophe économique et humanitaire, cet accord est aujourd'hui vitale pour la sécurité alimentaire mondiale, n'ose imaginer ce qu'il se serait passé si la suspension avait duré dimanche, un navire chargé de 40 tonnes de céréales aurait dû partir pour l'Éthiopie, il est resté à quai lundi, un autre bateau affrété par le Programme alimentaire mondial chargé de 30000 tonnes de céréales destinées à Djibouti est aussi resté bloqué cet épisode montre que la Russie fait peser une épée de Damoclès au-dessus de la sécurité alimentaire mondiale une suspension durable engendrerait une famine en Afrique et une nouvelle flambée des prix alimentaires, monsieur le Ministre se prépare-t-on à une telle éventualité, sur le plan intérieur comment éviter qu'une envolée des cours mondiaux de céréales n'atteigne l'élevage hexagonale qui dépend essentiellement du maïs et des oléagineux ukrainien, la présidente de la FNSEA FNSEA nous a récemment exprimé ses craintes à ce sujet et sur le plan international, pourrait-on en cas de crise débloquer avec nos partenaires européens et américains, une aide alimentaire exceptionnelle. On vous réponde, la parole était ministre délégué en charge. Commerce extérieur monsieur Olivier Beck. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pérou d'abord je voudrais excusez la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, d'autre part, vous l'avez dit madame la sénatrice, la Russie a annoncé aujourd'hui reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, nous la prenons au mot, en effet, en suspendant Soso qu'aux fondements sa participation en fin de semaine dernière, la Russie avait poursuivi dans son cynisme dramatique par un chantage alimentaire et en choisissant délibérément de se servir de la fin comme de moyen de pression et d'une arme de guerre, soyons clairs, l'initiative sur les exportations de céréales en mer Noire, porté par le secrétaire général des Nations-Unies est un succès 9 millions de tonnes de céréales et d'autres produits alimentaires ont exporté depuis le 22 juillet dernier par la voie maritime, l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture a confirmé que les prix du blé avait baissé sous l'effet de la reprise des exportations et c'est le meilleur moyen pour maîtriser le prix sur les marchés, y compris notre propre sécurité alimentaire dans sa guerre absurde et dramatique qui a la Russie est plus isolé que jamais la dernière résolution portée par l'assemblée générale des Nations unies en soutien à l'Ukraine, soutenu par 143 États, en attestent les conséquences de la guerre inquiète et d'ailleurs pas simplement chez nous sur tous les continents, tous les membres du Conseil de sécurité, y compris la Chine avait vivement regretté d'ailleurs lundi à la décision du Kremlin de suspendre l'accord sur les céréales, je rappelle que la France est à l'initiative pour endiguer la crise alimentaire, nous continuerons donc à nous mobiliser avec nos partenaires européens pour la mise en oeuvre des voies de solidarité qui ont permis l'exportation de près de 13 millions de tonnes de céréales et d'autres produits alimentaires nous soutenons également la création prochaine d'un mécanisme d'urgence d'achats groupés d'engrais pour l'Afrique et l'acheminement par le Programme alimentaire mondial des céréales vers l'Afrique et le gouvernement est évidemment à la manoeuvre pour faire en sorte que les prix restent il a et que les approvisionnements soit là, y compris sur nos marchés nationaux, je vous remercie. Madame Perraud quelques secondes. Monsieur le ministre, aujourd'hui nous ne pouvons que nous réjouir que le blocus et cesser, mais nous avons tous en tête les images atroces de la famille, on est de la famine en Éthiopie et vraiment plus jamais ça. Merci, la parole, c'est ça notre collègue Fabien Gay. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, qui avait la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, partout en France, les réseaux de transports en commun se dégrade et c'est la galère quotidienne pour les usagers dans toutes les régions, les autorités organisatrices sont confrontés aux mêmes difficultés avec l'ouverture à la concurrence, les recrutements sont de plus en plus difficile et les démissions sont légion, le service se dégrade et les TER sont en Île-de-France, les rames de métro, tram et RER sont bondés, le pire c'est le réseau de bus qui en grande souffrance avec des bus annulé sans raison et sans solution de report quelques exemples francilienne 80 minutes d'attente pour le bus 545 à Noisy-le-Sec ou encore 61 minutes pour le bus 322 à Montreuil, se rendre à l'école, au travail à tous types d'obligations est devenu un parcours du combattant, le pire c'est qu'en plus d'un service dégradé les régions qui voient leur budget, de plus en plus contraints et qui refuse d'augmenter le versement transport des entreprises envisagent d'augmenter le prix des abonnements pour les usagers en Île-de-France le passe Navigo pourrait passer de 75 à 100 euros par mois, c'est insupportable pour les millions d'usagers alors Monsieur le ministre ma question est simple : quels moyens supplémentaires sont prévus pour établir des transports en commun fonctionnel partout dans le pays. On vous réponde, la parole est au ministre délégué chargé des Transports, monsieur Clément Beaune. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Fabien gay, je vous rejoins sur le fait que, en Île-de-France, en particulier la situation, les transports publics n'est pas à la hauteur de la première métropole d'Europe aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens vivent des galères, ici à Paris et partout en Île-de-France cela s'est renforcée, disons-le clairement, par des pénuries de conducteurs je crois très sincèrement que si nous voulons être efficaces, nous devons partager le détail des constats, ça n'a, n'a pas grand chose à voir avec l'ouverture à la concurrence qui ailleurs effectif qu'en très petite partie et les secteurs qui sont ouverts, la concurrence connaissent exactement les mêmes difficultés que les secteurs qui ne sont pas ouverts à la concurrence maintenant pour répondre à cette difficulté, il faut je crois 2 choses essentiellement la responsabilité et la coopération, la responsabilité, c'est de dire qui fait quoi, nous avons besoin de rappeler que c'est la région Île-de-France Île-de-France mobilités qui est en charge de l'autre le transport qui doit définir qui doit l'améliorer, qui doit aussi fixer les prix, il n'appartient pas au gouvernement, vous pouvez le déplorer, vous pouvez vous en satisfaire de fixer le prix, en l'occurrence du Pass Navigo ni le prix du ticket au quotidien pour les transports publics franciliens la coopération aussi, car évidemment nous devons résoudre cette question ensemble, je rappelle que pendant la crise de la Covid en particulier, l'État a fait pour l'Île de France, il a été légitime mais cela mérite d'être rappelée aussi un effort qui n'a fait qu'il n'a été fait dans aucune autre région de de plus de 1,3 milliards d'euros, dont 150 millions d'euros de subventions et le reste en avance remboursable, nous devons aujourd'hui améliorer les choses, par exemple chez nos grands opérateurs à la RATP à la SNCF, c'est pour ça, je le soutiens que la RATP notamment, mettent en place des primes supplémentaires que la région, les soutiens d'ailleurs enfin et qu'un plan de recrutement de 1500 chauffeurs et déployé pour résoudre une partie de ses difficultés, c'est pour cela que nous devons prolonger aussi nos investissements et continuer à préparer l'avenir, nous aurons à négocier dans les prochaines semaines à nouveau contrat de plan État-Région, là aussi, c'est inédit, les termites 40 % dans le précédent contrat de plan État-Région avec l'Île-de-France nous seront aussi au rendez-vous pour le prochain contrat de plan qui sera en discussion, nous devons aussi continuer d'investir dans la préparation de l'avenir, c'est pour ça, je le rappelle, puisque ce budget sera en discussion devant le Sénat, très prochainement, qu'il y a un milliard d'euros d'investissement pour l'amélioration des transports publics au titre du développement de nouvelles lignes à travers la Société du Grand Paris, donc nous devons trouver une solution, je suis ouvert à d'autres options ensemble en responsabilité, dire qui fait quoi et en coopération aussi. aller. Le ministre-c'est tout un modèle économique, il faut revoir ce n'est pas aux usagers à payer l'ouverture à la concurrence vous voulez recruter des chauffeurs de bus alors augmenter les salaires augmenter le versement transport des entreprises et fait voter dans le prochain budget, une aide supplémentaire, il manque 700 millions à l'Île de France pour que les autorités organisatrices puissent investir dans les transports en commun, c'est une urgence sociale et écologique pour éviter que des millions d'usagers reprennent leur voiture individuelle, enfin le 10 novembre prochain il y aura une journée d'action des salariés de la RATP, la SNCF pour exiger plus de moyens, nous serons à leur côté et nous continuerons à porter ses propositions et à dire que il ne faut pas augmenter le prix des abonnements pour les usagers. La parole est à notre collègue Martin lévrier pendant ce moment gros. Qui au Rassemblement des démocrates progressistes et des. Non, non. Monsieur le président, madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Dussopt Ministre du Travail du plein emploi et de l'insertion, aides à domicile, aides-soignants, agents d'entretien, serveur, maçon, plombier chauffagiste, ouvriers des travaux publics, employé de libre-service, tous ces métiers ont un point commun celui d'être des métiers sous tension, phénomène accentué par une reprise économique post-Covid, plus rapide et plus forte, on ne compte plus les secteurs qui font actuellement face à ces pénuries de main-d'oeuvre, chacun d'entre nous le constate au quotidien dans son territoire, nous sommes nombreux à être saisie par des employeurs qui peinent à recruter et qui sont en manque de solutions concrètes de premières mesures ont été mises en oeuvre par le gouvernement bonus-malus alternance, apprentissage, pour n'en citer que trois cependant, au regard de la complexité de certaines réalités locales, cela ne suffit pas pour résoudre ces difficultés de recrutement, une autre piste pourrait être envisagée, celle du recours à la main-d'oeuvre étrangère déjà déjà présentes sur le territoire national, il importe de rappeler que le taux de chômage de ce public avoisine les 15 % alors qu'un grand nombre de ne demandent qu'une chose : travailler et avoir une c'est une situation stable régulière et sécurisé, en un mot s'intégrer par le travail, monsieur le Ministre, dans le cadre de la réflexion sur le futur projet de loi Asile et immigration que prévoyez-vous pour encourager cette insertion par le travail pour répondre à la problématique des métiers sous tension, vous avez évoqué dans une interview donnée avec Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer Gérard le Darmanin une 2ème idée, celle de créer un titre de séjour métiers en tension,

autour desquels nous aurons l'occasion de débattre avec vous, à l'occasion d'un débat parlementaire avant la fin de l'année, puis dans le cas de l'examen d'un futur texte de loi autour de l'immigration nos, nos objectifs sont très simples : en réalité, c'est à la fois mieux faire respecter les règles, faire en sorte que les décisions de justice, les décisions administratives soient mieux appliquée et ça nécessite aussi de la fermeté des moyens dans leur application, mais c'est aussi faire en sorte que les étrangers présents en France soit mieux intégré, nous sommes convaincus que le travail est le premier outil d'intégration des étrangers qui vivent sur notre sol ça a longtemps été le cas, et depuis, le chômage de masse, ce lien entre le travail, l'immigration, l'intégration s'est distendu, ce ce ce cette ce chantier en ordre et faire en sorte que le travail redevienne une valeur d'intégration notre système aujourd'hui ne le permet pas, nous avons des trappes à inactivité, avec un certain nombre de demandeurs d'asile dont nous savons pertinemment qu'ils viennent de pays suffisamment dangereux pour que l'asile soit accordée qui doivent attendre très longtemps avant d'avoir le droit de travailler, nous avons des immigrés qui bénéficie d'un titre de séjour pour raisons professionnelles qui doivent solliciter une autorisation administrative pour chaque contrat de travail, il faut aussi leur simplifier la vie, et puis nous le savons, nous avons aussi des travailleurs en situation irrégulière, mais qui travaillent parfois depuis longtemps et dans des métiers en tension, le métier de la restauration, le métier parfois du bâtiment, nous avons d'ores et déjà procédé à un certain nombre de régularisation, je pense à l'application de la circulaire prise par Manuel Valls, qui concerne 7000 admission exceptionnelle au séjour mais ces régularisations nécessite un engagement, un accompagnement de l'employeur, nous voulons que ces travailleurs en situation irrégulière, mais dont nous avons tant besoin puissent eux-mêmes solliciter leur régularisation, il ne s'agit pas d'une régularisation massive, c'est du cas par cas, c'est de l'étude de dossier, il faudra pouvoir prouver d'une ancienneté sur le territoire de l'exercice d'un métier apparaissant sur la liste des métiers en tension mais ça répondra à la fois aux besoins de l'économie et ça répondra encore plus profondément à un besoin et une volonté de construire un projet personnel un projet familial et ainsi de faciliter l'intégration de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sur notre sol, et qui vivent avec nous.

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, en raison des crises successives, un nombre croissant de nos concitoyens se trouvent en situation de grande précarité, et ils sont de plus en plus nombreux à devoir recourir à l'aide alimentaire pour se nourrir au quotidien dans mon département, les bénéficiaires de la Banque Alimentaire ont augmenté de 5 % en un an, ça ne représente aujourd'hui 42000 personnes, soit plus de 10 % de la population de la Haute-Vienne l'aide alimentaire, a su se professionnaliser pour répondre à ces nouvelles demandes, mais elle fait face à une grave pénurie de produits en raison de scandaleux gaspillage les organisations constatent avec amertume que la loi n'est pas respectée : de nombreux magasins et entreprises du secteur agro-alimentaire persiste à jeter d'importantes quantités de produits qui pourraient pourtant résoudre les problèmes d'approvisionnement, on compte d'ailleurs à ce jour, une baisse de 6 % de la ramasse de ces produits, pourquoi pour essentiellement une question de profit plutôt que de donner la totalité de leurs excédents aux associations, les grands groupes préfèrent revendre leur surproduction à des des Stocker, chez qui se retrouvent le gaspillage alimentaire car ils peinent à revendre, tous les produits récupérés, une solution multiples bénéfices consisterait à obtenir des produits en circuit court auprès des agriculteurs et des producteurs locaux disposant d'excédents, le problème est qu'ils ne bénéficient actuellement d'aucune mesure de défiscalisation pour les donc il pourrait effectuer, Madame la Ministre que comptez-vous faire pour faire appliquer correctement la loi, que proposez-vous pour soutenir l'achat local et plus largement l'aide alimentaire. On vous répond n'a pas volé. La secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire Madame Schiappa n'avait la parole. Merci monsieur le président, madame la première ministre monsieur le sénateur Christian renonce à je vous remercie d'abord pour votre question relative à la question du gaspillage alimentaire et vous avez raison de rappeler la loi portée par Guillaume Garot, qui a notamment permis d'interdire de rendre impropre les denrées alimentaires et d'obliger les acteurs à porter une convention de don avec une association habilitée, chargé de la vie associative, je veux bien sûr commencer par rendre hommage à toutes ces associations et à ses acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'engage très concrètement sur le sujet du gaspillage alimentaire mais je veux rappeler également que lors du précédent quinquennat nous avons continué à oeuvrer pour renforcer cette lutte, notamment avec les loi Egalim mais aussi avec la loi Hajek dans ce cadre, nous nous sommes fixé l'objectif de réduction de 50 pour 100 du gaspillage alimentaire d'ici l'année 2030 et pour cela nous un l'ensemble des acteurs de la chaîne en renforçant les exigences en matière de suivi de contrôle de qualité de dons d'obligation de dons d'ailleurs via la restauration collective et je vous annonce que nous lancerons prochainement un Label national anti-gaspillage afin de clarifier et de valoriser ces initiatives, il sera porté par Marc Fesneau et Christophe Béchu, chargé de l'Agriculture et de la transition écologique, merci pour eux, c'est donc une mesure de la loi Hajek que nous pourrons mettre en oeuvre, parce que comme vous le savez les français sont toujours plus sensibles à leur manière de consommer l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, Phoenix, dit par exemple que 84 % des Français privilégient un supermarché identifié par un Label de ce type, la question du gaspillage alimentaire et de l'accès à l'alimentation sont fondamentales pour nous, c'est d'ailleurs pourquoi demain la première ministre Élisabeth Borne ira en déplacement dans une banque alimentaire et nous aurons l'honneur de l'accompagner avec le ministre des solidarités Jean-Christophe Combe pour être toujours au plus près des acteurs de terrain, je vous remercie.

par les choix politiques et budgétaires qui ont été les siens dans ce contexte, le gap, le gaspillage alimentaire et le manque de solidarité sont intolérables pour nos concitoyens, lors du débat budgétaire qui vont s'ouvrir au Sénat, notre groupe proposera des mesures immédiates et concrètes pour faire face à l'aggravation de la crise à l'inflation record que subit le pays afin que la solidarité, et notamment la solidarité, la solidarité alimentaire soit dignement assuré. Merci, la parole est à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, 12 millions de Français sont victimes de précarité énergétique parce qu'ils vivent dans une passoire thermique ou ne peuvent pas se chauffer, comme il le souhaiterait, avec la crise énergétique et l'hiver qui arrive, il est à craindre que ce chiffre augmente de manière dramatique, la nécessaire rénovation massive des logements doit donc plus que jamais être une priorité, le rythme de rénovation et d'efficacité de MaPrimeRénov'doivent être renforcés, car la France compte encore plus de 5 millions de passoires thermiques, c'est aussi un enjeu de transition écologique le logement représente 43 % de nos consommations énergétiques et génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre après la défenseure des droits, qui a pointé de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des demandes de subventions, la Cour des comptes vient de publier sa dernière évaluation citant de trop nombreuses réformes ayant nuit à la lisibilité du dispositif, un suivi approximative de son efficacité, un pilotage inadéquate et la complexité des structures d'accompagnement beaucoup de territoires pourtant très engagée pour apporter un soutien technique et financier aux porteurs de projets font aussi remonter les obstacles à l'aboutissement des dossiers, procédure longue et complexe, instructeur qui ne répondent pas de vie trop spécifique qui mettent en difficulté nos artisans locaux, sans compter les dossiers complets qui attendent depuis un an, le versement de la prime. Par ailleurs, outre des problèmes techniques récurrents sur la plateforme, la dématérialisation totale de la procédure exclut certains bénéficiaires potentiels, je rappelle que 14 millions de Français souffrent d'électronicien problématique que mon groupe connaît bien puisque nous avons fait adopter par le Sénat une proposition de loi sur ce sujet l'an dernier, or les guichets rénovent action et les maisons France service n'ont ni le temps ni les moyens d'accompagner dans le détail, chaque demandeur Monsieur le Ministre, avec le coût de l'énergie qui explosent et qui impacte fortement le pouvoir d'achat des ménages, comment améliorer le dispositif pour ne laisser aucun bénéficiaire sur le bord du chemin, je vous remercie. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Gold, vous avez raison. Ma prime rénovent est un dispositif essentiel pour notre transition écologique comme vous le soulignez, ce dispositif doit être accessible au au plus grand nombre et à à ceux qui en ont le plus besoin, je tiens à dire que ce dispositif est perfectible, bien évidemment et et nous y travaillons tous les jours d'arrache-pied avec l'ensemble l'ensemble des membres du gouvernement, mais néanmoins c'est 1,5 millions de chantiers qui ont vu le jour depuis 2 ans, soit plus que l'objectif qui nous avait été donné par le président de la République et par madame la première ministre puisque l'objectif était de 700000 logements par an, néanmoins, il faut aller plus loin, au-delà de cette massification, il faut aller plus loin dans la performance de ces chantiers et dans la globalisation des des moyens qui sont donnés à chacun de porter ce projet de rénovation thermique, c'est pour ça que l'accueil France rénovent par un conseiller France rénove et renforcée que nous allons mettre en place des des accompagnateurs rénovent pour que chacun puisse avoir toutes les informations nécessaires et c'est aussi pour ça que dans le PLF 2023, nous avons encore augmenté le le projet MaPrimeRénov'à 2,6 milliards d'euros, bien évidemment, ces dispositifs touche l'ensemble du territoire 49 pour 100 des chantiers sont dans des chantiers en zone rurale et au regard de la population de ces zones, ça démontre que ces quartiers sont ces zones rurales sont particulièrement touchés, bien évidemment, les passoires thermiques sont aussi en zone dense et nous travaillons aussi d'arrache-pied sur la question de l'habitat collectif et des copropriétés, c'est le sens de MaPrimeRénov'que les copropriétés, sur lequel nous travaillons aussi pour ouvrir le champ permettre aux conseils syndicaux et aux copropriétaires d'un d'accéder à des chantiers en toute connaissance de cause, je peux vous assurer que nous sommes extrêmement mobilisés que nous disons, comme vous l'ensemble des rapports qui pointent des dysfonctionnements, comme on dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain il y a beaucoup d'effets qui ont déjà extrêmement positif sur MaPrimeRénov'juste un exemple, l'et 1 virgule 5 millions, c'est l'équivalent d'économie de des consommations d'énergie, de la ville de Lyon que nous avons déjà économisé pour le portefeuille et pour la planète, merci.

Monsieur le président, Monsieur le ministe revenons dans les Deux-Sèvres. Je savais que ça vous ferait plaisir je souhaiterais tout d'abord me concentrer sur le fond de cette question de l'eau ayant une vision d'ensemble une réflexion globale rationnel et scientifique, la question posée, hé bien qu'quelle l'utilisation de l'eau pour quelle agriculture, contrairement à ce que répète en boucle leurs promoteurs, il ne s'agit pas de récupérer directement l'eau de pluie le MBK bassines sont remplis, principalement par des systèmes de pompage dans les nappes phréatiques et les cours d'eau ceci accentue la pression sur les ressources alors que l'ENA peinent à se reconstituer sans recharge hivernale suffisante, les zones humides et les sols sont impactés, c'est donc l'agriculture et la biodiversité qui sont mises en danger, nous ne sommes pas là dans une logique collective de création de réservoirs d'eau qui se re-initiée par toutes les parties prenantes, mais bien dans une logique d'accaparement de ce bien commun par une minorité pour une production inadaptée destinés à l'exportation, où l'élevage industriel, nous dénonçons le déni démocratique et le court-termisme, la manière dont s'implante les mégabassine est révélateur d'une absence de gouvernance partagée autour des orientations agricoles d'un territoire pourtant d'autres solutions paysanne et innovant d'irrigation existe adapter au changement climatique, elles sont déjà pratiqués sur les fermes d'agro-écologie, monsieur le Ministre, quand allez-vous stopper ces projets n'ont pensé qu'il revienne à poser une rustine sur un schéma sans avenir, à quand une gestion de l'eau, transparent, démocratique et profitable à toutes et à tous votre gouvernement par uniquement de la violence et agite scandaleusement le mot d'éco-terrorisme une stratégie d'écran de fumée pour ne pas parler du fond. On vous répondre avant le au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le président, madame la première ministre, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Salmon. Oui. Vous avez raison, la question de l'eau mérite mieux que des postures. Elle mérite en tout cas certainement mieux. Que des cassage en règle comme ce à quoi nous avons assisté pendant tout le week-end. Vous avez soutenu à la primaire écologiste Yannick Jadot en défendant l'idée au moment où vous lui avez apporté son soutien, qu'il y avait besoin d'incarner une écologie politique qui soit faite de respectabilité, on a vu la manière dont l'écologie politique est respectable était accueillis par une minorité de manifestants : avec ces inscriptions très poétique sur les portières de la voiture maintenant pour aller sur le fond pour aller sur le fond, il s'agit de réserves de substitution. De substitution, c'est-à-dire très précisément que ce projet, il est soumis à des autorisations, il vise à faire baisser les prélèvements de 70 % dans les étages, vous invoquez la séance, les études du BRGM du mois de juillet démontre qu'on préserverait, à la fois le niveau des nappes pendant l'été et que nous aurions un impact positif en sécurisant les alimentation d'eau potable et en faisant en sorte de préserver la biodiversité si vous allez du côté de la science, vous avez des arguments maintenant j'aimerais qu'on s'arrête sur les slogans oui, la priorité c'est la préservation de l'eau sous et donc de diminuer nos prélèvements et nos usages, c'est la priorité, elle est au coeur, à la fois des Assises du Varenne et de la démarche que nous avons lancée avec Bérangère Couillard, à la fin du mois de septembre à Marseille. L'accaparement pour la grippe Business, on a affaire à 300 agriculteurs en coopérative, qui pour la plupart, sont dans la polyculture élevage, on a un projet qui n'est pas celui du gouvernement qui est celui, soutenu par la région socialiste par le département républicain par les élus ruraux de tous bords et quand on parle d'accaparement s'il vous plaît, un agriculteur quand il fait une réserve, il a fait, pas pour sa consommation personnelle, mais pour nous nourrir, à la fin on augmentera les importations si on condamne les adaptations notre modèle agricole. modèle agricole. Il ne vous a pas échappé que nous venons de vivre une année dramatique avec la canicule et la sécheresse avec des aléas climatiques, qui ne sont pas prises en compte dans les études du BRGM, on se base sur des statistiques sur les années les décennies passées, c'est pas ça qui va se produire demain votre politique du bulldozer pour soutenir un système obsolète, ne pourra pas durer longtemps comme ça. La parole est au président François Noël Buffet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous venons de vivre un week-ends dramatiques et pour cause : la violence à Sainte-Soline a atteint des sommets, dont on peut craindre qu'elle puisse éventuellement se renouveler ce que nous ne souhaitons pas. Des forces de l'ordre et des gendarmes ont été blessés, nombreux, cela est inacceptable, naturellement, d'ailleurs, il faut saluer leur travail ainsi que celui de la préfète qui a piloté les opérations cette montée de violence, elle est venue ailleurs sous d'autres formes, on a dégradé, à un moment des Oeuvres d'art. On a également bloqué la circulation, manifester, créer des tensions extrêmement fortes. Y compris avec des risques de conflit réel. Dans 2 ans la France organise des jeux Olympiques de 2024 dès l'année prochaine la Coupe du monde de rugby, monsieur le ministre, on nous a indiqué que tout ce travail était en préparation, vous êtes venus vous exprimer récemment devant la commission de la culture, ainsi que la commission des lois, au regard de ce que nous vivons en ce moment et de cette montée de violence inacceptable comment êtes-vous en train de préparer cette opération, avec quels moyens et surtout à quel moment déposerez-vous un texte devant le Parlement pour que nous puissions légiférer, je le pense en tous les cas au plus vite. On vous réponde : la parole au ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, buffet, comme vous, je constate, et c'est vrai dans beaucoup de pays qui nous entourent, que les grands événements ou les grandes expositions les grands moments médiatiques sont aussi le moment des contestations les plus violentes symbolique mais vous l'avez dit vous- même les plus violentes et que nous nous préparer à cela, au moment d'accueillir des grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby en septembre prochain et les Jeux olympiques de Paris, vous avez bien voulu souligner que je suis devenu avant, je suis venu à votre demande, détailler les moyens que va mettre le ministère de l'Intérieur, à la demande de la Première ministre et du président de la République pour garantir la sécurité en terme d'ordre public de lutte contre le terrorisme est évidemment de lutte contre la délinquance j'ai eu l'occasion de vous dire que les 45000 policiers gendarmes qui seront mobilisés chaque jour sont sans précédent dans l'histoire de notre pays pour prendre au sérieux, bien évidemment, cette menace, vous évoquez quel texte nous allons déposer j'allais vous dire que vous l'avez déjà en très grande partie étudier, monsieur le président, puisque la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, celles qui recréent 11 unités supplémentaires de forces mobiles qui renforce considérablement les renseignements et je pense que l'une des clés de notre réussite, si j'ose dire, ce week-end était le renseignement qui a bien fonctionné, qui nous a permis de proportionner la réponse en nombre de gendarmes, de pouvoir mobiliser l'action de Madame la préfète et empêcher la ZAD de s'installer un des travaux de la bassine de continuer à être effectuer ce renseignement va considérablement renforcer, vous le savez, monsieur le président, dans la loi qui est en ce moment en train de discuter, Assemblée nationale, il est par ailleurs des dispositions qui peuvent concerner directement les grands événements sportifs, il ne m'appartient pas, c'est à la Premier ministre de le faire que de pouvoir voir comment nous pouvons compléter ou améliorer avec la ministre des Sports, les moyens pour aider les préfectures et les forces de l'ordre d'intervenir le mieux possible, Monsieur le Président, que nous sommes tous très concentrés pour que la fête du sport, des coups de Coupe du monde de rugby des jeux ou des Jeux olympiques ne soit pas le lieu de l'ultraviolence, d'où qu'elle Vienne, hein, quelque soit le sujet. Monsieur le Président, buffet. Monsieur le président, 600 1000 personnes sont attendues sur les quais de Seine et plus dans Paris naturellement pour cet événement avec Laurent Lafon nous avons après les événements du Stade de France fait une quinzaine de propositions, vous avez indiqué vouloir les reprendre en compte c'est parfait mais parmi ces propositions, il y avait la manière d'associer les deux Commission et le Parlement à ce à ce travail préparatoire pour s'assurer qu'effectivement, il souhaite une véritable réussite pour la France et nous attendons évidemment vos propositions, de ce point de vue là merci La parole est à notre collègue Hussein Bourgi pour le groupe socialiste, écologiste. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Clément Beaune Ministre des transports, Monsieur le Ministre, le 15 décembre 2013, c'est dans la joie que la ligne à grande vitesse, relier le Languedoc-Roussillon et la Catalogne, la France à l'Espagne, à raison de 4 dessertes par jour entre Paris et Barcelone, en passant par Valence, Nîmes, Montpellier et Perpignan, ce sont des chefs d'entreprise des scolaires, des étudiants, des touristes qui ont voyagé dans les 2 sens, nous venons d'apprendre. Qu'en raison de l'ouverture à la concurrence et des accords commerciaux entre la reine fait la SNCF à compter du 11 décembre prochain c'est 4 dessertes quotidiennes à passer à 2 nous avons appris par la même occasion que la ligne à grande vitesse entre Lyon et Barcelone s'arrêter et la ligne à grande vitesse entre Marseille et Madrid s'arrêter aussi, monsieur le ministre, à l'instar de tous les élus de ma région l'Occitanie, mais des régions voisines aussi, à l'instar des chambres consulaires, des acteurs économiques, à l'instar de toutes celles et ceux qui ont oeuvré depuis tant d'années pour que nous puissions relier le sud de la France à l'Espagne, nous en appelons à votre autorité, ainsi qu'à celle de votre homologue espagnol afin que les dirigeants des 2 entreprises SNCF et Rennes fait reviennent à la raison dans l'intérêt de nos territoires, leur développement économique, je vous remercie. On vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des transports, vous avez la parole monsieur Boon. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous avez raison sur l'importance stratégique de cette lésion qui a été inauguré il y a un peu moins d'une décennie et il avait été indiqué à la suite on le redonne l'effondrement des trafics mais néanmoins de la nécessaire préservation de cette ligne par la SNCF d'une part, et son partenaire espagnol, la reine fait d'autre part, il y a quelques mois, qu'à la fin de l'année leur partenariat s'arrêterait, j'y reviendrai, cela n'est pas irréversible, mais aujourd'hui, cela signifie qu'il faut réorganiser cette offre se se fait par étapes, il y a une première étape qui commencera le 11 décembre prochain et qui permettra à la SNCF, seul d'avoir d'ores et déjà 2 allers-retours entre Paris et Barcelone, ça n'est pas l'offre que vous évoquez, mais c'est une première étape et ça n'est pas la fin de ce partenariat ou de l'histoire de cette liaison, c'est très important d'ailleurs de préciser aussi, puisque vous avez rappelé l'importance pour votre territoire, en particulier de cette liaison que ces 2 allers-retours passeront par le département de l'Hérault en particulier avec des arrêts à Montpellier, à Sète, Agde et nous continuerons à encourager cette coopération nouvelle coopération entre la SNCF et Rennes pour améliorer l'offre, je m'engage à mener ce travail avec mon homologue espagnol sur ce sujet, j'ai échangé avec elle le 21 octobre dernier je la rencontrerai à Madrid en début d'année en liaison évidemment avec les élus et les parlementaires concernés, en particulier sur les autres liaisons, je tiens à préciser aussi que ceux qui se mettent en place, à défaut de ce partenariat renouvelé, c'est que la reine fait va reprendre les liaisons entre Lyon et Barcelone, d'une part entre Madrid et Marseille, d'autre part, et donc il y aura bien une liaison qui là aussi sera reconduite, reconduite, même si les fréquences doivent être encore rediscuté je précise aussi, puisque cela est une autre liaison importante entre la France et l'Espagne, même si vous n'avez pas évoqué que il y a une à Khadr qui s'arrête à la fin de l'année aussi pour la liaison entre Perpignan et Figueras et que je me suis engagé avec mon homologue espagnol a demandé à nos 2 opérateurs de trouver aussi une solution de continuité pour cette liaison, donc je suis prêt à continuer de travailler avec vous pour que nous améliorions les choses pour que ce partenariat, même s'il n'est pas reconduit à l'identique, puisse déboucher sur d'autres types d'options qui n'est pas une pénalisation de ces liaisons qui sont importantes, je rappelle aussi, puisque vous avez évoqué la question de la concurrence que notre opérateur, la SNCF est est présent sur le marché espagnol je crois pour le bienfait de l'entreprise et aussi pour le bien fait de millions d'utilisateurs sur la liaison entre Madrid et Barcelone. Monsieur Régnier je vous remercie, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question : on avait répondu en n'apportant des éléments sur une offre qui sera dégradé et qui dit offrent dégradé, ça veut dire impossibilité de faire l'aller-retour dans la journée et ça concerne en particulier les chefs d'entreprise lorsque vous me dites que dans quelques semaines ou dans quelques mois, la reine fait pour exploiter ou reprendre certaines lignes, rien n'est acquis à ce jour, et puisque vous avez évoqué le Covid Monsieur le Ministre, je voulais vous dire que partout en France, sur le territoire national et je vais parler des liaisons entre Bordeaux et Paris, entre Brest et Paris, rien n'est satisfaisant parce que nous ne sont pas revenus à la situation antérieure au Covid aujourd'hui, les trains fonctionnent, ils sont pleins, remplis, les prix flambent, avec parfois une insatisfaction des voyageurs puisqu'effectivement il y a des retards et je vous demande vraiment de réfléchir à la stratégie de la France en matière de la LGV. La parole est à madame la présidente, Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adressait à la ministre des Affaires étrangères, le 14 septembre dernier le président Larché recevait le Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, ce médecin gynécologue obstétricien, opère chaque semaine dans son hôpital de Panzi des victimes de viols et de mutilations perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo, ces violences sont connues depuis plus de 20 ans en 2010 un rapport de l'ONU, le rapport Mappy dénonçait ces crimes de guerre, or depuis, rien ne bouge vraiment, et le tout sur fond d'enjeux économiques importants dans cette zone qui est un gros producteur de cobalt et de coltan donc ma question est la suivante : quel a été, quelle est l'action de la France pour porter la voix au niveau international de ces populations martyrisées qui mérite, certes la reconnaissance mais surtout condamnation des auteurs, justice et réparation.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente de Roche, en effet, la recrudescence des violences dans l'est de la République démocratique du Congo est préoccupante, en particulier la reprise des combats entre le M23 et les forces armées de la RDC depuis le 20 octobre après plus de 3 mois d'accalmie, nous condamnons depuis longtemps, les activités de tous les groupes armés, les appelant à cesser le combat à déposer les armes et à prendre part au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, il est nécessaire que toutes les parties mettent en oeuvre rapidement leurs engagements, notamment ceux qui ont été pris, lors d'une réunion initiée le 21 septembre dernier par le président de la République à New York pour établir un dialogue régional apaisée et contribuer à la stabilité dans l'est de la RDC, la situation actuelle démontre l'importance de la lutte contre l'impunité en RDC, la France joue un rôle moteur au sein du Conseil de sécurité des Nations-Unies pour ce que la Monusco continue à être dotée d'un mandat exigeant en la matière et elle soutient également la mise en oeuvre de mesures restrictives au niveau des Nations unies et de l'Union européenne contre des personnalités, responsables de graves violations des droits de l'homme, enfin nous soutenons depuis de très nombreuses années, l'action du Docteur Denis Mukwege en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, notamment à travers l'appui à son hôpital et à sa fondation à Bukavu, dans la droite ligne de l'engagement pris par le président de la République lors du sommet du G7, présidé par la France en 2019, notre pays a également mobilisé plus de 6 millions d'euros au profit du Fonds mondial pour les survivantes de violences sexuelles liées au conflit qui l'a qui a avec Nadia Mourad merci. En effet, le Docteur Denis Mukwege et compte beaucoup sur la France et sur les autres pays d'ailleurs, et je voudrais dire, redire ses propos qu'il avait tenu lors de son prix Sakharov en 2014, chaque femme violée je l'identifie à ma femme : chaque mère violée je l'identifie à ma mère, chaque enfant violée je l'identifie à mes enfants, quel est cet être humain doué de conscience qui se terraient quand on lui amène un bébé de 6 mois dans le vagin, été détruits, soit par la pénétration brutale d'un adulte, soit par des objets contondants, soit par des produits chimiques, comment me taire quand depuis 15 ans, nous voyons ce que même un oeil de chirurgiens ne peut s'habituer à voir, c'était il y a eu tant la France ne peut pas, ne doit pas détourner le regard et la France ne peut pas se taire. La parole est à notre collègue Michel qui en avait pour le groupe de l'Union, santé. Merci monsieur le président, madame la première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, la France est un grand pays maritime et nous souhaitons qu'elle le demeure à l'approche en fin de semaine des quatrièmes rencontres du transmanche à Saint-Malo et avant les Assises de l'économie de la mer, la semaine prochaine à Lille, je souhaite interroger le gouvernement sur les conditions de concurrence sur le transport maritime dans le transmanche et aussi il faut le dire, en Méditerranée, effectivement, les armateurs sont affrontés à des conditions de concurrence qui ne sont plus égales puisque un certain nombre d'opérateurs utilisent de la main-d'oeuvre à bas coût qui n'est pas européenne pour assurer les liaisons ceci n'est pas acceptable, parce que les conditions salariales imposées ne sont pas respectés, parce que les temps de travail ne sont pas respectées non plus donc il importe effectivement que je que ces conditions de concurrence puisse être restaurée, c'est pourquoi je souhaite demander ce que le gouvernement compte faire pour essayer de d'assainir la situation. Pour nous répondrons la parole. Au secrétaire d'État en charge de la mer Monsieur Hervé Berville. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur qu'veut merci de de votre question qui permet extérieure qui est plus large que la question des ferries du transmanche, qui est celle, au fond du modèle social pour notre économie maritime doit demeurer une puissance maritime importante et doit l'être dans le cadre de ces valeurs de son identité également du renforcement du modèle social, vous l'avez évoqué une entreprise piano a brutalement licencié 800 personnes par Visio cet été, c'est inacceptable, c'est révoltant et depuis le mois de juillet, nous entretenons des relations bien évidemment avec le gouvernement anglais mais aussi avec toutes les partenaires de l'Union européenne pour faire face à une situation et trouver des solutions et donc sous l'autorité de la Première ministre et aussi du président de la République, nous faisons de la lutte conte dumping social une priorité de ce gouvernement et donc cet été, j'ai rencontré notamment Jean-Marc Roué de l'entreprise bris d'indifférence mais aussi la CFE-CGC, la CFDT, la CGT, au fond, on a fait la semaine dernière une réunion Armateurs de France inédite entre les organisations syndicales, patronales et le gouvernement pour avancer très concrètement sur le sujet avec 3 orientations d'abord nous allons et je vous l'annonce : renforcer les contrôles dans le transmanche pour hé bien démontrer notre exigence pour la protection sociale de nos marins, deuxièmement en août, une mission de l'Inspection des affaires maritimes pour mettre sur la table toutes les options d'ici Noël, notamment la loi de police qui interdirait l'accès depuis un port le départ ou l'arrivée d'un port français à tous les navires qui ne respecteraient pas des mesures sociales élevées, et puis vous l'avez indiqué c'est un enjeu aussi, pas simplement pour le transmanche, mais pour la Méditerranée et au fond aussi pour toutes les activités maritimes et donc très concrètement dans le projet de loi de d'accélération des énergies marines renouvelables nous avons étendu là aussi un dispositif pour renforcer, hé bien des mesures sociales, renforcer le modèle social pour les questions liées aux énergies marines renouvelables vous le voyez, le gouvernement a pris conscience de ces enjeux, et je salue tous les députés et sénateurs qui se battent sur ce sujet aussi, et j'aurais très prochainement une discussion avec mon homologue anglais quand il sera définitivement installé pour à la fois renforcer les contrôles et à voir, hé bien une politique bilatéral qui nous permettent de lutter contres ces pratiques déloyales et inacceptable, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre de orientation effectivement à sont importantes parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de mettre plus d'argent sur les entreprises, mais bien de faire en sorte que que les conditions de concurrence soient respectées, et c'est bien et je l'apprécie ce que vous avez proposé à l'instant donc il apporte effectivement qu'on puisse à la fois convaincre les autorités britanniques pour ce qui concerne transmanche et espagnoles, italiennes, pour ce qui concerne la Méditerranée notamment à ce que nous soyons aussi exigeant pour ceux qui viennent dans nos ports que nous exigeons des entreprises de notre pays, il envoie bien sûr de l'avenir, notamment de la Brittany Ferries, ce qui est le premier amateur employant des marins en France et nous souhaitons que le modèle maritime français plus pour plus persévérer, il est important que demain la France, qui est un grand palais maritime comme je le disais tout à l'heure, puisse continuer à l'être et nous comptons sur vous Monsieur le Ministre pour cela. Merci, la parole est au président Jean-François Rapin pour le groupe. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la guerre entre la France et l'Allemagne redevient possible c'est moi interpelle, ils ne sont pas de moi mais de Jacques Attali, qui titrait ainsi sa tribune dans Les Échos au lendemain même de la rencontre à Paris entre messieurs Scholz et Macron pourtant qualifiée de constructive, elle ne l'était en tout cas pas assez pour déboucher, ne serait-ce que sur une déclaration commune à la presse qu'est-il sorti de cette rencontre, des groupes de travail, pas de quoi nous rassurer, Monsieur le Ministre, la guerre en Ukraine signifie un changement d'époque, mais l'Allemagne continue de jouer cavalier seul, elle sort du chapeau 200 milliards pour amortir la crise énergétique refuse notre demande de plafonnement européen du prix du gaz choisi SpaceX pour lancer ses satellites achète des équipements militaires américains sans égard pour nos projets communs de chars et d'avions de combat lance un bouclier antimissile européen sans la France se rend seul après-demain à Pékin, à qui elle vend le port d'Hambourg, monsieur le Ministre, vous nous devez la vérité. La confiance est-elle en perd avec l'Allemagne. Pour vous répondre, la parole est au Ministre délégué chargé du commerce extérieur, vous avez la parole monsieur le Ministre. Regardez. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Rapin, le couple franco-allemand a été à la fondation même des communautés européennes et il est depuis lors un moteur essentiel l'entretien entre le président de la République et le chancelier Scholz à Paris, mercredi dernier, a permis de réaffirmer une ambition commune et de définir une méthode de travail pour les prochaines semaines, la France et l'Allemagne sont convenus de rechercher dans tous les domaines, dans tous les domaines des perspectives communes face aux défis de notre temps, plusieurs chantiers, plusieurs chantiers ont été lancés la mise en place d'un fonds franco- allemand pour l'innovation, la rénovation des structures du partenariat franco-allemand ou encore la constitution d'un réseau entre les futures élites de nos 2 pays, nous allons approfondir le dialogue franco-allemand, en particulier sur l'énergie, la défense et le spatial, ou encore l'impact de la politique économique américaine sur l'Europe, notamment l'Insee Addiction acte nous avons travaillé tout lui était extrêmement bien, lors du conseil, commerce à Prague avec nos amis allemands, cette nouvelle approche nécessitera un travail important du gouvernement qui se matérialisera, nous l'espérons, dès le conseil des ministres franco-allemand prévu autour du 60ème anniversaire du traité de l'Élysée en janvier prochain, pour sa part la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna travaillera étroitement avec mesdames annéelà barbec qu'elle rencontra dans le cas du G7 en Allemagne à Munster puis le recevra plus longuement à Paris fin novembre, nous souhaitons définir les axes de travail pour agir en franco-allemand sur les sujets suivants : l'Ukraine et en particulier sa reconstruction à court et à long terme, le renforcement de l'autonomie stratégique qui a de lieux ou encore l'Afrique notamment notre présence au Sahel, vous le voyez, le couple franco-allemand demeure solide, il travaille en confiance et il est bien décidé à agir ensemble pour relever les défis de notre temps, je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez parlé de couples, j'ai parlé simplement de relation, la construction européenne s'est fait après-guerre grâce à la convergence d'intérêts entre une Allemagne qui cherchait la rédemption et une France qui voulait incarner sa puissance, les temps ont changé : l'Allemagne ne s'excusent plus, elle s'affirme et la France est à sa remorque déjà distancé en matière économique, notre pays risque à présent le déclassement diplomatique tout ceci parce que l'élargissement de l'Union Européenne va recentrer géopolitiquement l'Allemagne au centre de l'Europe est-elle capable, l'Allemagne aujourd'hui de mieux articuler ses intérêts propres, avec l'intérêt stratégique supérieure, que nos 2 pays partagent une Europe de la paix et de la liberté. La parole est à notre collègue Sébastien Pla pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. la souveraineté énergétique française est mise à mal la piste des énergies décarbonnées produites localement et la diversification des approvisionnements apparaît comme une solution d'avenir, l'hydrogène est une piste sérieuse qui présente de nombreux atouts, notamment celui de décarboner les activités industrielles et les mobilités, le plan d'action riz Power insiste sur la nécessité de créer un réseau de distribution à l'échelle européenne, cette dorsale concerne 21 pays et viserait à interconnecter les centres de production, régionaux et nationaux pour se prémunir de la dépendance au gaz russe, il permettra d'alimenter les usagers industriels parmi lesquels le 1er robe d'hydrogène Vert et d'éolien Offshore à pour la maillon essentiel de la transition énergétique en Méditerranée occidentale, porté par la région Occitanie et fortement par l'Europe, l'État et la BPI c'est dans ce contexte, avec la plus grande surprise que nous avons appris dans la presse, la naissance d'un nouveau projet de gazoduc sous-marin entre Barcelone et Fos-sur-Mer, baptisé barre, marre, ne peut ignorer et balayé d'un revers de main la stratégie de développement en Occitanie d'une filière industrielle de massification de production et d'énergie d'hydrogène décarboné déjà en phase opérationnelle, si le projet Barnard va dans le bon sens, nous n'avons aucune information ni sur son impact économique ni écologique, ni sur la stratégie énergétique visée, contrairement au projet initial, Mike Catt qui relie les centres de production régionaux et ici que les utilisateurs industriels de Bordeaux à Marseille, madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que lors du prochain sommet européen d'Alicante Les 8 et 9 décembre la région Occitanie aura confirmation qu'elle sera bien connectée au projet barbare via le pôle industriel de pour la nouvelle. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la transition énergétique, madame Pannier-Runacher. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, plat, d'abord je veux vous dire l'engagement de la France pour soutenir une filière hydrogène bas-carbone vous le savez, c'est un des grands axes de notre politique industrielle et de notre politique énergétique puisque nous investissons 9 milliards d'euros dans cette politique, au travers notamment du plan France 2030 9 milliards pour faire émerger toutes les briques technologiques de la filière hydrogène bas-carbone électrolyseurs pile à combustible, solutions de stockage et notamment pour porter un projet à Port la Nouvelle de production d'hydrogène décarboné pour la filière transport et également un projet qui va permettre de décarboner nos industries et d'accompagner les collectivités locales qui en feront à levier de décarbonation je pense au projet de l'agglomération de Dijon par exemple pour les transports en commun ou aux trains à hydrogène Vert que porte plusieurs régions dont la vôtre, celle d'Occitanie, pour revenir à la question que vous posez, ce que nous avons ce que le président de la République a décidé avec ses homologues portugais et espagnols, ces 2 décisions fortes la première décision, c'est de renforcer les interconnexions entre la péninsule idée ibérique et la et la France en matière d'électricité car c'est le 1er levier pour faciliter la production d'hydrogène sur base bas-carbone et c'est ce que nous allons en faire la 2ème décision, c'est effectivement de constater la difficulté à mener à son terme le projet quatre et de le remplacer par une solution sous-marine qui relierait Barcelone à Marseille pour en faire une infrastructure hydrogène cette infrastructure, elle viendra en support des autres infrastructures hydrogène que nous allons devoir développer pour porter nos ambitions hydrogène mais je veux vous rassurer ici l'Occitanie, a pris des engagements en matière d'hydrogène Vert qui sont forts et nous allons continuer à l'accompagner, parce que ce sont des solutions créatrices d'emplois parce que nous avons besoin, mais les misère sur notre territoire et parce que nous souhaitons faire de la France, un des leaders mondiaux de l'hydrogène Madame la Ministre ce ce n'est pas les moyens effectivement 8 milliards d'euros, vous l'avez dit, sur des moyens colossaux pour l'industrie, l'hydrogène décarboné c'est la méthode qui interroge pour pour la bonne et simple raison que le projet Barnard sort du chapeau et vous l'avez dit, c'est une décision du président de la République, directement, avec ces mots homologues espagnols et portugais, sans aucune concertation localement avec les acteurs qui portent des mythes quatre dans les acteurs industriels et les élus, il y a encore moins la DGEC qui était pas au courant de ce projet-là, donc il y a réellement un problème de méthode cela dit merci beaucoup au à l'ancien 1er ministre qui a mis énormément d'argent sur le projet de pour la nouvelle de projet industriel

La parole est maintenant notre collègue Philippe Tabarot pour le groupe Les Républicains. demander à monsieur le ministre délégué aux Transports de cesser de laisser entendre, comme il l'a fait, mercredi dernier, dans cet hémicycle que vous allez investir 12 milliards cette année dans le réseau ferroviaire car c'est faux et pour vous paraphraser c'est ça l'esbroufe, à la différence des moyens supplémentaires votée par le Parlement, nous sommes au dernier rang européen avec la Lituanie concernant la modernisation de notre réseau, nos lignes ferroviaires vont être ralentis ou les unes après les autres, faute d'investissements, si vous ne réagissez pas fortement pour cela écoutez plus souvent les appels du Sénat comme sur la question des ZFU zones à faibles émissions, nous avions proposé lors de l'examen de la loi climat et résilience, un certain nombre de mesures pour obtenir l'adhésion de nos concitoyens, car oui, il y a urgence à décarboner nos transports pour cause de santé publique, mais pour faire accepter une réforme qui va impacter d'ici à 2 ans près de 40 % du parc automobile et donc des Français, il faut informer, écouter, accompagner ce qui n'avait pas été fait jusqu'à, enfin, la semaine dernière devant les 43 présidents d'agglomérations concernées, vous avez repris quelques propositions du Sénat rejetée à l'époque par la ministre Pompili comme le prêt à taux la révision du schéma de restrictions et l'idée effectivité des contrôles mais le préalable à tout ça demeure un développement massif de l'offre de transports en commun de la France périphérique vers nos agglomérations pour réduire cette fracture qui mine notre pays, monsieur le Ministre, à défaut de freinage d'urgence ou de rétropédalage n'est-il pas temps avec pragmatisme de revoir l'ensemble du dispositif des zones à faibles émissions. émissions. On ne la parole est au ministre de la transition écologique et de la cohésion des. Territoire Monsieur Béchu. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Philippe Tabarot. D'abord, je vais m'beaucoup de de joie et de précision à vous répondre sur la 2ème partie de la question, j'ai trouvé que l'introduction était d'autant plus abrupt que immérité pour travailler avec Clément Beaune je peux vous assurer que il est pas dans l'esbroufe et ce à quoi nous travaillons dans le cadre de la planification écologique, c'est précisément à vous présenter des investissements massifs, avec, je le dis, une méthode, c'est d'abord d'avoir le rapport du c'est oui c'est oui, auquel vous appartenez, qu'il a pris soin d'auditionner tous les territoires, pour qu'on ait une remontée des besoins qui permettent ensuite de déterminer la feuille de route et pas de mettre l'argent avant de commencer par se mettent d'accord sur les sujets, c'était l'esprit de la l'homme hein, ça doit être la méthode pour le pour En ce qui concerne les et des feux, vous avez raison sur le fait qu'il y a 2 impératifs. Extraordinairement important, le premier, personne ne le conteste. En tout cas, je veux dire ici. Nous ne pouvons pas continuer à regarder les morts de la pollution atmosphérique sans réagir. Et même si Santé publique France l'ensemble des éléments dont nous disposons permettent de mesurer qu'il y a une amélioration de la qualité de l'air 47000 morts en 2021 liée aux particules fines ou dioxyde d'azote, ça nécessite de donner aux élus de proximité, les moyens pour agir. Mais à côté, si on mène une politique écologique si on mène une politique pour lutter contre le réchauffement climatique qui se fait contrôler plus fragiles, on perdra leur adhésion et on transformera une cause juste en une nouvelle levée de boucliers des uns contre les autres et on fera de l'écologie, un combat ou une guerre au lieu d'en faire un chemin et quelque chose de désirable c'est exactement notre ambition un comité ministériel tous les 6 mois pour les retours d'expérience, l'ouverture d'un travail spécifique sur l'accessibilité sociale la réflexion mesures d'accompagnement, les premiers moyens dans le cadre du fonds vers la réflexion sur des dispositifs un peu sur le modèle de Strasbourg qui permettrait à des voitures même qui ne sont pas dans les bons critères d'accéder à un certain nombre de fois dans le centre-ville, une intensification des primes avec l'abandon de la réciprocité sur la surprime ZF, une campagne de communication nationale l'année prochaine, autant de sujets ou 100 détricoter l'ambition, on pourra effectivement faire en sorte de travailler ensemble à améliorer le dispositif. Monsieur le Ministre, n'oubliez pas également de redonner la main aux élus locaux, sinon vous ZFE vont se transformer en zone à forte exclusion merci. La parole est à notre collègue Stéphane Le Rudulier pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Merci, merci Monsieur le Président. Madame la ministre de la culture, le monde de de la culture et est en émoi est en effervescence après la nomination par le président Macron de Pierre-Olivier Costa à la tête du musée marseillais le Mucem en effet plusieurs haut fonctionnaire spécialiste de l'art et de la culture ont dénoncé cette nomination, qui selon eux est du pur copinage copinage monsieur Pierre Olivier Costa, ancien directeur de cabinet de Madame Brigitte Macron, ancien chef de cabinet du président de la République ne répondrait pas aux qualifications nécessaires pour ce poste, alors Madame la ministre, ma question est simple, quels ont été les critères de sélection retenue pour asseoir la nomination de Pierre-Olivier Costa à ce poste. Costa à ce poste. La parole est au porte-parole du gouvernement Monsieur Olivier Véran. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Le Rudulier excusez le, l'absence de Madame la Ministre de la culture, elle est actuellement au cours de à l'A6 à la commémoration en l'hommage de, de, de Monsieur Soulages, vous m'interrogez sur la nomination de Pierre-Olivier Costa à la tête du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le fameux Le fabuleux Mucem marseillais d'abord sur les procédures de nomination, il n'y a pas eu d'appel à candidature, ce qui n'est pas une exception, monsieur le sénateur, ils ne sont en effet pas systématique du tout pour ce type de poste et pour une bonne raison, beaucoup de candidats souhaitent garder la confidentialité sur leur candidature car elle se trouve être eux-mêmes au moment où une candidate pour un poste à la tête de lieux de prestige en matière culturelle, c'était le cas par exemple pour le musée du Louvre, c'était le cas également pour le Théâtre national de Strasbourg, en revanche, la ministre de la Culture confirme qu'elle a reçu plusieurs candidats qui avaient manifesté leur intérêt pour le Mucem sur le profil maintenant de Monsieur Pierre Olivier Costa sa légitimité pour ce poste et est reconnue parce qu'il a exercé une grande partie sa carrière dans le secteur culturel, il a participé au lancement du journal des arts, il a eu diverses responsabilités au sein de la Réunion des musées nationaux, il a travaillé au sein au Centre Pompidou, au Centre national du cinéma avant de rejoindre à la Ville de Paris et la présidence de la République Monsieur Pierre-Olivier Costa à 54 ans ne limitait pas vos commentaires au 5 dernières années de sa carrière professionnelle, alors qu'il a dédié la quasi-totalité de sa vie professionnelle au monde de la culture, son parcours montre sa connaissance fine des enjeux et du fonctionnement interne des institutions que culturels des collectivités et de l'État, il a donc toutes les qualités pour porter une vision stratégique et insuffler une nouvelle dynamique au Mucem le projet qu'il porte pour le Mucem est apparu comme le plus solide et le plus innovant pour renforcer l'ancrage territorial du musée, ses relations avec les acteurs de la région, sa politique éducative mais aussi ouvrir de nouveaux de nouveaux champs d'action avec le nom de la santé ou sur les enjeux de la biodiversité. Monsieur le Rudulier. Merci messieurs Ministre mais je crains fort que vous n'ayez pas compris le sens profond de ma question car clairement, il s'agissait de nous dire, hein, où s'arrête la compétence et où commence la récompense la récompense car au-delà du du choix et vous l'avez souligné de la personne vos méthodes interpelle aucune publication de vacance de postes, aucune publication d'appel à candidature, à la suite de la décision de départ de du prédécesseur de Monsieur Costa je voudrais simplement vous faire un parallèle avec Monsieur Castanet, qui est pressenti pour diriger le grand port autonome de Marseille, rappelez-vous de de l'ancien monde, rappelez-vous, Jean-Christophe Mitterrand qui, en 1986 a été nommé par son père aux Affaires africaines parce qu'il aimait les voyages, j'ose espérer que Monsieur Castanet, n'est pas pressenti, parce qu'il l'aime les effluves du Vieux Port, ou encore mieux les Guez l'odeur des merguez de syndical qui s'est propagée dès l'annonce

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au gouvernement. Les prochaines auront lieu mercredi 9 novembre à 15 heures la séance va être suspendu, elle sera reprise à 16 heures 30 pour l'examen du projet de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027, la séance est suspendue.

Chers collègues, messieurs les Ministres, la séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi rejeté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 dans la discussion générale, la parole est à monsieur Bruno Lemaire, ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Merci madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Ministre, cher Gabriel Attal mesdames et messieurs les sénateurs. Je m'exprime devant vous, dans un contexte économique difficile. Marqué par de fortes incertitudes. Des incertitudes géopolitiques d'abord lié à la guerre en en Ukraine. Les incertitudes fortes. Lié à la politique protectionniste de certains de nos partenaires, je pense à la Chine. Je pense aux États-Unis avec l'inflation acte. Qui aujourd'hui pèsent sur nos industries sur nos implantations industrielles. Les incertitudes liées également à la forte volatilité des prix du gaz qui, après avoir été multiplié par 5 ou 10 ans, a baissé de près de 50 % en quelques semaines. Mais ce qui touche évidemment le plus nos compatriotes. Avant ces incertitudes géopolitiques, c'est l'inflation qui en résultent. L'inflation a atteint des niveaux inédits depuis 40 ans dans l'Union européenne. je voudrais que chacun d'entre nous à travers notre débat prenne conscience de la réalité de l'inflation dans les autres pays européens. 22 pour 100 dans les pays baltes. 17 pour 100 aux Pays-Bas. 11 pour 100 en Allemagne. 6 % d'inflation en France, c'est toujours trop. Mais je rappelle que c'est le chiffre le plus bas de la zone Euro, je rappelle que la France résiste mieux que nos voisins à l'inflation, grâce aux choix stratégiques qui été fait en octobre 2021, de mettre en place un bouclier énergétique sur le gaz et sur l'électricité grâce à ce choix stratégique, la France a aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone où. La France résiste aussi économiquement. Et. Nous avons réalisé 0 2 point de croissance au 3ème trimestre 2022. L'investissement des entreprises a progressé de 2 3 % contre 0 veut que 8 % au 2ème trimestre il continue donc de progresser, notamment dans l'aéronautique, dans l'automobile et dans l'informatique. Je ne sous-estime donc pas les difficultés économiques, mais je ne voudrais pas que nous cédions au pessimisme ou à l'auto-flagellation. Notre économie dépend des circonstances internationales mais pas seulement. Elle dépend aussi de notre détermination de la stabilité des choix de politique économique que nous avons fait depuis près de 6 ans et que je rappellerai tout à l'heure et de notre vision de long terme d'une économie compétitive innovante et décarboner. Dans les circonstances actuelles, notre priorité, celle qui figure dans le projet de loi de finances, c'est de protéger nos compatriotes contre l'inflation et de faire baisser cette inflation pour la ramener dans les meilleurs délais possible à un niveau plus raisonnable. Comment pouvons-nous y parvenir. D'abord, c'est la première nécessité absolue en garantissant la bonne coordination de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Nous ne pouvons pas avoir une politique monétaire restrictive et une politique budgétaire expansionniste, c'est pourquoi nous avons pris la décision, être la première ministre de mettre en place des aides ciblées pour les entreprises contre l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité 10 milliards d'euros d'aide, mais 10 milliards qui sont intégralement financés soit par les 3 milliards du plan de résilience, soit pour les 7 milliards d'euros de recettes supplémentaires du prélèvement sur les rentes infra-marginale des entreprises énergéticien 10 milliards qui sont plafonnés pour ne pas exposer le budget de l'État à la volatilité des prix du marché, c'est une décision protectrice, mais c'est aussi une décision responsable du point de vue des finances publiques pour éviter la divergence entre politique monétaire et politique budgétaire. Même chose au niveau européen on nous devons coordonner nos réponses de politique budgétaire pour garantir des niveaux de soutien comparables face à l'inflation, regardez ce qui s'est passé en Bretagne, qui doit nous servir de leçon à tous, tout n'est pas possible et on peut toujours promettre à nos compatriotes de dépenser 7 8 9 10 % de notre PNB pour lutter contre l'inflation, le résultat, c'est la sanction immédiate des marchés, l'envolée des taux d'intérêt et la nécessité de revenir en arrière. Nous, nous préférons avec le président de la République, aller de l'avant, coordonner nos réponses de politique budgétaire, je rappelle que, aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends trop souvent dire les niveaux de soutien des citoyens et des entreprises en France sont parfaitement comparables à ceux des autres grands pays de la zone Euro de 4 à 5 % du PNB sur la période 2021 2023, c'est cette coordination qui préserve la force notre réponse et qui évite une fragmentation de la zone où. En 2ème lieu. C'est la 2ème nécessité, ce n'est pas la plus simple à faire comprendre. Et c'est la plus courageuse. Il a plus responsable. C'est éviter la spirale inflationniste qui avait été provoquée dans les années 1970 par une augmentation générale et automatique des salaires totalement découplées de la productivité du travail. C'est très bien de promettre l'indexation des salaires sur l'inflation. Et je sais que beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui. Je souhaiterais avoir des salaires plus élevés. Le président de la République a fermé la porte à cette indexation générale je crois profondément que cette décision est courageuse. Responsable. Et nous évitera bien des déboires demain comme ce que nous avions connu dans les années 1970 car l'indexation générale des salaires sur les prix, sans considération de productivité du travail. Cela conduit à une nouvelle réduction de la marche des entreprises qui, du coup, seraient obligés de répercuter cette perte de marge sur l'augmentation des prix à la consommation, c'est une spirale sans fin d'augmentation des salaires, ah quelle répondent d'augmentation des prix et une nouvelle augmentation des salaires et une nouvelle augmentation des prix, c'est cette spirale inflationniste dans laquelle nous refusons en responsabilité de rentrer. Car nous serions perdants sur tous les tableaux. Nous aurions une inflation hors de contrôle. Alors même que notre objectif stratégique et de revenir à des niveaux raisonnables d'inflation pour protéger les plus modestes et protéger des entreprises les plus fragiles. Nous décroche Orion en terme de compétitivité au moment même où grâce à des efforts constants depuis plusieurs années, nous sommes en train de retrouver notre compétitivité. Enfin nous ruine Riom tous les efforts de réindustrialisation qui ont donné des résultats sur l'emploi, l'attractivité, l'investissement en France depuis 6 ans. Est ce que cela veut dire pour autant. Que nous devrions abandonner l'idée d'une meilleure rémunération du travail certainement pas. Mais faisons la différence entre les promesses démagogiques d'indexation générale des salaires sur les prix et le choix responsable qui est celui de notre majorité, de garantir une meilleure rémunération du travail. Cette meilleure rémunération du travail, elle passe d'abord pour les salaires les plus modestes, par l'indexation qui existe du SMIC, qui je le rappelle, a augmenté de 8 % en un an, les salaires les plus modestes chaud donc protéger contre l'inflation. Au delà, je l'ai dit à de multiples reprises depuis maintenant plus de 3 ans, avant même que l'inflation ne reviennent, les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Elles le font d'ailleurs, quand vous regardez le chiffre très largement depuis plusieurs mois. Il faut par ailleurs continuer à travailler sur ce qui me paraît le vrai débat, le débat juste sur le meilleur partage de la valeur entre capital et travail, c'est ça le véritable débat à l'intéressement quand nous poussons à la participation quand nous supprimons la taxe de 20 % sur l'intéressement quand nous facilitons la conclusion d'un accord d'intéressement pour les plus petites entreprises, quand nous mettons en place une prime défiscalisée à six mille euros quand nous facilitons l'accès à l'actionnariat salarié, qui a fortement augmenté depuis 5 ans, qu'est ce que nous faisons d'autre sinon garantir un meilleur partage de la valeur entre le travail et le capital au profit du travail, voilà le fil rouge de la meilleure rémunération du travail, voilà le vrai fil rouge, la justice sociale par de l'argent distribué gratuitement, mais de l'argent qu'est le fruit du travail. De la production et de la compétitivité retrouvée de nos entreprises, c'est pour cela que je souhaite qu'avec les partenaires sociaux, nous avancions plus rapidement sur notre proposition de dividende salarié, qui doit donner rapidement des résultats concrets, une entreprise qui distribue des résultats à ses actionnaires. Doit aussi distribuer des salaires à ses employés. Voilà le sens de ce dividende salarié qui était proposé par le président de la République et qui est une nouvelle illustration de notre volonté de mieux partager la rémunération du travail et du capital. La troisième réponse de long terme pour lutter contre l'inflation. ça va. Au au-delà de la coordination de la politique monétaire, la politique budgétaire, au delà de la rémunération du travail par un meilleur partage de la valeur, c'est un investissement de long terme dans l'énergie, 100 de l'inflation que nous connaissons aujourd'hui est une inflation importée qui est due à la flambée des prix des énergies fossiles qui représentent, je le rappelle encore 2 tiers de la consommation d'énergie dans notre pays. Si nous voulons réduire l'inflation, il faut renforcer notre indépendance. Et notamment notre indépendance énergétique car ne nous y trompons pas, cette flambée d'inflation en Europe se traduit par un transfert massif de richesses. Des pays européens vers les pays producteurs d'énergies fossiles, nous n'avons pas vocation à financer les pays producteurs d'énergies fossiles, nous avons vocation à investir dans le renouvelable et dans l'énergie nucléaire, c'est exactement ce qu'a proposé et décidé le président de la République, enfin un budget, ce sont aussi des constantes qui font la force d'une politique et c'est constant je voudrais réaffirmer ici, même si je sais que nous aurons dans les jours qui viennent, un vrai débat sur ces sujets. La première de constante, c'est le renforcement de l'appareil productif. Et donc la baisse des impôts. Je connais les doutes qui se sont manifestés dans cette assemblée, nous, nous avons discuté avec un certain nombre de présidents de groupe à l'égard d'une nouvelle baisse des impôts de production. Notamment la suppression en 2 temps de la CVAE après une première baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production qui nous a permis de revenir à près de 2 points d'écart avec l'Allemagne, là où il y en avait trois auparavant. Je sais que les doutes se sont exprimés, je continue à être profondément convaincu de la nécessité d'une nouvelle baisse des impôts de production de 4 milliards en 2023 et 4 milliards en 2024 je voudrais simplement rappeler des faits simple. à l'appui de cette conviction. Quand vous regardez la situation de l'économie française depuis 30 ans. Elle se caractérise, hélas, par le niveau d'impôt le plus élevé de tous les pays de la zone Euro et le niveau d'un des sessions le plus faible de tous les pays de la zone Euro. Eh bien, c'est ce sur quoi je continuerai à me battre, c'est ce contre quoi nous nous battrons avec toute la majorité, inlassablement, la France n'a pas vocation à avoir une industrie faible et des impôts élevés, je préférerais que des impôts. Plus faible et l'industrie plus forte, c'est le sens de cette baisse des impôts, de production, c'est le sens de cette baisse en deux fois de la CVAE qui doit nous permettent de continuer la réindustrialisation du pays, il n'y aura pas de réindustrialisation, avec un écart d'imposition aussi important par rapport à nos grands partenaires européens. certains me disent qu'il est trop tôt pour continuer la baisse des impôts, de production, ce sont à mon avis, les mêmes qui me diront demain que c'est trop tard. On me dit que c'est un cadeau qui est fait aux entreprises, mais ce sont les mêmes qui ensuite viennent pleurer dans mon bureau en disant nos industries ne sont pas suffisamment compétitive, on me dit qu'il faut protéger les collectivités locales, mais ce sont les mêmes qui essayent d'attirer sur leur commune, à juste titre des entreprises industrielles pourvoyeuses d'emplois, de richesse et de prospérité pour leur territoire. Certains me disent : mais vous vous trompez totalement de direction la bonne direction, c'est augmenter des impôts au nom de la justice fiscale. Je tiens à le rappeler que malgré les efforts que nous avons menée avec constance depuis 6 ans avec cette majorité, le président de la République, malgré la baisse de 10 milliards d'euros sur les impôts de production. Malgré la baisse des impôts sur les sociétés qui été ramené de 33 3 à 25 % malgré la baisse de l'impôt sur le revenu, malgré la suppression de la taxe d'habitation, malgré la suppression de la redevance audiovisuelle, malgré une baisse générale de près de 50 milliards d'euros d'impôts au cours des 5 dernières années, nous avons toujours le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé des pays européens. Derrière le Danemark. C'est donc vous dire qu'il nous reste une marge de manoeuvre pour baisser les impôts dans notre pays et être compétitif du point de vue fiscal, je voudrais dire également. à tous les sénateurs aujourd'hui à quel point je suis le 1er, défenseur de la justice fiscale. Mais je souhaite aller chercher de l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire pas dans la poche des Français. Mais chez les gens du numérique qui doivent payer leur taxe sur les activités digitales qui ne rapporte 660 millions d'euros cette année, la France a été la première à mettre en place cette mesure de justice fiscale, aller chercher l'argent où il se trouve, c'est mettre en place la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés pour éviter toute optimisation fiscale si nous n'y arrivons pas, au niveau européen d'ici la fin de l'année, nous le mettrons en place au niveau national. Au début de l'année 2023 et aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est évidemment refusé les rendent des énergéticiens en mettant en place ce prélèvement obligatoire qui va nous rapporter l'année prochaine 26 milliards d'euros, je suis pour la justice fiscale et je ne suis pas pour qu'on augmente les impôts des Français et je considère que les deux sont parfaitement compatibles la 2ème constante de ce budget que rappellera le ministre-les comptes publics, c'est la maîtrise de la dépense publique. Nous avons 2 lois de programmation des finances publiques qui doit nous permettent de revenir sous les 3 % en 2027. Et je viens ici dans cette assemblée de la sagesse, en comptant sur la grande sagesse des sénatrices et des sénateurs. Pour éviter les dérapages à 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires que nous avons connu à l'Assemblée nationale, car ces dérapages de 15 milliards d'euros, témoigne soit d'une indifférence totale à la bonne tenue des finances de la nation. Soit ce que je ne peux croire une indifférence totale à la vie de nos compatriotes, car je rappelle que c'est 15 milliards d'euros ont été gagés sur le bouclier électricité que nous avons mis en place et 15 milliards d'euros s'ils étaient financées par la suppression d'une partie du bouclier énergétique signifierait une augmentation de 40 % du prix de l'électricité, une hausse de la facture de près de 600 euros par an en moyenne sur les ménages français. Ni l'indifférence à la bonne tenue des finances de la nation, ni l'indifférence à la vie quotidienne de nos compatriotes ne sont acceptables et ne correspondent aux orientations notre majorité enfin la 3ème notre politique budgétaire, c'est notre engagement européen. De ce point de vue, je compte sur les sénatrices et les sénateurs pour que nous trouvions ensemble un accord sur la loi de programmation des finances publiques, je pense qu'il est bon pour la nation française d'avoir de la visibilité sur nos finances publiques à 5 ans, je pense qu'il est bon pour nos partenaires européens, de savoir que les finances publiques de la France, la 2ème économie de la zone Euro sont bien tenus, je pense qu'il est bon de prendre des engagements. En terme de réformes de structure sur l'assurance chômage ou sur les retraites, je pense qu'il est rassurant pour nos compatriotes rassurant pour les entrepreneurs, de se dire : mais voilà où nous allons, voilà quand va commencer la baisse, la dette publique, voilà quand nous retrouverons les 3 % de déficit public et la seule garantie législative que nous ayons de donner de la visibilité à nos contacts. Sur les finances publiques, c'est la loi de programmation des finances publiques, votre proposition consiste à aligner la baisse des dépenses publiques de l'État sur celle des collectivités locales, moins 0 virgule cinq en volume, je pense que c'est une proposition qui est juste et qui s'entend, et qui est honnête. Vous avez proposé pour cela 37 milliards d'euros de réduction des dépenses, nous allons dire que cet ambitieux, très ambitieux, mais je suis certain en tout cas que notre travail en commun doit nous permettent de faire émerger des propositions réalistes et concrètes et je l'espère, de trouver un compromis sur cette loi de programmation des finances publiques dont je persiste à penser qu'elle est rassurante pour nos compatriotes rassurante pour nos partenaires européens et responsable du strict point de vue de la bonne tenue de nos finances publiques, je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le Ministre, Cher Bruno Lemaire, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis pour examiner le projet de loi de programmation des finances publiques qui, le 25 octobre dernier a été rejeté par l'Assemblée nationale ce jour là, j'ai pris acte du choix souverain des députés, mais je n'ai pu m'empêcher d'exprimer une conviction que je veux partager avec vous aujourd'hui, nous pouvons avoir des désaccords, il est d'ailleurs normal sain que les groupes politiques n'est pas la même analyse de ce qu'il convient de faire pour les 5 prochaines années, oui, nous pouvons avoir des désaccords sur l'évolution des dépenses ou sur la manière dont les collectivités territoriales, contribue à l'effort de maîtrise, j'ai bien vu qu'un certain nombre d'amendements avaient été adoptés sur ce point, en commission des finances, il me semble que laisser notre pays sans cadre et sans trajectoire écornerait profondément sa crédibilité, notamment vis-à-vis de nos partenaires européens, ce n'est ni une menace ni un épouvantail, c'est simplement le rappel d'un principe de réalité, principe de réalité et même principe de bon sens qui peut croire que notre pays se porterait mieux parce que nous aurions décidé d'avancer sans balises ou sans point de repère qui peut croire que le rejet du sérieux budgétaire est une réponse aux problèmes que nous devons résoudre : qui peut croire que notre pays serait plus fort ou plus libre, hein, parce qu'il aurait renoncé à la maîtrise de ses finances publiques à plus forte raison dans le contexte que nous connaissons, marqué à la fois par la hausse des prix et par la hausse des taux. La réalité, la responsabilité, le bon sens votre assemblée, on a à nouveau fait preuve en adoptant, jeudi dernier en commission des finances, hein, une loi de programmation des finances publiques, sur laquelle nous sommes saisis aujourd'hui, je vois qu'une question préalable a été déposée par le groupe CRCE, je forme le souhait qu'elle ne soit pas adopté puisque, je le dis, nous avons besoin de ce cadre pour les années à venir, c'est un enjeu de crédibilité, pour notre pays, et contrairement à ce que j'ai pu entendre ce projet de loi de programmation n'est pas un carcan mais un cadre, c'est un cadre qui rappelle les objectifs que nous avons fixé les engagements que nous avons pris durant les Français devant la campagne présidentielle, ces engagements sont clairs : ramener le déficit public sous la barre des 3 % d'ici la fin du quinquennat et stabiliser notre endettement public à partir de 2026 cette trajectoire et crédible, elle est d'autant plus crédible qu'elle est déjà engagé, le déficit était, je le rappelle, de 9 % en 2020, nous l'avons descendu à 6 5 % en 2021 il sera cette année de 4 virgule 9 % 01 points de mieux que la Berd prévisions réalisées en juillet dernier, j'aurai l'occasion d'y revenir demain puisque je serai auditionné par votre commission des finances sur le 2ème projet de loi de finances rectificative pour 2022 cette trajectoire est déjà engagée et cette trajectoire ne peut être différé en tant que ministre des Comptes publics, j'ai le devoir de rappeler que l'effort de maîtrise de nos comptes ne peut pas être remis à plus tard, quand un pays comptabilise plus de 3000 milliards d'euros de dette, plus tard, c'est trop tard, quand les taux d'intérêts remontent plus tard, c'est trop tard, quand la charge de la dette augmente, elle sera de 51 milliards d'euros l'année prochaine, plus tard, c'est trop tard, alors oui nous devons poursuivre l'effort de maîtrise des dépenses publiques, il ne s'agit pas de mettre en oeuvre un plan programme d'austérité, mais simplement d'éviter le dérapage et de se fixer un cadre d'évolution de la dépense, j'ai bien conscience que la majorité souhaite sénatoriale souhaite que nous allions plus loin en ce qui concerne la maîtrise des dépenses de l'État, à cet égard des amendements ont été présentés, adopté en commission des finances sur les articles 2 3 et 4 pour que l'effort fait par les administrations centrales sur les dépenses soient alignés à celui proposé pour les collectivités locales, c'est-à-dire une baisse annuelle de 0 5 % en volume, Bruno Lemaire là dit il y a un instant, nous sommes ouverts effectivement à ce que il y est parité dans l'effort, puisqu'il était prévu un effort de 04 % pour l'état et de 0 5 % pour les collectivités locales, vous avez également proposé adopté un amendement qui exclut une grande partie des dépenses de l'État, prises en compte pour la maîtrise des dépenses publiques, il s'agit d'un agrégat qui exclut la charge de la dette, ainsi que toutes les mesures de soutien, notamment économique et sanitaire, bien entendu, nous sommes ici pour discuter de la trajectoire, c'est même l'objet de ce débat, je veux simplement préciser et Bruno Lemaire l'a rappelé il y a un instant, que cela représenterait une baisse des dépenses supplémentaires par rapport aux économies déjà prévues, de l'Ordre de 37 milliards d'euros à horizon 2027 par rapport à la trajectoire que nous avons présenté ce qui ramènerait le solde de fin de quinquennat de de neuf selon la trajectoire que nous proposons à 1 virgule 7 % nous aurons ce débat dans un instant et tout au long de la soirée, mais permettez-moi juste de dire qu'un tel ajustements. Doit pouvoir être atteint de manière crédible. 37 milliards d'euros à trouver d'ici à 2027 25 milliards d'euros à trouver d'ici à 2025 il y a un article dans cette loi de programmation, je crois que c'est l'article 12 qui prévoit l'évolution des dépenses pour les grandes missions budgétaires de l'État dans les 3 années à venir, par cohérence si votre assemblée décidait de baisser ou un effort supplémentaire d'économies de 25 milliards d'euros à horizon 2025 cet article devrait également être pour dire où c'est où, c'est 25 milliards d'euros serait pris et ce qui serait prise sur la défense je l'éducation nationale. Sur la transition écologique ne pouvons avoir ce débat, mais 25 milliards d'euros à trouver en plus d'ici à 2025, c'est une somme d'économies importantes mais Bruno Lemaire là dit nous sommes toujours ouverts à faire davantage d'économies, a montré que nous faisons davantage d'efforts, s'agissant de l'État et nous aurons le débat, le gouvernement a déposé, je les défendrai des articles et des amendements pour rétablir les articles 2 3 et 4 dans leur version originale puisque nous pensons que la trajectoire qui figure dans cette loi de programmation des finances publiques permet une maîtrise de la progression des dépenses, mais le fait dans un cadre soutenable. Une politique austéritaire trop brutal qui sabreur est dans les services publics dans les toutes prochaines années, aurait un impact très difficile dans la vie quotidienne des Français, et probablement dans la conduite de la nation et donc dans l'activité économique au cours de ce débat, nous ferons preuve d'ouverture sur le rehaussement donc de la trajectoire que nous proposons, elle n'a rien d'intangible et Bruno Lemaire là dit nous chercherons toujours à trouver un compromis dans les différentes étapes de l'examen de ce texte mais nous ne pouvons pas adhérer à un objectif qui nous semble totalement inatteignable, sauf à faire des choix qui serait dommageable pour nos services publics ou qui reviendrait à pratiquer une forme d'austérité, je le disais il y a une minute, nous proposons le sérieux, nous ne voulons ni de la gabegie, ni de l'austérité, j'en reviens donc à la conviction que je veux partager avec vous aujourd'hui ce projet de loi de programmation des finances publiques est un élément central de notre crédibilité, pas seulement celle du gouvernement mais aussi celle de la France, crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens puisque nous traduisons dans ce texte, les objectifs fixés dans le programme de stabilité que je vous avez présenté début août crédibilité vis-à-vis des investisseurs, les agences de notation, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt en France comme chez nos voisins, là dessus, il faut que chacun mesure que nous avons changé d'époque, il y a encore seulement un an, nous en train de Sion a tenu le désormais le taux d'intérêt sur les OAT à 10 ans aussi entre 2 5 et 3 la crédibilité de notre pays, sa capacité à honorer ses engagements, je sais que vous y êtes tout autant attaché que nous le sommes, donc jamais je n'emploierais cet argument comme une parade comme une manière d'esquiver le débat pour laisser entendre qu'il faudrait accepter un texte sans modification, je sais bien que nous avons des points de désaccord et notamment à des accords importants sur la manière dont les collectivités territoriales doivent contribuer à l'effort de maîtrise je n'esquive pas ce débat et j'y reviendrai dans un instant, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que la discussion qui démarre aujourd'hui doit nous permettent de doter la France d'une loi de programmation, c'est notre responsabilité et c'est notre devoir, car la situation inverse aurait pour seul effet d'affaiblir le pays la 2ème conviction que je veux partager avec vous, c'est que cette trajectoire des finances publiques est aussi un contrat que le gouvernement passe avec le Parlement, et donc avec les Français qui sont représentés, être un deux doit être un texte pour le Parlement, pour partager un cap pour mieux piloter les finances publiques pour s'assurer que les lois de finance annuelles s'inscrivent en cohérence avec la trajectoire que le gouvernement propose je veux rappeler d'ailleurs que la nouvelle version de la LOLF issu de la révision dite Woerth Saint-Martin Martin donc d'une initiative parlementaire a renforcer la portée de la loi de programmation pluriannuelle une traduction concrète en est que le gouvernement doit désormais justifier devant le Haut Conseil aux finances publiques les éventuels écarts par rapport à la trajectoire pluriannuelle de la loi de programmation des finances publiques en amont du dépôt du projet de loi de finance de l'année, donc pour dire les choses simplement, il me semblerait un peu baroque que le Parlement après avoir à juste titre, oeuvrer pour renforcer son pouvoir de contrôle se prive d'un important instrument de ce contrôle. Et je dis une chose simple : si l'on veut passer du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, comme nous le souhaitons tous, il faut renforcer la capacité du Parlement, évaluer les dispositifs, je sais que vous partagez ce constat et les travaux que vous avez conduit en commission des finances en témoigne ce texte prévoit, c'est son article 7 le bornage à 4 ans des dépenses fiscales, j'ai noté l'adoption en commission des finances d'un amendement proposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain qui propose de ramener ce bornage à 3 ans, ce texte prévoit, et c'est son article 15 que les créations extension ou prolongation d'un dispositif d'aide aux entreprises, instauré après le 1er janvier 2023 ne sont applicables que pour une durée précisée par le texte qui les instituts dans la limite de 5 ans cet article prévoit aussi la remise systématique d'une évaluation, là encore, il renforce le rôle du Parlement dans sa capacité à contrôler le pilotage des finances publiques par l'État, ce texte prévoit, c'est son article 21 des évaluations de la qualité de la dépense publique, dont les conclusions seront transmises au Parlement au plus tard le premier avril de chaque année, à cet égard un amendement adopté à l'initiative du rapporteur général propose d'introduire un certain nombre de précisions pour renforcer l'information et donc la capacité de contrôle du Parlement. Je le disais, nous ne pouvons différer les ports de l'effort de maîtrise de nos finances publiques y parvenir suppose de partager un même sentiment de responsabilité : responsabilité vis-à-vis de notre pays de sa crédibilité de sa capacité d'action de son indépendance aussi y parvenir suppose aussi de répartir l'effort entre l'ensemble des administrations publiques, l'État et ses opérateurs, la sécurité sociale et les collectivités locales, l'article 23 qui précise les modalités de respect de l'eau de Dell fixé l'article 16 a fait l'objet d'un amendement de suppression lors de l'examen du texte en commission des finances, cet amendement de suppression n'a d'ailleurs pas été porté uniquement par le rapporteur général, mais par un certain nombre de groupes d'opposition, j'en prends acte, tout en rappelant que ce mécanisme constitue à mes yeux une solution d'équilibre pour faire en sorte que les collectivités territoriales contribue de façon juste, équitable, équilibrée à l'effort collectif. Vous le savez, les associations d'élus nous ont toutes fait savoir qu'elle ne souhaitait pas la reconduction à l'identique des contrats de Cahors, cette forme de contractualisation avait succédé en 2017 oh baisse massive de DGF et était vécue par beaucoup comme une mise sous tutelle, nous avons donc abandonné, tourner la page des contrats de Cahors et à l'issue d'une très longue concertation avec les associations d'élus que nous avons menée avec mes collègues, Christophe Béchu et Caroline Cayeux, nous avons proposé les pactes de confiance à ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'un glissement sémantique, je leur dis : regardez les déclarations des associations d'élus, je ne dis pas ici, évidemment, que toutes les associations d'élus ont applaudi des 2 mains la mise en place ou la proposition des pactes de confiance, mais un certain nombre d'associations d'élus ont eu des propos. En soutien à la logique qui sous-tendent les les pactes de confiance, je peux citer les représentants des intercommunalités de France qui ont clairement exprimé que le pacte de confiance, tourner la page des contrats de Cahors je peux citer l'association des départements de France et je cite ici un communiqué du président Sauvadet : nous sommes prêts à une participation de tous les départements à la trajectoire en volume et non en valeur avec une réduction de nos dépenses de 0 5 % par rapport au niveau d'inflation, je pense que la solution à laquelle nous sommes parvenus est un effort supportable et tenable dès lors que le gouvernement ne nous met pas de dépenses supplémentaires sur le dos pour être totalement complet, il disait même qu'ils validaient ce dispositif des pactes de confiance dès lors que l'État s'engageait à sortir des dépenses prises en compte les fameuses Hayes, qui sont des dépenses évidemment non pilotables pour les départements et je me suis engagé à l'Assemblée nationale à ce que les Hayes ne figure pas dans les dépenses prises en compte pour le mécanisme de l'article 23, une large majorité, dans cet hémicycle, considère qu'il faut abandonner tout mécanisme de. Prise en compte des dérapages pour corriger une trajectoire de dérapage, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 23 été supprimé en commission là dessus, je vais vous dire notre conviction. Ce dispositif, quand bien même il serait adoptée par le Parlement ne serait probablement pas activée, parce que j'ai vu des associations d'élus des collectivités locales parfaitement consciente et lucide de la situation budgétaire de notre pays parfaitement consciente et lucide, de leur capacité à maîtriser aussi leurs dépenses, mais avoir un cadre qui permet de garantir que lorsque si un dérapage venait à arriver, alors nous regarde aurions pour les 500 plus grandes collectivités de notre pays, on parle des 500 plus grandes collectivités de notre pays, celles qui ont contribué à faire déraper la trajectoire pour voir avec elles, comment revenir vers une trajectoire plus soutenable, c'est une mesure de crédibilité aussi pour la trajectoire que nous fixons vis-à-vis de celles et ceux qui nous regardent. Je ne partage pas, donc l'idée selon laquelle la suppression de cet article 23 serait justifier sa vocation n'est pas de punir ou d'enfants civilisés d'infantiliser l'objectif, c'est de nous donner un cadre et un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement pas pour entraver les collectivités, mais au contraire pour les aider à dégager de la capacité d'autofinancement pour investir oui nous pensons toujours que le mécanisme proposé à l'article 23 et juste et pertinent, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a déposé un amendement pour qu'il soit rétabli, nous aurons donc l'occasion d'en discuter de façon beaucoup plus approfondie voilà Mesdames et messieurs les sénateurs, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous, avant d'entamer l'examen de ce projet de loi de programmation des finances publiques, en somme, nous pouvons avoir des divergences sur les paramètres sur les points de passage ou sur la manière dont chaque catégorie d'administration publique doit contribuer à l'effort collectif. Mais nous devrions tous nous retrouver autour du fait que la 6ème puissance mondiale ne peut pas se dérober à ses obligations de sérieux budgétaire et à en juger les échanges que nous avons d'ores et déjà eu des travaux que vous avez eu en commission des finances, je crois que nous nous retrouverons autour de cet objectif, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à. Présent à notre rapporteur de la commission des fils Jean-François Husson, vous avez dix minutes chers collègues. Madame la présidente, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Nous y voilà : nous examinons aujourd'hui le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027 un exercice important en principe puisqu'il est appelé à définir la trajectoire des finances publiques qui guidera ensuite et loi de finances pour les 5 prochaines années, en outre, ce texte concrétise nos engagements européens au niveau national, toutefois son examen au Sénat intervient dans un contexte un peu différent, a voulu cette année d'une part, les gouvernements du précédent quinquennat n'ont pas jugé utile de modifier la loi de programmation 2018, 2022, laissant ainsi en place une trajectoire totalement décorrélées des événements traversé par notre pays et aux répercussions pourtant majeur sur la trajectoire de nos finances publiques, qu'il s'agisse par exemple du mouvement des Gilets jaunes ou ensuite de la crise sanitaire, économique. Cela a, à mon sens quelque peu écorné la portée de ce texte depuis 2018. D'autre part et surtout, le Sénat est appelé à se prononcer sur le texte déposé par le gouvernement dans la mesure où le projet de loi a été rejeté en première lecture à l'Assemblée nationale, saisi en 1er lieu. Ce contexte étant posé, que penser de cette loi de programmation. S'agissant d'abord du scénario macroéconomique du gouvernement, il est clair que celui-ci repose sur des hypothèses très si ce n'est trop favorable, les prévisions de croissance effective potentiels sont en effet très éloigné du consensus des économistes s'agissant de l'hypothèse de réduction du taux de chômage à 5 % en 2027 je pense, messieurs les ministres qu'il serait bon que le gouvernement ne confondent pas le slogan de campagne avec la rigueur de la prévision d'un scénario macroéconomique, même si je souhaite à notre pays d'atteindre ce résultat, cette situation s'explique notamment sur le fait que le gouvernement surestime dans son projet de loi de programmation les effets à court terme de quelques réformes structurelles qu'souhaitent pourtant engagé. J'en viens maintenant à la trajectoire des finances publiques qui nous est proposé par le gouvernement. Une trajectoire qui n'est pas assez ambitieuse, en prévoyant en effet une réduction du déficit à 3 % du PIB mais seulement à partir de 2027. En effet, nos partenaires européens devraient retrouver ce niveau dès 2025, l'endettement public ne referai quant à lui, pas avant 2000 26 et resterait à des niveaux encore très important, près de 111 % du PIB en 2027, le rythme de redressement de nos comptes publics est insuffisant, il est beaucoup trop long. Cette trajectoire, je le disais, n'est pas à s'ambitieuse, mais elle est aussi en trompe l'oeil, le gouvernement revendique de diminuer la dépense publique en volume entre 2023 et 2027, toutefois il ne retraite ni les mesures liées aux crises sanitaires, économiques, énergétiques, ni la charge de la dette. Et en retenant pour périmètre les seules dépenses ordinaires, les dépenses publiques, enregistre en réalité une progression de 0 6 % en volume. En outre, le gouvernement impose aux administrations locales et sociales de réaliser un effort d'économies compris entre 25 et 27 milliards d'euros, alors que dans le même temps, les administrations centrales ne réalise pas. D'ailleurs, la trajectoire de hausse des crédits des missions budgétaires de l'État, inscrite dans le projet de loi montre que si le gouvernement a choisi les politiques sur lesquels ils souhaitent ajouter des crédits, il a par contre. Renoncer à identifier celles sur lesquelles des économies pourraient être réalisées. élèves des de ces éléments, la commission des finances considère en l'état que la trajectoire du gouvernement n'est pas acceptable d'une part parce qu'elle manque d'ambition en termes de redressement des comptes et de maîtrise de la dépense et, d'autre part parce qu'on demande moins d'efforts à l'État qu'aux administrations publiques. La commission des finances n'a pour autant pas choisi de rejeter ce projet de loi est là pour répondre aux 2 principaux écueils adopter une nouvelle trajectoire de baisse des dépenses plus sérieuse et plus ambitieuse pour retrouver le chemin de l'équilibre. Ainsi, le texte issu de nos travaux prévoit que les dépenses, je le redis, hors mesures de crise et, hors charges de la dette des administrations centrales devront ainsi diminué de 0 5 % en volume chaque année dès 2023, ce qui correspond exactement à ce que le gouvernement demande aux collectivités territoriales, laissant d'ailleurs le soin à ces collectivités de trouver les voies et moyens pour y arriver, cette nouvelle trajectoire permettrait ainsi de ramener le déficit public en dessous de 3 % et dès 2025, ce qui nous paraît être un objectif ambitieux, certes, mais aussi réaliste, cette proposition d'abord et d'ailleurs, répond à 4 objectifs : premièrement, faire refluer le déficit et l'endettement public plus rapidement que ne le prévoit le gouvernement, deuxièmement, et c'est important, assurer la pleine contribution des administrations centrales, troisièmement, préserver nos dépenses sociales et régaliennes et enfin quatrièmement conserver des marges d'intervention face à la crise cette trajectoire impliquerait de réaliser des efforts dès 2023 à hauteur de presque 4 milliards d'euros en l'état actuel du projet de loi de finances. Au cours des années 2023 2027, nous devons donc trouver de nouvelles sources d'économies en mettant en oeuvre des réformes structurelles baisse à long terme des effectifs engagement d'une réforme des retraites ambitieuse réorganisation, pourquoi pas, de certains pu service public comme l'audiovisuel éventuel décalage dans le temps de certaines trajectoires programmatique d'évolution des crédits de certaines politiques publiques non régaliennes, réforme des prestations sociales, nous avons du travail et des possibilités notre commission des finances, a d'ailleurs rendu 109 rapports depuis 2015 riche à eux seuls de mesures qui nourriront nos réflexions. Cette trajectoire repose également sur un parallélisme des exigences pesant sur l'état et les collectivités territoriales, offrant ainsi. Injuste, même s'il est difficile équilibre dans la répartition de l'effort réalisé pour maîtriser la dépense publique entre les administrations, cela nous paraît de bon sens, mais je le dis, cela nous paraît aussi juste, nous ne proposons pas de revenir sur la trajectoire des administrations de Sécurité sociale qui apparaît d'ailleurs déjà relativement ambitieuse au regard des défis qui les attendent pour les prochaines années. S'agissant des collectivités territoriales, ici au Sénat, les efforts qui leur sont demandées dans le projet de loi de programmation telle que déposée par le gouvernement sont conséquents, il faut, il ne faut pas le nier, en prévoyant notamment une trajectoire des concours financiers de l'État, dont la croissance en valeur masque en fait et en réalité une contraction de 4 milliards d'euros en volume. Parallèlement, est également prévu un objectif d'évolution de la dépense locale, le fameux ODEDEL, correspondant, lui, à une diminution des dépenses de fonctionnement de 0 5 % en volume, soit un effort plus rigoureux encore que sous les précédentes lois de programmation. Déjà par le passé, leur contribution au redressement des finances publiques a été déterminante, je veux rappeler ainsi à cet instant qu'entre 2013 et 2016, les collectivités locales ont porté les 2 tiers de la réduction du déficit public alors même qu'elle représentait moins de 20 % de la dépense publique de même elles ont su réaliser 11 milliards d'euros d'économies sur leurs dépenses de fonctionnement entre 2000 19 et 2021 alors même que les contrats de Cahors n'ont pas été appliqué en 2020 et 2021. Les collectivités locales ont donc démontré leur esprit de responsabilité face à la nécessité, et à l'urgence de redresser pour les rétablir nos comptes publics. C'est la raison pour laquelle la commission. à supprimer le système de surveillance et de sanction des collectivités proposée par l'article 23 je vois Monsieur le Ministre, des comptes publics que nous n'avons pas tout à fait la même lecture et en tous les cas pas la même vision des conséquences d'un encadrement soft d'ailleurs vous avez rappelé ou à à l'instant que ça n'était pas forcément nécessaire, hé bien effectivement c'est pas nécessaire qu'y a rien à craindre. Vous verrez, on va s'en occuper dans le débat qui arrive tout à l'heure, il paraît en effet tellement à rebours des engagements du gouvernement à mettre en place une nouvelle méthode fondée sur la confiance dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales. La commission des finances a enrichi le texte, on a de temps plusieurs amendements qui s'inscrivent dans un objectif de maîtrise plus rigoureuse de la dépense. Où sont guidée par un souci de vigilance quant à la mise en oeuvre effective des mesures figurant dans ce texte, en conclusion, c'est ce texte telle qu'issue des travaux de la commission des finances, et complétée des éventuels amendements que nous pourrions retenir au cours des prochaines heures que je vous propose d'adopter, je vous remercie. Merci madame la présidente, messieurs les ministres, messieurs les présidents et rapporteur général de la commission des finances, chers collègues, la commission des affaires sociales a exprimé un réel scepticisme face à la trajectoire financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du Fonds de solidarité vieillesse et de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie contenues dans ce projet de loi, elle a d'ailleurs réitéré ses doutes ce matin même, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, s'agissant de l'Ondam à à l'ont fait, monsieur le Ministre, qui devrait frôler la barre des 250 milliards d'euros dès 2020 soit plus de 5 fois le budget de la Défense, où plus de cinq de 4 fois celui de l'éducation nationale, ça me permet de aussi de de conceptualiser si je puis dire, les sommes en question la trajectoire bien bien que dynamique semble pour le moins ambitieuse et même, pour tout dire, difficilement tenable difficilement tenable, pourquoi, parce que les incertitudes sont grandes sur l'impact financier de la crise sanitaire en 2023 et dans les années ultérieures difficilement tenable car nous voyons bien l'ampleur des besoins de santé l'ampleur des attentes en matière de rénovation de l'hôpital, mais aussi l'ampleur de l'impact financier que représente aujourd'hui le choc d'innovation dans le secteur du médicament difficilement tenable car le contexte inflationniste rend le taux réel de progression bien moindre que celui affiché et sur ce point, si le ministre des Comptes publics considère que l'inflation ne se reproduit pas de manière identique sur les dépenses de santé, force est de constater qu'elle est parfois plus forte encore sur certaines des charges principal des hôpitaux comme l'énergie. Difficilement tenable, enfin et surtout, car le gouvernement comme le directeur de la CNAM, reconnaissent qu'il faudra prendre des mesures fortes d'économie pour garantir le respect de cette trajectoire or quelles seraient ces mesures, nous n'avons obtenu aucune information sur ce point, réglera-t-on enfin l'Ondam de ville et si oui comment ou bien cela signe-t-il le retour explicite d'économies sur l'hôpital, quant au reste des robes s'je ne peux là aussi que regretter le caractère particulièrement lacunaire des informations transmises par le gouvernement pour m'en tenir à l'exemple le plus significatif, l'évolution des dépenses de la branche vieillesse est censée intégrer dès 2023, les effets d'une réforme des retraites, mais nous ne connaissons ni les paramètres, ni même son impact financier, ils ne sont pas précisés dans un quelconque document et malgré mes demandes réitérées, je n'ai pas eu de précision néanmoins du fait du rôle d'une loi de programmation, c'est-à-dire en 1er lieu permettre au Parlement de vérifier chaque année si la trajectoire fixée respecté ou non, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à l'adoption des articles dont elle était saisie se relève, sous réserve de l'adoption de cinq amendements que la commission des finances, et je l'en remercie, a intégré dans le texte qu'elle a établi, outre un amendement de précision à l'article 18 relatif aux charges de gestion des organismes de Sécurité sociale, ces amendements ont pour objet de rendre tout effort sur l'Ondam plus équitable entre les différents acteurs du monde de la santé et d'améliorer également l'information du Parlement sur les finances sociales ainsi à l'article 17 nous avons prolongé la trajectoire des dépenses des robes s'et de l'Ondam jusqu'en 2000 26 et 2027 j'attire votre attention, messieurs les ministres, sur le fait que le compteur des écarts entre les dépenses prévues par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale et celles figurant dans la loi de programmation des finances publiques doit concerner toutes les lois de financement de sécurité sociale jusqu'à l'année 2027 si vous nous dites qu'il y aura une autre loi de programmation avant 2026 je vous invite à compléter le dispositif du Sénat en ajoutant vous- même l'objectif de dépenses des robes s'et du FSB pour 2027 dans le même esprit à l'article vingt-quatre: nous avons souhaité qu'une décomposition des recettes des dépenses et du solde des administrations de Sécurité sociale relatives à l'exercice clos soit adressé au Parlement, au moment du dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale, enfin, messieurs les Ministres, à l'initiative de la commission des affaires sociales, le texte de nos collègues des Finances précise que la mise en réserve de l'Ondam devra concerner de manière égale tous les sous-objectifs en d'autres termes, il nous faudra cesser de faire porter les gels de crédits principalement à l'hôpital, j'espère que nos débats en séance publique nous permettront de confirmer ces avancées, je vous remercie. Merci, cher collègue, et enfin la parole est à Claude Raynal, président de la commission des finances, un président, vous avez 5 minutes. Madame la présidente, messieurs les Ministres, Monsieur le rapporteur général madame la rapporteure générale, mes chers collègues, les lois de programmation des finances publiques, non pas dans notre ordre juridique de caractère contraignant, elles sont néanmoins les marqueurs des débuts de quinquennat en ce qu'elles exposent et les grandes orientations de notre pays en matière de finances publiques, qu'il s'agisse de sa politique fiscale ou de ses priorités budgétaires, elles sont également importantes, vous l'avez dit, à l'égard de nos partenaires de la zone Euro, la précédente loi de programmation 2018, 2022 avait de grandes ambitions : réduire l'endettement public de plus de 5 points de PIB et ramener nos finances publiques, pratiquement à l'équilibre entre temps de nombreux événements sont survenus, qu'il s'agisse du mouvement des Gilets jaunes du Covid est désormais de la crise énergétique et des tensions internationales, chacun sait que ces objectifs donc pas été atteint, aucune révision de la programmation n'a cependant été réalisé comme le réclamaient pourtant le Sénat dès septembre 2019, nous pouvons donc nous ont félicité que le gouvernement présente enfin une nouvelle loi de programmation, même si celle-ci ne débute pas sous les meilleurs auspices son cadrage macroéconomique qui fonde sa crédibilité est entouré de nombreuses incertitudes rappelés par le rapporteur général mais rappeler également par vous, Monsieur le Ministre, le gouvernement apparaît optimiste au regard du consensus des économistes en prévoyant une croisière en croissance moyenne du PIB 6 % sur la période et l'atteinte du plein emploi, même si j'ai eu l'occasion de dire qu'il était dans notre rôle, messieurs les Ministres, de retenir une perspective la moins défavorable possible pour notre pays, sans vous écarter de trop cependant du consensus, ce qui me préoccupe davantage, ce sont les perspectives qui sont dressés pour nos finances publiques, je constate que le gouvernement entend sur la période quinquennale réduire les prélèvements obligatoires de plusieurs milliards d'euros, principalement sur les 2 premières années de programmation 2023 et 2024, poursuivant ainsi sa stratégique qualifié de désarmement fiscal de notre pays après la suppression de la taxe d'habitation dont les conséquences n'ont pas été suffisamment anticipé de toute évidence, le gouvernement s'emploie à finir doté aux collectivités locales, les recettes fiscales dont elle dispose, avec une suppression sur 2 ans de la CVAE sans proposer de mécanismes crédibles de compensation pour ce qui relève des comptes de l'État, le gouverneur de la Banque de France, comme le 1er président de la Cour des comptes, l'ont pourtant dit à multiples reprises, nous n'avons pas les moyens de procéder à de de nouvelles baisses d'impôts, surtout si celles-ci ne sont pas gagées je je note d'ailleurs que, on regarde toujours sur les comparaisons internationales, les entreprises des des sujets par ainsi eau on regarde l'impôt sur les sociétés, on compare, on regarde les impôts de production compare mais par contre sur les niches fiscales en faveur des entreprises, c'est curieux, on fait assez peu de comparaisons internationales, notamment par exemple sur l'Avantage du crédit impôt recherche et ce qu'elle a lieu partout dans les même donc il faut tout regarder, quand on fait une comparaison internationale, il faut la regarder dans son ensemble et donc cette stratégie conduit inévitablement à contraindre toujours plus la dépense publique, même si la trajectoire est vu par certains comme un peu ambitieuse, nul doute que la faiblesse entretenus et volontaire de nos recettes publiques conduira à de nouvelles coupes budgétaires sur des politiques publiques pourtant prioritaires et à mener à bien des réformes dites structurelles visant immanquablement notre modèle social, qu'il s'agisse de réduire l'indemnisation des demandeurs d'emploi ou de rehausser l'âge de départ le risque est réel également de contraindre l'investissement public local alors même que celui-ci est indispensable pour notre transition énergétique et la modernisation de nos infrastructures, par ailleurs, je ne peut que déplorer comme la majorité de mes collègues, la manière d'envisager les relations entre l'État et les collectivités locales et monsieur le ministre des Comptes publics nous avons ne savez pas tout à fait convaincu dans votre vision de l'article 23 car sous la force dehors retour de nouveaux contrats de Cahors, dotée de mécanismes de correction individuelles et d'une possibilité d'exclusion de certaines dotations de l'État fort heureusement notre assemblée je le crois, s'apprête à supprimer ce funeste article 23 en conclusion, si une loi de programmation est nécessaire, je partage cette idée hein, ce qu'elle fixe une trajectoire pluriannuelle pour nos finances publiques, cette trajectoire doit être revu et nos débats devraient permettre à chacun d'exprimer ses priorités, je vous remercie. Merci monsieur le président, monsieur Pascal Savoldelli, les membres du groupe communiste. Ce républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion distribuée sous le numéro 60 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion, la parole est au sénateur Savoldelli pour nous présenter la motion, vous avez dix minutes monsieur le sénateur. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, messieurs les Ministres et mes chers collègues, nous aurions pu avoir ce débat déjà il y a quelques mois. Contact. Avant que vous transmettez à Bruxelles, le programme de stabilité de la France, puisque la copie est exactement la même, la loi de programmation est validé par des instances non élues avant les représentants du pop rassemblés au Parlement et il y a meilleur façon nous semble-t-il, d'associer la nation la trajectoire des finances publiques que nous avons à discuter. Comme à chaque occasion de pareilles circonstances, les travailleurs et les travailleuses ont le droit à un affront supplémentaire. Il faudrait faire la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, car, je cite là qu'on peut raison inopportune du président de la République sur France 2, je le cite : 47 1 % de prélèvements obligatoires, on est au-dessus de tous les voisins européens et ça nous a été re-répété par le ministre-Lemaire, par contre, le président dit aussi, par contre, il y a une chose sur laquelle on est en dessous de tous les voisins c'est ça et là, le voilà qui loue brandit une carte, une carte du nombre d'heures travaillées tout au long d'une vie. Hé ben écoutez, monsieur le président de la République, messieurs les ministres, il y a d'autres cartes 15 virgule un pour de l'emploi salarié temporaire, selon les chiffres de l'OCDE, 10 points de plus que le Royaume-Uni, 5 points de plus que la Grèce 3 7 points de plus que l'Allemagne 13 8 % de l'emploi total est à temps partiel, c'est plus que la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Lituanie, la Croatie, le Portugal, la Pologne et j'en passe, avec 80 virgule 8 % des 25 64 ans en âge de travailler sont au travail. La France et 2 points au-dessus de la moyenne européenne, des pays de l'OCDE et de se l'Union européenne et même selon les heures travaillées par travailleur, la France et devant l'Allemagne devant le Danemark devant le Luxembourg devant les Pays-Bas, la Norvège, l'Islande, l'Autriche et la Suède, enfin un travailleur en France produit 67 dollars par heure travaillée, soit 20 % de plus que la moyenne européenne. Donc ils sont massivement en emploi trop souvent dans des conditions précaires et demeure davantage productifs que nos voisins européens, telle est la vérité économique et social qui devrait servir de base à la programmation des dépenses publiques dans notre pays, la casse sociale entreprise par la réforme de l'assurance chômage et fondé sur des hypothèses irréalistes qui sous-tend ce projet de loi de programmation et là, je cite, le Haut Conseil des finances publiques, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027 repose sur un scénario macroéconomique quasiment identique à celui du programme de stabilité, de 2022 2027 alors même que le Haut conseil avait estimé nécessaire dans son avis du 26 juillet 2022 dans corriger plusieurs éléments, le Haut Conseil avait notamment appelé à revoir les hypothèses d'écart de production et de croissance potentielle sur des bases plus prudente, Alors il faut comprendre ce qu'est l'écart de production pour percevoir derrière ces indicateurs de ce que veut dire le Haut conseil, l'écart de production est un indicateur économique, qui mesure la différence entre la production réelle d'une économie et sa production potentielle, c'est-à-dire le volume maximal de biens et de services qu'elle peut produire quand elle fonctionne à plein régime en utilisant toutes ses capacités, messieurs les Ministres, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je vous le dis avec beaucoup de respect, vous n'avez pas le monopole de la responsabilité. Pour faire une phrase qui, par certains qui étaient sur le monopole du coeur à l'époque. Le Haut Conseil herbe que la croissance française est déjà à son niveau maximal que les réformes dit structurel de l'assurance chômage et des retraites notamment n'y changeront rien ou ou pas grand chose, la raison, elle est simple, je me répète, en France, en France, les gens travaillent déjà beaucoup et les emplois les mieux mais rémunérés et les plus attractifs sont déjà pourvus et tout le monde le sait ici, tout le monde le sait, basé sur une combinaison d'hypothèse optimiste, le gouvernement prévoit une réduction de 2 points du taux d'épargne des ménages par rapport à celui de 2022 constat sont ensemble que beaucoup de Français tentent déjà de jongler avec des consommations subi plus de 9 % pour l'énergie, hein, moins 1 virgule 6 % de la commission sommation alimentaire sur le dernier trimestre malgré une envolée des prix de près de 10 % sur un an, il faut savoir que beaucoup de nos concitoyens arbitre entre se chauffer et manger. Mais qu'adviendra-t-il ensuite, je vous le dis, c'est une source d'inquiétude majeure pour les parlementaires communistes. Une autre hypothèse est optimiste : la hausse des investissements des entreprises, c'est un pari risqué, la question est posée que lorsqu'on connaît les versements record de dividendes de la période récente, et je vous le dis avec esprit de responsabilité au détriment de l'investissement, donc de la relance, rien qu'en 2021 les bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40 ont atteint un montant record en 2021 à près de 160 milliards d'euros en augmentation, je dis bien Avant la crise sanitaire sur ce montant 160 milliards d'investissements, vous les avez vus dans vos territoires. Non, vous avez eu des augmentations de salaires dans la plupart des entreprises concernées par ces évident non pensez-vous plus d'un tiers, 57 5 milliards d'euros sont allés dans la poche des actionnaires, je sais pas qui est concerné, ici, en tout cas, celui qui vous parle ne l'est pas l'investissement doit être tirée par le haut, par les grandes entreprises, lorsqu'on sait que 2 % des entreprises ayant investi ont généré 87 % du montant des investissements totaux dernière hypothèse qui ne sauraient pas être tenu malgré une dépréciation historique de la parité euro-dollar, alors là, c'est l'amélioration de la balance commerciale, le rapport entre importations et exportations est en déficit, et je vous le concède, messieurs les Ministres, il en déficit depuis 2006, ce n'est pas seulement de d'aujourd'hui. Et vous cherchez souvent mes chers collègues, à à vous exprimer sur ce qui devrait être un déficit structurel et bah franchement si celui-là est pas structurelle depuis 2006 chercher Zhang un meilleur par contre, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas amendable. Je le dis et je le répéterai à l'envi, ce texte est d'ores et déjà caduc, parce que les prévisions du gouvernement sont trop optimistes, s'il était respecté, il mettra en cause des acquis sociaux, la capacité d'intervention de l'État et des collectivités Tériade territoriale pour protéger les Français les plus vulnérables, je vais le résumer comme ça mais ce cette loi de programmation c'est l'antithèse de la formule de Jean Jaurès, belle formule toute la nation sera comme une immense assemblée possédante et dirigeante le tour de la croissance publics seront en moyenne et en volume des croissants de moins 0 2 % dans le projet du gouvernement, et là je me tourne sur ma droite et et en écoutant aussi le rapporteur général grâce à la droite sénatoriale, on va passer à 0 6 % c'est du jamais vu, hein, c'est du jamais vu, nous n'avons connu un tel rétrécissement de la dépense publique en 2018, mais ce n'est que parce que les gouvernements sont dépensiers par plaisir, personne ne le pense, ici, le pire c'est que la baisse des dépenses publiques et déjà miné par des restes à payer important et des engagements de dépenses à la hausse. Prévu dans les lois de programmation, je pense aux militaires à l'enseignement supérieur et d'autres encore, qu'il convient d'honorer les restes à payer sur le budget de l'État s'élevait à 178 5 milliards en 2021 dont 83 milliards pour les dépenses militaires, par exemple, les lois de programmation, elle représente 115 milliards en 2022 soit 40 % des dépenses pilotables pour chacune des années de 2023 à 2025, elles feront augmenter la dépense publique a de 5 à 6 milliards d'euros sur le budget de l'État. Il faudra couper ailleurs. Mais là, je vous pose la question, c'est pour c'est sens aussi de cette question de motions préalables mais où mes chers collègues, va falloir couper sur la transition écologique va falloir couper sur la mission Travail emploi va falloir couper sur la mission Solidarité insertion va falloir couper sur l'enseignement scolaire ou faut couper d'ailleurs dans tous ces domaines, vu l'ampleur des chiffres, le gouvernement a le mérite, et moi je lui reconnais ce mérite par exemple de dire ce qu'il va faire perdre des crédits en volume, oui, il le dit, c'est clair, au moins dans le document, il va faire part des crédits en volume à l'outre-mer, il va faire perdre des crédits aux sports et à la jeunesse et à la vie associative, c'est tout, dit c'est clair, c'est dans l'article 12 si le rejet global du texte par cette motion n'est pas voté, nous inviterons évidemment à supprimer cet article sur les bancs de nos collègues de droite où vous comptez réaliser des économies supplémentaires, dites-nous, et excusez-moi mais je, je vous le dis avec beaucoup de respect, mais c'est quand même un peu, peut-être un peu trop facile d'être libéral quand on parle de dépenses. Et d'être très interventionniste quand vous constatez les besoins dans vos départements, il y a quelque chose qui est un paradoxe difficile à gérer, me semble-t-il, vous consentez mes chers collègues de droite une ponction des concours financiers aux collectivités territoriales c'est l'article 16 plus de 6 % d'augmentation des dépenses en valeur, c'est une baisse des dotations d'au moins 4 points l'année prochaine, selon les prévisions d'inflation dans la même logique, l'article 13 entend plafonner les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à la louche pour de toute la même façon, c'est à mon avis, je comprends et je comprends la difficulté, c'est carrément inavouable, politiquement. Jusqu'où va aller l'asphyxie de nos services publics, les départements en moyenne des dépenses contraintes les allocations individuelles de solidarité qui représente 30 % de leurs dépenses de fonctionnement si les allocataires du RSA augmente si les bénéficiaires de l'allocation personnalisée autonomie augmente est synonyme de mauvaise gestion, bien évidemment que non, c'est la conséquence de la précarité, promue par les politiques gouvernementales comme l'ensemble des membres du groupe communiste, républicain, citoyen, écologique, je crois que nous devons rejeter ce projet de loi de DEC, programmation des finances publiques, c'est un moment solennel, ce débat, c'est le moment de la déprogrammation des finances publiques car le contexte conjoncturel est insuffisamment pris en compte, avec des prix des prévisions à l'aveugle à à l'influence à l'inflexion durable qui s'installe une déprogrammation des soins une déprogrammation des départs à la retraite une déprogrammation des investissements publics locaux, toutes les strates de l'action publique, sont concernés par l'austérité promises une démo déprogrammation aussi de la démocratie, empêchant à long terme de penser les finances publiques dans un scénario tenable et tenu dans le respect des engagements pris ce texte comme 11 fois sur les 14 dernières années verra le déficit dépasser la dette publique, diminuer et la croissance ne pas être au rendez-vous, je vous invite vraiment à voter cette motion préalable et merci de m'avoir laissé 45 secondes de plus merci madame la présidente, et merci à vous de votre attention. Je ne pense pas qu'il y ait d'inscription pour prendre la parole dix minutes contre la motion. Je vais demander quel est l'avis de la commission avant de vous passer la parole monsieur le Ministre.

je pense que les Français n'attendent pas de rajouter du désordre au chaos à la difficulté après l'interruption du texte et et songer à l'Assemblée nationale, nous avons défini d'abord, je pense qu'on s'inscrit dans un esprit de responsabilité le on va l'entendre effectivement ce mot oui bien sûr, mais effectivement, il n'est le monopole de personne, ça ne pose, mais il y a absolument aucun problème, par contre, une fois qu'on a donné cette nouvelle trajectoire qui est celle d'un effort partagé parce que il me semble, il nous semble qu'au regard de la situation à un moment donné, nous devons concentrer nos efforts ciblés effectivement les dépenses que l'État doit consentir. Et éventuellement à l'à son côté les le bloc des collectivités locales et et faire ce que j'ai appelé le parallélisme des exigences parce que là où il y a une vraiment une une injustice, c'est dans la proposition faite par le gouvernement de s'exonérer des efforts qu'il demande aux collectivités locales, on va vous le dire pendant plusieurs heures dans ce débat, j'ai entendu que le gouvernement, au moins dans les paroles et dans les intentions semblent partager l'avis de du Sénat, raison pour laquelle la le motions préalables du du groupe communiste et républicain reçoit un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. avis défavorable également, je voudrais juste répondre à à certaines remarques qui ont été faites sur. Notre réponse aux problème immédiat qu'est l'inflation et nos réponses aux problèmes structurels de l'économie française que nous essayons de résoudre depuis un peu plus de 5 ans. Sur l'inflation ou vous nous parlez de précarité. c'est une précarité à 100 milliards d'euros qui ont été dépensés de 2021 à 2023 pour protéger nos compatriotes et protéger les entreprises contre l'inflation. La vraie précarité. C'est celle qu'ont voté vos alliés de la NUPES en supprimant le bouclier tarifaire sur l'électricité sur le gaz. Pour financer une explosion de MaPrimeRénov'. ça, c'est 580 euros à débourser chaque année en moyenne par ménage, ça c'est de la vraie précarité. Et si les votes ont un sens et en démocratie, ils en ont, hein, la NUPES a voté la précarité énergétique généralisé pour nos compatriotes en supprimant le bouclier énergétique qui protège depuis près de 2 ans, nos compatriotes contre la flambée des prix, d'électricité et la flambée des prix du gaz et les votes ont un sens, nous, à l'inverse, nous avons mis en place ce bouclier nous avons indexer l'ensemble des prestations sociales nous avons indexer le SMIC, je rappelle que nous sommes l'un des seuls pays européens à avoir un salaire minimum qui est indexé sur l'inflation, le seul salaire qui est augmenté de près de 8 plus de 8 % même c'est le SMIC depuis un an, parce qu'il y a une indexation du SMIC sur l'augmentation des prix, aucun autre pays européen, là, ce type de dispositif, nous venons de mettre en place l'augmentation de 50 % monsieur le sénateur de l'allocation de soutien familial qui passe à 184 euros, qui touche 800000 femmes seules, enfin si c'est pas de la lutte contre la précarité, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on peut critiquer par tous les biais notre politique, mais certainement pas dire que nous ne luttons pas avec efficacité contre la précarité, nous sommes l'un des seuls pays en Europe où, malgré la crise du Covid malgré la crise de l'inflation, le taux de pauvreté n'a pas augmenté. 14 %, c'est toujours trop. Mais c'est mieux que les autres pays européens, c'est mieux, évidemment, que les États-Unis, ou à cause de l'inflation, à cause de la crise du Covid les inégalités et la pauvreté honte exploser. S'agissant des salaires, je le redis, si les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires, ils ont augmenté d'en moyenne 3 5 % depuis le mois de juillet, et j'invite toutes celles qui le peuvent à augmenter les salaires, enfin, s'agissant des entreprises nous avons protégé aussi puisque nous avons mis en place des mesures à hauteur de 10 milliards d'euros pour amortir le choc de l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz sur les entreprises, mais je crois que nos vraies différences et c'est tout l'intérêt du débat que nous avons ici c'est sûr. Le diagnostic que nous portons. Sur la situation de l'économie française et des comptes publics depuis je dirais 3 décédé, qu'est ce qui caractérise la France depuis 3 décennies et qu'est ce que nous essayons de renverser pour opérer cette révolution économique, il doit donner de la prospérité de la justice à nos compatriotes, la première chose qui caractérise la France par quelque bout qu'on le prenne, c'est que c'est le niveau de dépenses publiques le plus élevé des pays européens, juste derrière le Danemark, donc si la dépense publique, faisait le bonheur d'une nation, la nation française serait la plus heureuse de toutes les nations européennes, j'ai peur que ce ne soit pas encore tout à fait le cas pour une raison qui est simple, c'est que je pense que les Français estiment à juste titre. Qui n'en ont pas, pour leur argent. Si on regarde ce niveau très élevé de dépenses publiques, il se disait, tout va bien à l'hôpital, tout va bien à l'école, tout va bien dans les collèges, tout va bien dans les universités, je pense qu'ils accepteraient ce taux de prélèvements obligatoires à ce taux de dépenses publiques très élevées, mais comme ça n'est pas le cas, nous devons avec résolution chercher un meilleur emploi de la dépense publique, une plus grande efficacité de la dépense publique, je suis le rapporteur général sur la nécessité que l'État donne l'exemple aux côtés des collectivités locales pour réduire la dépense publique et avoir une dépense plus juste et plus efficace, notamment pour nos services publics, la 2ème chose qui caractérise la France et que, là aussi avec la majorité avec Gabriel Attal avec le président de la République, avec tous les sénateurs de la majorité, nous avons voulu renverser comme tendance depuis maintenant plus de 5 ans, c'est que nous avons les impôts les plus élevés de tous les pays européens, juste derrière le Danemark et viennent de tomber, on a réussi à les baisser d'un point en moyenne. On a un peu amélioré la situation, mais malgré tout il y a toujours plus d'impôts toujours plus de taxes, toujours plus de prélèvements obligatoires, d'autres pays qui sont proposés par les uns par les autres, je voudrais que, comme l'on disait dans la Bible, les écailles tombent des yeux de certains qu'ils s'aperçoivent que ce taux de prélèvements obligatoires est insupportable pour nos compatriotes qui se disent : pourquoi tant d'impôts pourquoi tant de taxes pourquoi 30 prélèvements obligatoires et pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, vous nous dites : augmenter les impôts, augmenter des taxes augmenter les prélèvements obligatoires, je considère une bonne fois pour toutes que c'est la mauvaise solution et que si on veut de la justice fiscale et je veux la justice fiscale et des mois sur la taxation des géants du numérique et des mois sur la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés des mois, pourquoi pas sur la taxation de l'utilisation des infrastructures numériques par les géants du digital et des mois sur le prélèvement que nous faisons de la rente des énergéticiens qui va nous rapporter 26 milliards d'euros, ça c'est de la vraie justice n'allait pas chercher l'argent dans la poche des Français, ce n'est plus la solution, et d'ailleurs, je considère que ça ne l'a jamais véritablement été enfin le dernier point sur lequel nous serons en désaccord, c'est sur le volume global de travail. Le volume global de travail en France est insuffisant par rapport aux autres grandes nations européennes et petit à petit, par quoi est-ce que ça se traduit par un appauvrissement relatif de la France par rapport aux autres grandes nations européennes, donc où il faut avoir le courage de baisser les impôts, oui il faut avoir le courage de réduire la pression fiscale, oui il faut avoir le courage de réduire la dépense publique pour que nos services publics auxquels je tiens autant que vous, je vois bien financé, et oui il faut avoir le courage d'engager une réforme des retraites, avec le souci de la justice, du respect des carrières longues, du respect de la pénibilité des métiers, mais tout simplement pour accroître le volume global de travail qui fera la prospérité de la France et la prospérité des Français. Merci, a-t-il d'autres explications de vote. Je n'en vois pas, je vais donc consulter le Sénat sur la motion tendant à poser à opposer la question préalable, je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion : avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote pour Monsieur Savoldelli oui mais, et ce serait bien de lever, voilà, si vous pouviez exprimer vos votre voilà merci qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous poursuivons donc la discussion générale, la parole est à monsieur Christian Billac du groupe RDSE pour cinq minutes chers collègues. madame la présidente, monsieur les ministres, madame la rapporteure, où je suis, le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances à mes chers collègues. L'Assemblée nationale a donc rejeté le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2003 2027, c'est quelque chose d'inédit et les conséquences d'un rejet définitif on difficile évaluer, laissant craindre le nom versement de fonds européens à la France les objectifs des lourd de programmation budgétaire ont rarement été respecté par le passé, je ne serais pas surpris que ce texte, comme les précédents, soit un exercice imposé plutôt que la feuille de route, et ce malgré les nouvelles disposition du juge hâtive si je partage la volonté de redresser les comptes publics, je regrette que ce projet repousse en toute fin de période, le retour attendu plus de rapidité ferait, me semble-t-il nécessaire ce texte répond aussi au calendrier budgétaire européen et aux engagements pris par la France, mais le jour de la certains principes prévalent et permet de frein sur lors de l'examen du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes 2021, je rappelle que les comptes en désordre sur la marque des nations qui s'abandonnent, je rappelle aussi que les paysans disent qu'il convient de dépenser moins, ce que ce que l'on gagne et de faire des économies en prévision des mauvaises récoltes à venir, c'est le simple bon sens,

prévoyant de réduire le déficit structurel et là pour poursuite d'impôts, tablant sur des taux d'intérêt de de 6 à court terme et 3 à long terme en 2027 ce scénario me semble plutôt optimiste la situation financière dans notre pays et pour le moins préoccupante mais à votre décharge, messieurs les Ministres, je dois convenir que la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et maintenant la crise énergétique sont grandement responsables la situation j'espère et nous aspirons tous revenir rapidement à une situation qui pourra être normal, même si la géopolitique n'apporte pas un vent d'optimisme

fort des administrations locales 27 milliards d'euros, fort de l'État administration centrale 0 euros. Le responsable fait donc payer les autres, et en particulier les collectivités locales qui ne sont aucunement responsables du déficit puisqu'elles ont l'obligation de voter des Budgets en équilibre. La progression des dépenses de fonctionnement doit rester inférieure à l'inflation, moins 0 5 mais comment réussir à le contexte actuel et les collectivités n'atteignant pas l'objectif riche collège plus lourde des suivre une sorte de l'État, le texte issu de la commission ne va pas fait changer d'avis, cette loi de programmation de nos programmes, rien du tout, je regrette qu'elle ne prévoit pas un partage de responsabilités acteurs locaux qui ont fait leurs preuves sur le terrain, ce serait utile pour l'État qui doit se concentrer sur ses millions sur ses missions régaliennes, donne les moyens sont notoirement insuffisants, plutôt que de s'entêter à tout faire tout seul, quand on fait tout, on fait tout mal à quand une nouvelle étape de la décentralisation, en ce qui concerne les administrations de Sécurité sociale, le projet de loi prévoit 27 milliards d'économies. Le gouvernement table sur la réforme des retraites pour réduire le déficit, mais chacun sait qu'elle ne portera pas ses fruits au revoir l'exécution de cette loi de programmation pourtant les besoins sont immenses dans la branche maladie avec les déserts médicaux que se multiplient les urgences saturées et la fermeture des lits, voire l'établissement mais aussi dans la branche autonomie avec une âge situation alarmante des Ephad et en particulier des j'ai pas ce ne sont pas les 3700 créations de postes prévues au PLFSS 2023 qui vont régler le problème, cela représente la création d'une demi-poste par établissement pour conclure ce texte traduit une gestion molle des finances publiques, j'ai créé dire semble aussi balancer comme les feuilles mortes au gré du vent et, comme l'a écrit Sénèque à Lucy, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, c'est pourquoi je voterai personnellement contre ce projet de loi de programmation, les membres du groupe RDSE conformément à notre position traditionnelle détermineront leur vote en fonction des débats, je vous remercie. Merci, Charles, collègue, la parole est à présent à Madame Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains, vous avez 8 minutes chers collègues. Monsieur le Ministre, le 13 juillet devant la commission des finances du Sénat le 1er président de la Cour des comptes, président du Haut Conseil des finances publiques préconisé d'établir une loi de programmation crédible et global, c'est-à-dire avec des hypothèses réalistes des mesures d'économies détaillées articulée articulée avec les lois de programmation sectorielles ne reportons pas l'effort en fin de période et associant l'ensemble des acteurs publics, le gouvernement ne semble pas avoir fait Sciences mantra tout d'abord le conseil des finances publiques et les analystes économiques considèrent les hypothèses macroéconomiques improbable l'avis du Haut Conseil relève que la trajectoire de la LPFP repose sur 3 hypothèses favorables soit un mouvement de des épargne des ménages au 3ème trimestre, la croissance de la consommation et de 0 % après 0 3 au 2ème le maintien à un niveau élevé de l'investissement des entreprises, et enfin une contribution positive du commerce extérieur au 3ème trimestre elle est négatif à moins 0 5 permettez-nous donc d'avoir des doutes sérieux sur la possibilité que ces 3 critères soient réunies pendant les 5 prochaines années, au regard des dernières données publiées par l'Insee dans son dernier repère l'institut Rexecode écrit que si des perspectives de croissance du PIB plus prudente mais sans doute plus vraisemblable se réaliser le déficit public ne se résorberait pas et la dette publique continuerait d'augmenter, en pourcentage du PIB, pour atteindre 120 % en 2027 ceci montre combien la trajectoire est sensible à son point de départ, dans ses perspectives sur l'économie mondiale d'octobre, le FMI anticipe que plus de la moitié des pays de la zone Euro connaîtront une récession technique cet hiver, la France est relativement épargnée puisque le truc même instituts tablent sur une croissance de 0 7 % pour 2023 en deçà cependant de l'hypothèse du gouvernement malgré une anticipation très optimiste de la croissance, le déficit reste de 5 % et ne retrouve son niveau de 3 % qu'en 2027, nous serions donc pendant 2 ans les plus mauvais élèves de la zone Euro, mais ce chiffre de 5 pour fait oublier tous les ordres de grandeur le déséquilibre des finances publiques est plutôt de 45 % le PLF dont nous discuterons prévoit bientôt prévoit 500 milliards de dépenses, contre 345 milliards de recettes, la maîtrise des dépenses publiques est pourtant devenu un totem, combien de fois avons-nous entendu que le temps du quoi qu'il en coûte, est derrière nous, que maintenant nous sommes à l'euro près, je vous cite, qu'il s'agit désormais de décider en fonction du combien ça coûte, or les dépenses courantes augmentent de 62 milliards dans le PLF déposé le 26 septembre et depuis cette date plusieurs dépenses nouvelles ont déjà été annoncées : hausse du bonus écologique élargissement du bouclier tarifaire et tant d'autres, la baisse du ratio de la dépense publique inscrite dans la programmation repose en grande partie sur la disparition progressive des dépenses exceptionnelles, soit encore 61 milliards en 2022 concernant la dépense courante, le rapporteur général, a rappelé la trajectoire suit celle des dépenses publiques du quinquennat précédente 140 milliards en plus l'objectif de moyen terme de solde structurel fixées par l'article 5 d'un règlement européen depuis 1997 ne sera pas atteint pendant l'ensemble du quinquennat il sera au mieux égal à la moitié de l'effort attendu, soit 0,3 point par an de 2000 24 à 2027 l'insuffisance de réduction du déficit structurel, souligne le manque d'engagement de réformes, les mêmes réformes reviennent dans les PNR successifs, toujours aussi peu documentée en 1er lieu la réforme des retraites, l'État demande des efforts aux Français et aux collectivités territoriales, qu'il ne s'impose pas à lui-même, l'effort exigé des APUL n'a jamais été atteint au cours des 40 dernières années, pourtant, le rapporteur général à l'Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve a reconnu que la situation sera difficile pour les collectivités territoriales année prochaine et elle le sera aussi pour l'État français pour les entreprises et pour tout le monde, je le cite toujours, il faut partager cet effort entre les les différentes administrations, c'est une question de responsabilité l'effort que nous demandons à l'État qui viendrait exposées par le rapporteur général et toutes choses égales par ailleurs, plus faible que pour les collectivités, en effet, l'indice des dépenses communales ou encore le panier du maire estimé sur le 1er semestre 2022 fait apparaître une évolution de 4 8 % sur quatrième 4 trimestres glissants sur la même période l'indice des prix à la consommation hors tabac n'avait progressé que de 3 4 % le différentiel s'est encore accru au cours des 2ème et 3ème trimestres par ailleurs plusieurs textes législatifs récents contraignent les Budgets locaux à plus ou moins long terme, en tout 1er lieu la loi climat et résilience d'août 2021, c'est un effort nécessaire auquel les collectivités sont prêtes, encore faut-il qu'elles en aient les moyens, la maîtrise de la dépense publique ne se décrète pas, elle se construit dans la durée, Gérard Longuet reviendra sur cette thématique en l'illustrant avec des politiques publiques, c'est parce que vous nier cette réalité que vous avez imposé aux grandes collectivités, les contrats de Cahors, vous vous êtes félicité des résultats, alors même que ce n'est que la conséquence des efforts de gestion rendue nécessaire par la contraction des concours financiers de l'État sur la période 2014, 2017, le gouvernement indique avoir conçu un nouveau dispositif, les contrats de confiance, comment osez-vous dire que le dispositif est différent, alors que l'article 23 et partiellement un copié-collé de l'article 29 de la précédente LPFP les collectivités sont tenus de présenter un budget en équilibre, elle ne participe donc pas la dérive de nos comptes publics, contrairement à l'État qui, cette année encore, va devoir financer 158 milliards d'euros de déficit et en comptant les refinancements 270 milliards de dettes par ailleurs la référence retenue est mauvaise, c'est sur la base de l'autofinancement et non pas de la dépense que s'effectue le pilotage financier des collectivités locales, car ce dernier permet la couverture des dotations aux amortissements et de financer les investissements, messieurs, le ministre l'effort demandé à l'État et réaliste, nos collègues de l'Assemblée nationale dans la continuité des travaux de parlementaires de la majorité vous ont proposé de passer d'un État bedonnant et le mal-voyants à un État et clairvoyant en 20 ans le nombre de décrets d'application, a augmenté de 310 pour 100 en 2019, le Conseil d'évaluation des normes évaluer le coût des obligations normative à 790 millions d'euros pour les collectivités, atteindre la moyenne des pays de l'OCDE pour le ratio coût de production des services publics sur le PIB, permettre de dégager 84 milliards d'économies dans une note récente l'Ifrap estime la charge administrative de 12 à 25 milliards pour les collectivités, les services publics et les particuliers, cet effort réaliste est indispensable si nous souhaitons faire refluer notre endettement dans la programmation du gouvernement, la dette ne serait tués qu'à partir de 2026 uniquement grâce aux excédents budgétaires des APUL et des assauts, comme l'a justement souligné Élisabeth Doineau, rapporteur pour la commission des affaires sociales, la trajectoire de l'Ondam apparaît fragile et parfois d'une crédibilité discutable dans leur sagesse, les membres de cette commission ont amendé le texte afin que le compteur des écarts trouve à s'appliquer à toutes les lois de financement de la Sécurité sociale jusqu'en 2027, les Français doivent prendre conscience que le gouvernement fait vivre le pays avec une épée de Damoclès un biais optimiste dans les projections projections de finances publiques devient problématique dès lors que les conditions de financement de la dette sont plus dépendante des marchés dans un environnement rendu moins favorable au financement des dettes publiques par le resserrement de la des politiques monétaires, un déficit de crédibilité peut induire une prime de risque qui viendrait augmenter la charge de la dette et par conséquent contraint le financement de l'action publique cette prophétie pourrait malheureusement se réaliser après plus 0,5, juillet plus 0 75 points en septembre, jeudi dernier, la BCE a augmenté ses taux directeurs des euros 75 points le taux des OAT à 10 ans a dépassé 3 % le 21 octobre alors qu'il était encore négatif en décembre 2021 pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains soutient le texte issu des travaux de la commission des finances, vous aurez d'ailleurs noté notre sobriété en matière de dépôt d'amendements car la trajectoire concilie quatre objectif: réduire le déficit et l'endettement public plus rapidement que dans la programmation du gouvernement, assurer la pleine contribution des administrations centrales, préserver les dépenses sociales et régalienne conserver des marges d'intervention dans un contexte où une crise en chasse une autre. Les 2 ministres nous ont appelés à être responsable avec cette LPFP, amender, nous le sommes. Merci, la parole est à présent à notre collègue le sénateur Emmanuel Capus pour le groupe des Indépendants et vous avez 5 minutes chers collègues. monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a 3 cas de figure, où l'on refuse de se fixer un objectif, le 1er c'est lorsqu'on n'est pas sûr de l'atteindre le 2ème c'est lorsqu'on est sûr de ne pas l'atteindre et le troisième, c'est lorsqu'on ne veut rien atteinte du tout. Je me réjouis que la commission des finances du Sénat considère que nous ne sommes dans aucun de ces cas, en choisissant d'amender le texte, nous nous mettons dans l'objectif dans l'optique de fixer un objectif clair pour nos finances publiques, c'est une démarche responsable qui fait honneur à notre chambre, notre groupe là soutient pleinement à l'Assemblée nationale, les oppositions se sont ligués non pas pour amender le texte, elles sont incapables de trouver un accord, mais pour le rejeter en bloc, je regrette qu'elle cède à l'appel du chaos, comme l'a rappelé le rapporteur général plutôt que de s'accorder sur une programmation qui donne de la visibilité à nos finances publiques. Bien sûr, il est toujours possible d'améliorer un texte, nous avons d'ailleurs déposé plusieurs amendements afin de renom de renforcer 3 ambition du projet porté par le gouvernement, la première de ses ambitions, c'est la maîtrise des dépenses publiques, je salue la démarche du gouvernement qui présente une trajectoire qui ramène le déficit sous la barre des 3 % du PIB à horizon 2027 ce n'est ni une obsession, ni une lubie, c'est simplement un engagement que nous avons que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens, vous l'avez parfaitement bien rappelé, Monsieur le Ministre, lors des débats pour la modernisation de la LOLF il y a un an, notre groupe avait toutefois fait adopter un amendement pour préciser que le projet de loi de programmation dans son rapport annexé devait présenter une comparaison européenne cette comparaison, à défaut d'être réjouissantes est éclairante, tous les autres États ont adopté une loi de programmation et tous de la Grèce, au Portugal, en passant par l'Italie et l'Espagne, tous sont prévus de repasser sous la barre des 3 % d'ici 2025, tous sauf nous qui attendront 2027, c'est pourquoi nous avons présenté plusieurs amendements visant à encadrer plus fortement les dépenses de l'État qui porte l'essentiel du déficit et la dette mais Monsieur le Ministre, les filles sont clairs pour rétablir nos comptes, nos efforts doivent porter principalement sur les administrations centrales, c'est une question d'équité et d'efficacité, de ce point de vue, les propositions de la commission des finances, me paraissent intéressantes, nous à Roland, occasion d'en débattre plus longuement tout à l'heure et monsieur maire tout à l'heure avant son départ avait à juste titre, rappeler que les propositions qui étaient faites était bonne et honnête. La seconde ambition que nous souhaitons renforcer c'est le verdissement du budget, il s'agit d'un levier indispensable pour accélérer la transition écologique, nous avons fait adopter en commission un amendement pour le budget général, nous vous ont proposeront un autre pour engager une telle dynamique au sein des collectivités locales, la 3ème ambition c'est le respect des libertés locales, l'article 23 il faut le rappeler est bien meilleure que la baisse brutale des dotations imposées sous le sous la présidence du président Hollande mais vous savez, Monsieur le Ministre, que c'est un sujet de préoccupation du Sénat, les collectivités ne sont pas responsables de l'aggravation de notre déficit public et de notre dette en 2021, elles ont même dégagé près de 5 milliards d'euros d'excédents, elle ne représente que sept % l'endettement public et 20 % de la dépense publique,

particulièrement vigilants quant au l'autonomie financière des collectivités, j'espère donc que nous trouverons une solution pour donner des gages à nos partenaires européens sans contraindre excessivement les collectivités, il faut éviter de monter l'État contres les collectivités, la crise nous la rappeler les collectivités ont besoin de l'État et l'État a besoin des collectivités, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Daniel, Daniel, pardon du groupe écologiste, vous avez 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la Commission, messieurs les Ministres, chers collègues. Penser l'avenir, c'est l'idée que l'on se fait d'une loi de programmation, je ne parle pas ici de boucliers nécessaire, même lorsqu'ils sont mal ciblées, ni d'orthodoxie budgétaire réaffirmer et amplifier sous le nom de sérieux budgétaire, mais bien de penser l'avenir et notamment le bouleversement climatique et les désordres qu'il va induire les moyens de l'indispensable mutation pour y répondent, ce n'est pas possible en poursuivant le désarmement financier de l'État et la mise au pain sec des collectivités, entendez les scientifiques, messieurs les Ministres, la dette climatique coûte et coûtera plus cher que la dette financière chaque année d'inaction ou de petits pas nous condamne à devoir faire face à des sécheresses durables et étendue des inondations, des canicules des incendies des tempêtes qui détruisent des villages entiers Bihucourt dans le Pas-de-Calais, oh Shany en Corse, après la Roya et avant qui ce sera de plus en plus dur et de plus en plus douloureux mais d'abord pour les plus modestes d'entre nous sur le plan social, cette loi de programmation et libérale, elle est encore durci par la volonté de la majorité sénatoriale. De coupe massive des dépenses publiques et de réduction accélérée de la dette, cela fait courir le risque au pays de basculer dans la récession, l'aggravation du sentiment d'injustice et l'effondrement continu des services publics, l'hôpital l'écoles, les universités, l'Office national des forêts putain de service public sont déjà à la peine, mais cinq minutes qui me sont accordées ne suffirait pas à les citer pourtant cet entêtement de baisse des prélèvements obligatoires a réussi sur un point : par le passé, c'est la hausse record des dividendes, nous avons le triste record d'Europe triste à mon sens, quand la France entière et des kilomètres de queue à la pompe pour payer un carburant trop cher au détriment d'autres dépenses essentielles : comment accepter qu'une entreprise comme Total énergies des 6 6 milliards de bénéfice au 3ème trimestre 2022 c'est indécent pour les salariés comme pour les citoyens, comme le sont les presque 60 milliards de dividendes versés par le CAC 40 l'an passé dans notre pays, car oui, il y a de l'argent total est l'illustration ultime et caricatural du système que vous soutenez mordicus la baisse de la contribution des plus aisés n'est pas plus acceptable car l'impôt reste l'outil indispensable d'une société juste et civilisée, c'est pourquoi les écologistes refusent la suppression de la CVAE revendique une taxation des dividendes supérieure à celle du travail et propose un ISF climatique, c'est un encouragement à être vertueux et solidaire qui repose sur l'inclusion dans le calcul de l'impôt des plus fortunés d'un malus assis sur l'empreinte carbone de leur Patrimoine financier, nous vous proposons aussi. La création d'une loi de programmation pluriannuelle des financements de la transition écologique qui assurerait une meilleure visibilité aux entreprises et aux ménages, aux investisseurs comme aux collectivités territoriales pour les entreprises, il serait de bon sens que l'octroi des aides publiques soient systématiquement conditionnée à des contreparties sociales et écologiques, il y a urgence, urgence aussi pour les collectivités, vous ne cessez de diminuer leur autonomie et la capacité à agir des communes, vous ne les protégeaient pas ou pas assez face à l'inflation et au coup spéculatif de l'énergie, vous leur avez retiré la quasi-totalité, vous et vos prédécesseurs de leurs pouvoirs fiscaux mais ça ne vous suffit pas, vous voulez aussi contrôler leurs dépenses, la réduction des charges de fonctionnement n'est plus chez vous, du domaine de l'entêtement mais de l'obsession, surtout quand il s'agit des charges de fonctionnement des autres. Baisser le fonctionnement, cela signifie cesser d'accueillir les tout petits dans les crèches, les enfants à la cantine, fermer des médiathèques, des espaces culturels, des équipements sportifs, des centres de loisirs ou encore des centres de santé, dont vous étiez pourtant satisfait qu'il permette la vaccination de tout le monde, voilà quelques mois, rien ne le justifie, car les collectivités sont gérées sainement sans déficit, contrairement à notre état jacobin et avec un fort investissement utile à l'ensemble du pays, vous devriez au contraire soutenir les collectivités, elles sont le laboratoire innovant de nombreuses politiques publiques nécessaires pour la transition, elles sont enfin en cette période de crise, un rempart démocratique que sur tous les bancs, nous devrions soutenir et respecter, il faut miser sur elle avec résilience, elle gère le quotidien construisent l'avenir, c'est ce que nous attendons des lois de programmation et c'est pourquoi nous ne voterons pas celle-ci. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Didier Rambaud, sénateur du groupe RDPI, vous avez six minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui devant un choix décisif qui engagera notre responsabilité pour les 5 années qui viennent et, en cela, c'est même de l'avenir de notre pays et de ses finances que nous sommes amenés à discuter, cela fait des mois que le Haut Conseil des finances publiques, nous affirme qu'il sera nécessaire de modifier les règles communes du pacte de stabilité européen mais quelle que soit la souplesse qui sera apportés pour permettre aux États de d'affronter les crises avec une politique contracyclique ambitieuse, il est impératif que nous gardions le cap des 3 % de déficit, réduire la dette doit également être un cas prioritaire en sortie de crise car depuis le début des années 2000, cette dette n'a jamais des des crues, tous gouvernements confondus, l'ampleur des 2 crises survenues depuis 2007, il n'y est pas étrangère, lorsque le monde s'est arrêté en 2020, l'État a soutenu l'économie, les collectivités locales et les Français, au prix d'un effort budgétaire sans précédent, donc nous ne devons pas oublier le poids, poids considérable qui rappellent à radoter à redresser le cap en sortie de crise, nous avons une trajectoire fixée dans le cas du programme de stabilité qui nous engage vis à vis de nos partenaires européens le devoir de responsabilité qui doit nous a dit, mais les élus locaux le connaissent bien, c'est celui qui anime au quotidien dans la gestion de leurs comptes si nous poursuivons la trajectoire fixée par le gouvernement, nous tiendrons l'objectif de 5 % de déficit l'an prochain après avoir l'objectif pour cette année et nous serons revenus sous les 3 % en 2027 la trajectoire, présenté par le gouvernement prévoyait de diminuer la dépense publique de de 6 % en volume en 2023 en part de PIB, elle doit ces de 57,6 % à 56,6 % l'an prochain, est tombé à 53,8 % en 2027 c'est le l'effort le plus soutenu depuis 20 ans certains ma à ma droite, affirme pourtant que l'effort n'est pas suffisant qui les réformes structurelles qui a appuieront cet effort ne sont pas assez documenté, permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas une loi de programmation d'inscrire dans la dans le marbre, ni le calendrier ni les modalités des réformes à venir, c'est frustrant, j'en conviens mais nous devons fixer un cap pas préempter ce qu'il appartiendra au gouvernement et à la discussion parlementaire du fixé en temps voulu, j'ajoute également que nous avons des éléments sur les réformes à venir, la réforme des retraites devrait pouvoir aboutir dès l'été 2023 pour ce qui est de l'assurance chômage, il appartient désormais à la commission mixte paritaire de se prononcer, monsieur le rapporteur général je je tenais à vous citez l'ensemble des réformes structurelles évoquées par le gouvernement soit absolument nécessaire, nous avons besoin d'une réforme de retraites, nous avons besoin de renforcer le taux d'activité des seniors, nous avons besoin de réformer le fonctionnement de l'assurance chômage et du service public de l'emploi pour réduire le taux de chômage vous réclamer une réforme des retraites plus importante que celle annoncée par le président de la République, sans nous dire au juste ce que vous entendez par là, l'instant d'avant, vous nous disiez que les contours du projet présidentiel n'était pas clair, il faudrait savoir, je m'interroge aussi sur vos propos en commission, vous avez détaillées à grand renfort de chiffres et de et de graphiques que les effets des réformes du gouvernement sur la croissance et le déficit serait surestimer et sous-de documenter et l'instant d'après vous préciser que la trajectoire à Paris peu ambitieuse, chers collègues de la majorité sénatoriale pour vous pourriez-vous alors nous expliquer comment vous comptez procéder pour aller plus loin, je constate en réalité que toute cette apparente radicalité vole en éclats lorsqu'il s'agit des collectivités locales vous valider la trajectoire des concours financiers aux collectivités locales prévues par le gouvernement, et c'est tant mieux, vous nous dites que les collectivités territoriales ont pris leur part dans le redressement des comptes publics au cours des derniers qu'un quinquennat c'est exact dans le précédent quinquennat là l'État a pris plus que sa part pour protéger les collectivités face à la crise, le déficit des collectivités en 2000 vas était à 0 virgule 15 quand celui de l'État et de la sécurité sociale s'est envolé 8 8, dès collectivités ont retrouvé des marges excédentaire, quand l'État a continué d'absorber le choc, c'est le choix courageux que nous avons fait dans le contexte actuel, chacun doit prendre sa part des erreurs du passé et contribuer au rétablissement des comptes de la nation, je partage cependant votre inquiétude sur les fortes incertitudes face à l'inflation et elle et la crise énergétique, les dépenses de fonctionnement des collectivités sont terriblement contrainte et nous pouvons nous interroger sur la soutenabilité d'une trajectoire à cinq ans, si l'inflation venait à dépasser les seuils de référence monsieur le Ministre je compte sur vous pour nous rassurer dans cette hypothèse sur la souplesse du mécanisme que vous réintroduisez à l'article 23 le dispositif permet par ailleurs de répondre aux principales critiques qui ont été formulées à propos des contrats de Cahors et sous réserve de cette précision, je soutiendrai son rétablissement avec ce nouveau dispositif qui ne concernent, je rappelle que les collectivités dont le budget dépasse les 40 millions d'euros, soit à peu près 500 collectivités donc de notre pays, les objectifs seront fixés par strates et après un an, nous si la strate a atteint c'est donc a priori une relation de confiance puisque les mesures de correction qui s'imposent n'interviendront que si les objectifs ne sont pas un tas et je rappelle que intercommunautés de France a salué ce dispositif, l'association des départements de France également, sous réserve de certains aménagements qui devraient être retenus, le gouvernement aurait pu, comme sur le quinquennat Sarkozy rogner peu à peu sur la DGF jusqu'à son gel brutal en 2011, nous aurions pu, comme sous le quinquennat Hollande sabrer dans la DGF qui a baissé, je vous rappelle, de 12,5 milliards d'euros, mais au contraire en proposant pour la première fois depuis 13 ans, d'augmenter la DGF de 320 millions d'euros au PLF 2023, le gouvernement fait le choix de la confiance, un choix que le groupe RDPI soutiendra. Cher collègue, la parole est à présent à monsieur Rémi Féraud, sénateur du groupe socialiste, vous avez 9 minutes de temps de parole cher collègue.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général chers collègues. Il y a 5 ans intervenant au nom du groupe socialiste, sur le même document qui trace les perspectives budgétaires du quinquennat notre collègue Thierry Carcenac alerter sur plusieurs points essentiels qui lie relever l'injustice fiscale et sociale des mesures annoncées, les relations déjà dégradée de l'état avec les collectivités territoriales et le manque criant de soutien aux services publics de notre pays en étudiant la loi de programmation des finances publiques qui nous intéresse aujourd'hui, je crois que rien n'a fondamentalement changé dans la politique menée, sauf que vous n'avez pas trouvé cette fois une majorité à l'Assemblée nationale pour l'approuver et surtout la loi de programmation présentée ne tire pas les enseignements des 5 années précédentes, ainsi la crise des gilets jaunes a montré, et avec quelle acuité la nécessité de renforcer la présence des services publics sur l'ensemble du territoire, ainsi que l'enjeu crucial du pouvoir d'achat et de la justice sociale, la crise sanitaire, a mis en lumière les défaillances de notre système de santé et bouleverser l'économie mondiale, le retour de la guerre en Europe à entraver la reprise de l'activité et amplifier l'inflation qui pousse nombre de nos concitoyens dans la difficulté ou dans la pauvreté, la remontée des taux d'intérêt, a commencé, et personne ne sait où elle s'arrêtera et enfin la politique du ruissellement et de plus en plus largement reconnu comme un échec jusqu'à la Maison Blanche, désormais, mais malgré tout, malgré la accession de crise et l'accroissement des inégalités dans notre pays, malgré l'impréparation écologique malgré les alertes sur l'état de nos finances publiques, ce projet de loi de ce projet confirme l'orientation libérale choisie par le gouvernement depuis 5 ans et il faut le reconnaître totalement assumé il poursuit le mouvement de désarmement fiscal et une maîtrise entre guillemets de la dépense publique qui est la conséquence de l'appauvrissement de l'État, tout en restant pourtant toujours insuffisante aux yeux de la majorité sénatoriale, votre politique budgétaire Monsieur le Ministre, celle que vous prévoyez pour les 5 prochaines années, elle, mais à notre avis en péril à la fois le redressement de nos services publics et les marges de manoeuvre des collectivités locales, déjà fortement mise à mal. Que ce soit pour les collectivités territoriales ou l'hôpital public, ce ne sont pas simplement les Ségur ou le pacte de confiance que vous proposez, qui leur permettront de sortir la tête de l'eau et qu'en est-il pour les salaires des enseignants et leur augmentation si urgente, qu'en est-il pour les investissements dans le ferroviaire, qu'en est-il pour l'investissement dans la rénovation énergétique, la liste des besoins et longue et le train, le tableau que dresse le gouvernement sur les différentes missions budgétaires reste entièrement centré sur les missions relevant du régalien qui ont besoin de moyens supplémentaires, mais les chiffres sont d'autant plus inquiétant sur l'ensemble des autres missions, surtout lorsqu'on tient compte de l'inflation nous pensons au contraire que pour sortir par le haut des crises, économique, sociale, écologique, démocratique actuel, notre pays devrait répondre avec volontarisme à 3 grands enjeux, réduire les inégalités de revenus et surtout de Patrimoine, redonner de la force à nos services publics qui se sont tant dégradée et accélérer la transition écologique en mobilisant beaucoup plus de moyens à cet effet, pourquoi n'en avez-vous pas les moyens, pourquoi la dette budgétaire et la dette climatique continue-t-elle de gonfler toutes les deux parallèlement. parce qu'en 10 ans, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, auront organisé la perte de près de 400 milliards d'euros de recettes pour l'État si on intègre les annonces qui sont faites pour ce quinquennat cela représente une moyenne de 39 milliards d'euros par an, à titre de comparaison, si on prend le chiffre du budget 2023 fin du projet de budget, c'est 2 fois et demie le budget du ministère de l'Écologie et votre politique de baisse des impôts, elle se révèle impuissant font le ministre Bruno Lemaire là d'ailleurs dit lui-même, tout à l'heure à demi-mot, il en faut toujours plus et qui devra payer les nouvelles mesures fiscales favorables aux entreprises comme la suppression de la CVAE puisqu'elle est entièrement elle devient automatiquement une dépense supplémentaire de l'État, hé bien ce sont les Français les mêmes français qui ont déjà compensé depuis 5 ans, les baisses des impôts de production, la suppression de l'ISF, la mise en place de la flat tax pour les revenus du capital, etc. Car pour équilibrer le budget après toutes ces réductions d'impôts au profit des entreprises des plus aisés et des détenteurs du capital, le gouvernement est bien contraint de mettre à contribution tous les Français et aussi les collectivités territoriales et aussi les bailleurs sociaux et aussi les chômeurs en faisant passer une réforme de l'assurance-chômage qui pénalise les plus fragiles et surtout désormais le gouvernement engage une réforme du régime des retraites que nous considérons, à la fois inutile et injuste, vous souhaitez ainsi prolonger l'âge de départ à la retraite, le reporter, pardon, dans le seul but de réaliser des économies 8 à 9 milliards d'euros estimés sur 5 ans, fini la réforme des retraites dites systémiques, dont on nous parlait dans le précédent quinquennat qui était présenté comme une mesure d'équité de progrès etc, elle n'a plus aujourd'hui la réforme des retraites qu'un seul objectif, et il est comptable boucher les trous de votre politique de l'offre menée à marche forcée, le goût, le rôle de la gauche de le dire, tout au long du quinquennat qu'une autre politique est possible, remettant les choses à l'endroit ne privant pas l'état de recettes indispensables, redonnant à notre pays les moyens de ses ambitions sans aggraver le déficit public, par le rétablissement d'une fiscalité équitable entre les revenus du capital et du travail par la réduction progressive des niches fiscales qui devraient être évalués conditionnés pour être maintenu par l'arrêt des baisses d'impôts, d'où nous n'avons pas les moyens, encore moins avec la remontée rapide des taux d'intérêt et par la mise en place sans attendre d'une taxation exceptionnelle sur les profits, enfin, cette loi de programmation, elle souffre d'un manque de crédibilité, beaucoup diront que c'est la loi du genre et qu'aucune loi de programmation des finances publiques n'est jamais respecté, mais en l'occurrence dans son entêtement à vouloir réduire le taux de prélèvements obligatoires et, surtout, a refusé de faire participer à l'effort national, les plus riches et les grandes entreprises, le gouvernement ne parvient pas dès le départ, à établir une stratégie convaincante de rétablissement des comptes publics, c'est le Haut Conseil des finances publiques qui le dit lui-même, en qualifiant la trajectoire de peu ambitieuse et particulièrement fragile car elle s'appuie sur des hypothèses très et donc trop optimiste alors en commission, la majorité sénatoriale a certes un peu modifié la trajectoire en l'aggravant de notre point de vue sur les dépenses, mais n'a pas révélé de désaccord majeur sur le fond avec le gouvernement, il reste même chers collègues une certaine ambiguïté sur la question des collectivités locales, avec la suppression de l'article 23 mai en maintenant l'objectif de baisse des dépenses des collectivités locales sur lesquelles vous alignez l'État lui-même, vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous y reconnaître Messieurs, Monsieur le Ministre, pardon monsieur le rapporteur général, vous l'avez compris le groupe socialiste, écologiste et républicain ne soutiendra pas ce texte, ni dans sa version gouvernementale ni dans sa version sénatoriale, nous avons des propositions à faire, de justice fiscale, nous, je les ai fait tout à l'heure, j'ai entendu que Bruno Lemaire disait et des mois pour faire de la justice fiscale, j'ai considéré que c'était pas de l'humour et que nous essayons, mais enfin il faut quand même nous aider à vous aider, plutôt que d'appeler simplement à la rescousse ce côté-là de l'hémicycle, nous ne nous ne soutiendrons pas ce texte, puisque cet effort de justice fiscale n'a pas été fait aussi parce qu'il est trop fragile dans ces hypothèses, parce qu'il est contestable, de notre point de vue danser orientation idéologie idéologique déséquilibré dans la répartition de l'effort inapte à répondre aux besoins du pays en matière sociale et écologique dans les prochaines années et risqué aussi, il faut le dire, quand on connaît le mécontentement social qui couve dans notre pays face aux face aux injustices, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Jérémy Bacchi pour le groupe communiste, vous avez 5 minutes chers collègues.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous venons d'apprendre le déclenchement nouveau 49 3 par la première ministre la première année de la programmation aura donc été enjambé par le gouvernement, et nous continuons de débattre, comme si de rien n'était ici au Sénat, j'aurais aimé vous dire que j'ai accueilli ce projet de loi de programmation des finances publiques avec enthousiasme, tant il aurait répondu à l'urgence dans laquelle se trouve le pays mais il n'en est rien, j'aurais aimé, a minima, pouvoir dire que ce projet de loi de programmation des finances publiques, comprenez la gravité de ce qui traversent la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, mais une fois de plus, il n'en est rien, en réalité, vous avez choisi de verrouiller l'ensemble des échelons de la puissance publique l'ensemble des parties prenantes des politiques publiques au service de nos concitoyens viennent et concitoyens dans ce projet de loi de programmation, alors que les Françaises et les Français sont de plus en plus nombreuses et nombreux à ne pas savoir comment ils vont se chauffer cet hiver alors que les Françaises et les Français voient leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil, sous l'effet de l'inflation galopante, alors que les Françaises et les Français, toujours plus nombreuses et nombreux se demandent s'ils vont pouvoir trouver un emploi ou conserver le leur, votre seule réponse c'est la réforme c'est la réforme la contre-réforme plutôt celle des retraites, du RSA de l'assurance chômage à croire que vous ne voulez pas entendre le sentiment d'injustice et le vent de révolte qui souffle dans le pays, il y a à peine 6 mois, le président de la République était élu grâce à l'ensemble des républicains de ce pays dont des millions de voix issu des rangs de la gauche, ce vote m'oblige, disait-il au soir du second tour, renchérissant par une formule déjà daté, je le cite : je sais que nombre de compatriotes ont voté pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, ce projet de loi de programmation constitue un projet d'exclusion de ses électrices, les électeurs qui l'ont porté au pouvoir, je viens à présent au projet de loi en tant que telle dans le rapport annexé à l'article 1er de ce projet de loi la capacité productive qui sous-entend la croissance serait, je cite, soutenu par les réformes du gouvernement ces dernières contribuerait notamment à accroître l'offre de travail et parvenir au plein emploi à l'horizon 2027, il s'agit en particulier de la réforme des retraites, de la réforme du RSA de la réforme du contrat cyclicité de l'assurance chômage, fin de citation, le mot est lâché plein emploi mais bien loin de monde idéal, il s'agit d'un plein emploi hypothétique, bâti, non pas sur les besoins et la croissance, mais sur la précarité et un salariat corvéables à merci, avec toujours moins de droits, d'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques dans son avis sur le projet de loi de programmation ne dit pas autre chose de votre tautologie sur l'hypothèse de, je cite : la croissance potentielle est optimiste, notamment parce que cette dernière suppose des effets importants et immédiats de réforme du Revenu de solidarité active des retraites de l'assurance chômage, de l'apprentissage dont ni les modalités ni les impacts, ni le calendrier ne sont documentés, la réforme des retraites en voulue par votre gouvernement, ni le fait que le taux d'emploi des sexagénaires et le 3ème pire, de l'Union européenne, seul un tiers des 60 64 ans est en emplois, ils sont considérés comme musées trop vieux par un patronat qui délaisse ce qui ne correspondent plus aux normes, ces travailleurs extrêmement qualifiés sont en réalité trop cher, trop cher par rapport aux jeunes d'abord un réel il main oeuvre peu qualifiée, mais surtout peu onéreuses, le niveau des salaires et votre question taboue qu'elle devrait être pardon une question politique fondamentale de la décennie qui vient, depuis le début des années 80 la part de la rémunération salariale dans la valeur ajoutée a chuté de 8, dans le pays, ce à quoi il faut ajouter les inégalités salariales dans le secteur privé qui augmentent d'au moins 5, des dizaines de milliards d'euros en salaires et en cotisations qui rendent relativement insignifiant, les économies d'une dizaine de milliards d'euros générés par le report de l'âge légal de la retraite, nous revendiquons, en plus de l'augmentation des salaires, évidemment, le partage du temps de travail comme principal levier pour financer le système des retraites, il s'agit de travailler moins longtemps dans la journée dans la semaine et dans la vie pour que toutes et tous puissions travailler pour que les conditions de vie et de dignité soit restaurée, je veux y avoir ici un mot pour ces femmes, ces hommes totalement absents de ce projet de loi de programmation et sans qui, pourtant, la France ne tournerait pas ce sont des métiers pour lesquels les politiques publiques qu'ils font qu'ils accompagnent qu'il porte, verront leur budget baisser dans les 3 prochaines années, les enseignants, les bénévoles d'associations, les aides-soignantes, les agents territoriaux, les travailleurs sociaux sont autant de professions aussi utile que mépriser, par cette programmation, les exonérations absolument massive des cotisations sociales, elles qui ne représentent aujourd'hui plus que 50 % des recettes de la Sécurité sociale, comme 82 % en 93 c'est toutes ces choses, toutes choses étant égales par ailleurs une perte de 100 milliards d'euros qui échappent aux travailleurs, je conclus d'une citation, madame la présidente, celle d'Ambroise Croizat de la sécurité sociale qui disait vivre sans l'angoisse du lendemain de la maladie ou de l'accident de travail en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses besoins, voilà où se trouve le véritable courage, bien loin des logiques austéritaires qui prévalent aujourd'hui mais n'est pas en bras croisant qui le veut, merci. Merci, la parole est à présent à notre collègue Michèle Canet être pour le groupe Union centriste. 4 minutes, chers collègues, merci. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, c'est un exercice assez ambitieux auquel nous nous attelons maintenant ambitieux parce que lorsqu'il s'agit de prévoir l'évolution des finances publiques pour une période quinquennale, bien entendu, ça reste extrêmement difficile, on le voit, on le mesure Monsieur le Ministre, parce que ce n'est pas la première fois que l'on procède à cet exercice, on l'a déjà fait en 2009 puis en 2012 puis en 2014 puis en 2017 qu'observe-t-on lorsqu'on a fait antérieurement, hé bien tout simplement, c'est qu'en fin de période quinquennale, le résultat est fondamentalement différent de celui auquel on s'attendait, rappelons-nous sur les deux trois premières lois de programmation des finances publiques, c'était à peu près 3 % de PIB de niveaux différents de lit que nous pensions atteindre dans l'objectif que nous nous fixions pour celle de 2017 endetté à 5 6 % d'écart l'année dernière par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, c'est dire : c'est dire que cet cet exercice est particulièrement ambitieux, il est légitime que nous nous fixons un cap en Bretagne on dit régulièrement que tous les marins doivent fixer un cap, hé bien il faut aussi que, qu'on puisse le faire pour nos finances publiques, nous, les membres du groupe de l'Union centriste nous sommes attachés à un certain nombre de d'objectif de préoccupations une première préoccupation qui porte bien entendu sur la question de la maîtrise des dépenses publiques, c'est quelque chose qui est absolument essentiel si l'on veut aller assez loin, nous sommes également attachés à ce que il y ait un traitement identique entre les collectivités territoriales et puis l'état, il n'y a pas de raison que seules les collectivités territoriales, par exemple, soient astreintes à l'effort et que l'État s'en exonère on a plutôt le sentiment, nous, que celui qui donne les orientations d'habitude, il faut qu'il montre le cap et qu'ils montrent l'exemple et donc ça c'est important et puis une 3ème préoccupation porte sur la question de l'endettement public et pour nous, c'est un vrai sujet de préoccupation, quand on a fait ces constats, hé bien il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut que l'on on que qu'il faut que l'on réalise bien sûr cette maîtrise des dépenses publiques, nous nous pensons que l'objectif à la fin du la période quinquennale doit être autant que possible de se rapprocher de l'équilibre des finances publiques, alors c'est un exercice difficile parce qu'il est toujours difficile d'économiser et de ne pas dépenser plus que ce qu'on a, mais c'est quand même un objectif que l'on devrait se fixer et puis, pour cela, il y a d'une part la question de la maîtrise des dépenses, mais aussi la question des recettes et on le voit bien, pour ce qui concerne les recettes, nous nous sommes d'accord avec ce qu'a dit le le ministre Lemaire tout à l'heure, il y a effectivement un niveau de prélèvements obligatoires dans notre pays qui est trop élevé, donc il faut que, on le diminue, mais il faut qu'on soit attentif à ce que les priorités soient vers ce qui est vraiment productif et force est de reconnaître, puisque nous sommes à cet Automne, au moment où on aurait dû payer la contribution à l'audiovisuel public que de supprimer cette contribution ne fut pas pour nous la meilleure des choses à faire, tout simplement parce que il eut mieux valu que l'effort portant sur la CVAE par exemple et si on n'avait pas procédé ainsi, nous pourrions effectivement soutenir une réduction significative de la CVAE mais la prudence nous conduirait à justement se dire puisque l'effort a porté sur la contribution à le de le public, il faut attendre sans doute pour la CVAE et puis il y a pour les collectivités, je l'ai dit tout à l'heure, ben la nécessité de ne pas leur demander un effort supérieur à celui qui allait être réalisée par l'État pour nous, il est important que l'effort soit partagé les collectivités sont en général très vertueux, cela a été dit avant moi, il faut que l'état le soient le plus possible, on proposera en ce sens, notamment je crois un amendement pour le FCTVA je vois le montant été écoulé, donc je vais m'arrêter, en tout cas, le groupe de l'Union centriste, votera le projet présenté par le rapporteur général. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue Monsieur Gérard Longuet pour le groupe des Républicains. madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon excellent collègue Michel Canevet a rappelé que beaucoup des lois de programmation n'avait pas été confirmée et quand on va aux résultats, il y a un écart. La vérité c'est que cet exercice est utile mais qui n'est pas suffisant et mon excellente collègue elle aussi excellente Michel Christine Lavarde m'a renvoyé le bébé en se disant mais c'est c'est très simple, puisque nous sommes d'accord pour pas nous battre sur les paramètres, parce que c'est un débat qui n'en finit plus, nous avons l'intention d'étudier votre projet de loi de l'amender et de le voter, c'est parfait, mais avec évidemment ces préoccupations qui viennent d'être rappelé qu'avait rappelé notre et que rapporteur général Jean-François Husson, faire en sorte que les efforts soient partagés puisque si on ne se bat pas sur les paramètres, au moins, reconnaissons qu'il ait à un effort d'équilibres dans les des efforts d'équilibres pour administrations publiques centrale le évidemment les collectivités locales et le social, alors la question : et ben 25 milliards, vous trouvez ça beaucoup car en bout de parcours, on arrive en effet à 25 milliards alors comme j'ai peu de temps je vais vous dire l'essentiel, l'essentiel c'est que premièrement sur le marché du travail, vous avez six mesures de réformes qui sont intéressantes, les retraites, évidemment, le RSA l'indemnisation du chômage, vous avez également prévu l'apprentissage Pôle emploi est important pour les jeunes ménages la jeune enfant le contrat jeune enfant enfant Petite enfance pardon,

Une partie de ses 8 points d'écart avec ces mesures-là on dégage de l'argent, dégage de la marge parce qu'évidemment, des gens qui travaillent, ça rapporte et ça rapporte à tout le monde et notamment à l'État, le 2ème sujet c'est naturellement l'énergie, et alors là, il y a qu'une seule solution : arriver à obtenir de l'Union européenne, qu'elle cesse de un marché unique où l'on met sur le même plan l'électron fossiles et l'électron décarbonnées et si la bataille essentielle que votre gouvernement doit livrer parce que si nous avons un électron décarbonnées vous allez pouvoir mettre fin une machine, une espèce d'usine d'une complexité effrayante qui consiste à aider les hein, parce que la taxe carbone parce que le le noeud de la volonté de faire des énergies renouvelables, qui ne soit pas nucléaire non séparer les deux et il y aura un électron décarbonnées et à ce moment-là, les investisseurs n'auront pas besoin de subventions pour pour investir, parce qu'ils auront des éléments fixes en effet l'électron décarbonés a une particularité, c'est qu'il n'est pas sensible aux éléments extérieurs alors que l'électron carbonées issues du fossile et totalement dépendants de marchés internationaux et, naturellement, des des relations monétaires, ça c'était la 2ème idée la 3ème idée c'est de tenir compte simplement de la démographie, il y a, hélas, dans notre pays une diminution de 10 % des classes d'âge, et là je le poserai demain en commission des finances, une épreuve de vérité pour un certain nombre d'administrations et au 1er rang d'entre elles, l'éducation nationale, nous ne pouvons, on doit faire du qualitatif, parce que nos jeunes ne sont pas assez formés, les classements internationaux sont sévères pour nous mais on aurait pu faire de quantitatif et c'est un vrai sujet et cela peut dégager des marges sur le 1er budget civil de l'État 60 milliards d'euros, ah si on ne gagne pas un peu pour nourrir les 25 en fin de parcours, c'est que vraiment n'est pas bon 4ème et dernière proposition d'économie. La productivité du service public, une chose que je ne comprends pas le même président avec le même enthousiasme en 2017 proposé moins 50000 emplois publics en cinq Il a, il est réélu. Ben non, il y a plus rien, comme si il n'y avait plus de productivité possible, là vous êtes dans un ministère qui pratique la productivité et vous avez certainement de toutes les administrations centrales de l'État, vous êtes à la tête d'une administration qui a su à la fois maintenir un service et adapter les effectifs sans trahir les administrés, hé bien je crois qu'il faut reprendre cette question de la productivité du service public, ce n'est pas injurieux, ce n'est pas déshonorant, il y a des façons différentes de travailler et nous devons entrer dans le détail les ministères doivent être dirigées par des ministres qui ont le souci de la réalité de l'efficacité en revanche une question. Nous avons ce cette loi de programmation et on annonce une loi de progression militaire, l'ancien ministre de la Défense, que je suis, se félicite de l'intérêt. Mais, s'interroge le membre de la commission des finances s'interroge sur la compatibilité de l'un et de l'autre, puisque les sommes avancées sont spectaculaires : la situation internationale peut l'expliquer, mais il serait intéressant que vous assuriez une coordination dans la même semaine entre les efforts d'économie et les annonces de dépenses, le débat parlementaire y gagnerait en clarté. La La parole est enfin au président monsieur Vincent De La Haye pour le groupe Union centriste. madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, en général, j'aime l'optimisme. Mais en matière de gestion de l'argent public, je pense que l'optimisme et souvent dangereux. Pour ai pour bien gérer l'argent public, il faut être rigoureux et prudent. Vos prévisions de croissance Monsieur le Ministre, sont très optimistes, elles sont très supérieurs à ce que l'on a constaté sur la les 2 dernières décennies et à ce que prévoit le consensus des économistes. Je pense que ce n'est pas prudent, bien sûr, ça gonfle artificiellement les recettes futures mais ça n'est pas prudent aux prévisions ne sont pas sincères, vous mélangez les dépenses courantes et dépenses exceptionnelles qui sont liées à vos choix de gestion de la crise sanitaire et de la crise énergétique. Je vous avez pourtant demandé Monsieur le ministre, en commission des finances de bien vouloir distinguer à partir de 2023 et pour les années suivantes, ce qui était du courant de l'exceptionnel et là, vous mélangez tout allègrement et vous faites croire que la dépense publique baisse alors qu'en fait ce sont que les dépenses exceptionnelles qui baissent et que les dépenses courantes, elle augmente de façon importante, donc pour moi, elles ne sont pas sincères ses dépenses. En plus, elle ne sont pas juste vos prévisions de sont pas juste parce que, en réalité, vous demander un effort aux collectivités théâtre territoriale que vous n'imposez pas à l'État, et quand on regarde les dépenses courantes, les dépenses courantes augmentent fortement, et les dépenses des ministères augmente aussi fortement, donc nous aimerions bien que l'État s'impose le même effort que celui qu'il demande aux collectivités, ça ça serait juste. Et puis ensuite, vos prévisions pour moi ne prépare pas bien à l'avenir, quel est le problème numéro un de notre pays aujourd'hui, c'est de produire le plus vite possible un maximum d'énergies décarbonnées je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, on nous annonce des coupures cet hiver, on sait que pour l'industrie, c'est indispensable pour notre compétitivité, c'est indispensable pour nos concitoyens, c'est indispensable, donc il faut en produire le plus vite possible, pour moi, il faudrait un véritable plan Marshall de l'énergie aujourd'hui et dans vos prévisions, il n'y a quasiment rien quasiment rien pour les 5 prochaines années sur ce sujet, moi je suis effaré. Donc. Pas prudent pas sincère, pas juste préparant mal l'avenir comme vous voulez-vous qu'on accepte votre programmation financière alors heureusement et je salue le travail du rapporteur général et la commission des finances, heureusement nous allons profondément modifié ce texte. C'est une chance, mais ma conviction reste la même : on fonce dans le mur et on accélère encore pour moi, c'est suicidaire. Donc, Monsieur le Ministre, je pense qu'il est grand, grand temps de changer de politique budgétaire et pour cela je vous ai apporté un cadeau. Ce que je vais vous remettre un livre sur les vertus de l'équilibre ou l'anti-quoiqu'il en coûte, je pense que sa lecture vous sera utile, c'est un très bon auteur merci Gérard Longuet et je pense vraiment que vous verrez à travers ce livre que les pays dont les économies se porte mieux que la nôtre, et il y en a quand même à quelques-uns toutes ses économies, toutes ces pays ont des finances saines, donc je pense qu'il est grand temps de reprendre cette ligne et de la suivre, pour les années prochaines voilà. Merci de m'avoir écouté. La discussion générale est Close, je vous laisse remettre le livre au Ministre mais je vais donner la. Par le au ministre pour réponse Monsieur le Ministre, si vous voulez répondre aux différentes Pardon, madame la présidente, on hésitait à demander une suspension de séance pour que je puisse lire le livre avant de vous répondre, mais je le lirai un peu plus tard dans la soirée, en tout cas merci à tous les orateurs qui se sont. Exprimez c'est un beau débat, c'est un débat riche que nous avons commencé à voir et que nous allons continuer à avoir, moi ce que je veux retenir d'abord, c'est que j'ai entendu une majorité d'orateurs reconnaître, en tout cas, s'inscrire dans un objectif d'assainissement de nos finances publiques est de retour à une trajectoire plus maîtrisé, d'équilibre, c'est d'abord ça que je veux reconnaître, ensuite il y a un débat effectivement sur le rythme, c'est vrai que nous prévoyons un rythme de retour à sous les 3 % à horizon 2027, c'est ce que nous avions annoncé pendant la campagne présidentielle, stabilisation de la dette en 2026 retour sous les 3 % en 2027 plusieurs orateurs parmi vous, c'était notamment le cas de du sénateur kaput c'était le cas également d'autres sénateurs ont insisté sur le fait que ce rythme nous plaçait madame Lavarde je crois parler de mauvais élève en tout cas en queue de peloton dans le calendrier-t-elle. Que les différents programmes de stabilité pacte stabilité ont annoncé un retour sous les 3 % c'est vrai, c'est vrai que les derniers pays européens avant nous et notamment l'Espagne annonce un retour sous les 3 % à horizon 2025, là où nous prévoyons un retour sous les 3 % à horizon 2027. Il faudra voir quand même au moment de la présentation des prochains P. stable si ces trajectoires sont toujours les mêmes, nous avons l'occasion à plusieurs reprises de réactualiser nos prévisions, avec notamment la présentation du PLF et autres, je suis pas sûr que cela soit le cas dans tous les pays, qu'un certain nombre de pays, après avoir présenté leur programme de stabilité, ont annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre l'inflation, de bouclier tarifaire, il faudra voir s'il prévoit toujours le même calendrier de retour sous les 3 %. Mais de toute façon nous assumons, nous assumons de dire que plutôt qu'une politique brutale d'austérité budgétaire, nous préférons un retour maîtrisé planifié sous les 3 qui tire les enseignements aussi de certaines politiques qui ont été menées dans d'autres crises par le passé, notamment après la crise 2008 2010 ou à vouloir établir trop brutalement et trop rapidement les finances publiques ont fini par casser la dynamique de croissance et une fine et à créer du chômage en plus et donc des recettes en moins pour les finances publiques et donc des déficits et une dette qui s'accroît, on assume de dire qu'on veut que le retour sous les 3 % et le rétablissement de nos comptes publics soit compatible avec l'activité économique. On a vu en 2021 qu'on avait une croissance locomotive en Europe on voit en 2022 qu'on a une croissance qui résistent et qu'on a une économie qui résiste remarquablement madame Lavarde a cité les 3 dimensions importantes, consommation, investissements, commerce extérieur, vous ne vous êtes pas beaucoup attardé sur l'investissement, je pense, pour ne pas relever le fait et c'est l'Insee qui l'a salué, que l'investissement repart continue à progresser assez nettement au dernier trimestre 2,8 % dans notre pays, ce qui est un signe positif, encore une fois, je ne dis pas ça pour le mettre au crédit du gouvernement, je le mets au crédit de toutes les femmes et tous les hommes qui investissent et qui entreprennent dans notre pays et qui permettra à notre économie de tenir, qui permettent d'embaucher des Français d'investir, de stimuler l'activité économique et donc les recettes pour notre pays parce que oui Monsieur Féraud, nous avons assumé de baisser la pression fiscale sur les entreprises, mais nous collectons davantage de recettes fiscales venant des entreprises depuis que nous avons baissé les taux, nous avons passé l'impôt sur les sociétés de 33 % à 25 % ces 5 dernières années on collecte plus d'impôt sur les sociétés à 25 % qu'on en collecter à 33 on est en train de faire la démonstration que quand vous taxez moins un gâteau qui grossit, vous gagnez plus que quand vous surtaxés un gâteau qui se rétrécit parce que vous le surtaxer c'est ça qu'on est en train de démontrer, donc oui, nous assumons de vouloir continuer à baisser la pression fiscale qui pèse sur l'activité économique, c'est aussi ce qui permet à l'activité économique de continuer à se développer et, in fine, et qui nous permet d'obtenir des recettes supplémentaires, alors on voit il y a une proposition d'une autre ligne qui est défendu par la majorité sénatoriale qui est de dire : allons beaucoup plus vite dans le rétablissement des comptes, beaucoup plus vite dans le rétablissement des comptes, c'est-à-dire autour, sur les 3 pour 100 2 ans j'ai entendu Madame l'Avare défendre cette trajectoire, je redis, hein, cette trajectoire elle implique 25 milliards d'économies supplémentaires à trouver non pas en fin de période, monsieur Longuet, mais en 2025, il se trouve qu'il y a dans cette loi de programmation des finances publiques à l'article 12 la programmation des missions budgétaires de l'État à horizon 2025 et donc je pense qu'en toute cohérence, parce que vous défendez, 25 milliards d'économies en plus à horizon 2025 que vous pourriez amender cet article pour dire où vous prenez les 25 milliards d'économies est-ce que c'est sur la défense est-ce que c'est sur l'éducation nationale est-ce que c'est sur la transition, écologie, j'ai entendu les propositions qui ont été faites et moi je le dis vraiment hein, moi je suis favorable à ce qu'on fasse le plus d'économies possibles et j'ai dit en en en entrée de ces débats, que si on ressort de l'examen de cette LPFP dans les différentes lectures dans les différentes chambres, on ressort avec un compromis qui conduit à ce que les l'État rehausse le niveau d'effort prévu par rapport à ce qu'on avait proposé dans le texte initial mais en serai le 1er ravi, je pense juste qu'il faut que ce soit crédible et soutenable par rapport à ce qu'on est capable de faire, j'ai entendu les pistes que vous avez évoqué, monsieur Longuet oui, évidemment, que la réforme des retraites, la réforme du RSA, la réforme de l'assurance-chômage, la réforme de Pôle Emploi, le service public de la petite enfance, ont vocation à nous permettent de rétablir nos finances publiques, certaines, pour certaines de ses réformes, elles permettent des économies budgétaires directes des fois la réforme des retraites, par exemple, pour d'autres, en tout cas pour la totalité d'entre elles, elles permettent d'élargir le marché du travail, le taux d'emploi dans notre pays et donc des recettes supplémentaires, mais elles sont intégrées dans la programmation des finances publiques dans le texte du gouvernement, ça nous est d'ailleurs reproché régulièrement par la partie gauche de cet hémicycle, ou de celui de l'Assemblée, qui nous disaient régulièrement vous intégrez dans votre trajectoire les bénéfices de réformes, ils n'ont pas encore été adoptée notamment sur la réforme des retraites, mais tout cela est déjà intégré dans la trajectoire et donc les économies supplémentaires ou les recettes fiscales supplémentaires que vous appelez de vos voeux, elles doivent être trouvées par d'autres réformes que celle-ci, qui sont d'ores et déjà intégré mais je vous rejoins totalement sur le fait que si on avait le même taux d'emploi que nos voisins allemands, moi j'aurais beaucoup moins de travail et on se poserait beaucoup moins la question de savoir comment est-ce qu'on équilibre de nos finances publiques, si on avait huit a dit point de plus en taux d'emploi dans notre pays, évidemment que la question des finances publiques se poserait dans des termes bien différents, parce qu'on aura des recettes supplémentaires et qu'on équilibreraient davantage. La réforme des retraites, elle vise à améliorer le taux d'emploi, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage, la réforme du lycée professionnel qu'on engage elle vise aussi à améliorer le taux d'emploi, notamment chez les sur les jeunes générations, ça vise à faire en sorte qu'il y ait plus de français au travail dans notre pays et donc plus de recettes pour les finances publiques. Pour la sécurité sociale, sur la question de la décorrélation prix l'électricité, prix du gaz, on est totalement aligné avec ce que vous appelez de vos beuh on veut on mène ce combat au niveau européen, c'est pas facile, mais je crois qu'on progresse, je suis pas immédiatement en charge de ce dossier là, j'écoute ce que me disent mes collègues Bruno Lemaire et Agnès Pannier-Runacher je crois qu'on progresse, de ce point de vue là avec le dernier Conseil européen a permis quand même de dessiner certaines avancées, notamment dans un 1er temps un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité, ce qui serait quand même une première marche importante et particulièrement utile sur la démographie, oui, il faut en tenir compte, on en tient compte, dans la programmation, c'est vrai qu'il va y avoir 500000 élèves de moins dans l'éducation nationale dans les 5 ans qui viennent, 500000 élèves de moins, on a connu ces dernières années une un boom démographique, on les on arrive là dans le creux de la vague et donc 500000 élèves de moins dans l'éducation nationale on veut maintenir et même continuer à améliorer le taux d'encadrement pour nos élèves, je pense que pour le coup, dans tous les départements, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans toutes les circonscriptions, s'est demandé quand même de pouvoir garder un taux d'encadrement important pour les élèves mais tout en faisant ça, évidemment, que, il y a un certain nombre de marche qui se retrouver, c'est intégrer dans la trajectoire que nous avons proposé sur la productivité du service public, comme vous l'avez appelée ou la réduction du nombre de fonctionnaires, c'est vrai, je l'assume, qu'il y a eu, pour le coup, un changement de logique par rapport à 2017, c'est vrai qu'en 2017, je me souviens, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron et s'est engagé sur un objectif avec un nombre de fonds que de postes de fonctionnaires qu'ils seraient supprimés dans le quinquennat et puis on a assumé après la crise des gilets jaunes de dire que nous n'avions plus d'objectif de nombre de suppressions à attendre, mais que nous devions engager des réformes qui permettrait ensuite de dégager des marges de postes de fonctionnaires, le prélèvement à la source, ça a été ça : la suppression d'un certain nombre d'impôts nous permet aussi de trouver des marges mon ministère, celui de Bercy, je crois que c'est 4 ou 6 % de l'emploi public, c'est 80 % des efforts de réduction de l'emploi public, ces 10 dernières années, donc on sait ce que c'est que de faire des efforts en matière d'emploi public mais on le fait après des réformes de modernisation qui permettent de dégager ses marges et c'est vrai qu'en 2022, le président de la République ne s'est pas engagé sur un nombre de postes de fonctionnaires à supprimer, il y a une candidate et en l'occurrence la candidate DLR qui s'y est engagé, mais sans vraiment dire à mon sens, ou est-ce que ces postes seraient retirés mais le président de la République ne s'est engagé, au contraire, moi c'est le mandat qui m'a été donné à une stabilité de l'emploi public sur le quinquennat il a un certain nombre de créations importantes qui sont prévues en 2023, notamment dans le secteur régalien mais le mandat qui nous a été confié, c'est stabilité de l'emploi public sur le quinquennat ce qui ne veut pas dire qu'on bouge pas, on va créer 8500 postes dans la justice 8500 postes de policiers et de gendarmes, ça veut dire pour atteindre une stabilité qu'il faut en supprimer ailleurs et donc cet effort là va être fait, mais notre logique, c'est plutôt d'avoir des postes davantage dans les territoires déconcentrée des administrations centrales, donc moi j'entends qu'il y a des efforts qui peuvent être faits en la matière. Si je schématise un calcul 10000 postes de fonctionnaires, ces 500 millions d'euros, donc si on veut atteint des montants d'économie tels que ceux que vous évoquez, ça fait beaucoup de postes de fonctionnaires à supprimer, en Net, pour le coup, donc je suis pas sûr que cela soit suffisant, mais il faut évidemment tout je voulais dire un mot sur la question des prévisions qui sont prévues dans ce dans ce texte, c'est évidemment toujours difficile, la prévision c'est un art qui fait l'objet de controverse on peut enfin, on peut discuter longtemps des prévisions, vous me direz qu'elles sont trop optimistes trop ambitieuse, moi je vous dirais qu'elles sont réalistes étayer mais à la fin, ce qui fait la croissance telle qu'elle se réalise, c'est ni les prévisions, ni les politiques ou les experts, qui en débattent l'année précédente, c'est la confiance pour notre secteur économique pour nos entreprises qui sont capables d'investir, de produire et d'embaucher et ce dont je suis absolument sûr, c'est que les prévisions de croissance que nous portons aussi optimiste ou volontariste soit-elle, ne se réaliseront pas si nous ne poursuivons pas dans notre politique pour redonner des marges à nos entreprises pour qu'elles puissent investir, produire et recruter, d'où la suppression de la CVAE qui est prévue dans le PLF qui est extrêmement importante, d'où la poursuite. De nos mesures en faveur de l'emploi, de la formation et de la compétitivité je crois que j'ai fait le tour, peut être un mot sur les collectivités locales, on aura l'occasion d'y revenir au moment des discussions sur l'article 16 et sur l'article 23 il me semble, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait dans la discussion parlementaire un rééquilibrage qu'un plus grand équilibre dans l'effort demandé à l'État par rapport aux collectivités locales dans le texte du gouvernement, il est prévu une baisse de 0 4 % pour l'État en volume sur le quinquennat de 0 5 % pour les collectivités en volume sur le quinquennat vous avez proposé une première chose, c'est dire on fait 0 5 pour l'État 05 pour les collectivités locales, moi je suis très ouvert à ça, ça nécessite un effort supplémentaire pour l'État, mais je pense qu'on doit être capable de l'assumer. Mais ce que vous dites aussi et c'est ça ou, ce qui implique de trouver 25 milliards d'euros, c'est que l'effort des dépenses de maîtrise des dépenses de l'État doit se faire sur des dépenses qui ne concerne pas la relance ou la crise on demande pas la même chose aux collectivités locales dans la copie qui, pour qui elle les dépenses relatives à la crise et à la relance, sont prises en compte dans le calcul est donc derrière un apparent équilibre entre l'État et les collectivités locales, il y a en effet un très grand déséquilibre puisque ça veut dire que les dépenses de l'État sur les 5 années qui viennent dans la copie qui est proposé par la commission des finances augmenteront de 1 virgule 5 % en valeur, là où elles augmenteront de 10 % en valeur pour les collectivités locales. ça veut dire par ailleurs qu'il faut trouver, je le redis, 25 milliards à horizon 2025, 37 milliards à horizon 2027. Il s'agit pas, encore une fois, de dire qu'on va imposer une austérité aux collectivités locales, ça, on a vu ce que c'était sous le quinquennat Hollande avec les baisses brutales de DGF, j'ai entendu tout à l'heure monsieur broyeur dire vous allez baisser les dépenses de fonctionnement des collectivités non dans la copie telle qu'elle est présentée par le gouvernement dans la LPFP, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, elles augmentent de 21 milliards d'euros sur les 5 années qui viennent, elles augmentent de 21 milliards d'euros s'agit pas de dire qu'elle baisse, elles vont continuer à progresser dans la copie que nous avons proposé nous mettons un cadre pour l'État et pour les collectivités locales de maîtrise dans la durée. Vous appelez à soutenir, vous dites, vous, vous avez dit : vous devriez soutenir les collectivités locales, enfin nous on n'a pas fait des baisses brutales de DGF massive, comme ça a été le cas sous le quinquennat de François Hollande et à l'époque, les écologistes faisait partie de la majorité de François Hollande on a sanctuarisé la DGF depuis 5 ans, alors on l'a sanctuarisé au niveau global et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires qui viennent ensuite vous voir et qui vous disent : vous dites que vous avez sanctuariser la DGF mais moi ma DGF baissé, il trouve que je suis partie des quelques membres du gouvernement qui sont élus locaux je, je, je, j'ai pas eu la chance ou l'honneur d'être maire, je ne suis, je suis un modeste conseiller municipal depuis près de 10 ans et c'est vrai que j'ai pu voir que moi dans ma commune, quand bien même nous avons sanctuarisé la DGF depuis 5 ans la DGF a légèrement baissé du fait de la péréquation précisément ce que nous proposons dans le PLF pour 2023, c'est historique, c'est 320 millions d'euros en plus pour neutraliser les effets de la péréquation, ce qui veut dire qu'en 2023 pour la première fois depuis 13 ans, la DGF de 95 % des communes augmentera 95 % des communes, c'est inédit et historique pendant la crise sanitaire, il y a eu 10 milliards d'euros de transferts de l'État aux collectivités locales, ces 5 dernières années, les concours financiers de l'État aux collectivités locales, augmenté de 5 milliards d'euros, franchement, on a vu plus grande maltraitance des collectivités locales que ces 5 dernières années, il faut avoir l'honnêteté quand même de le dire et j'entends les comparaisons sur le déficit de l'État par rapport à celui des collectivités locales qui ne font pas de déficit qui représentent une part de la dette qui est plus faible, mais enfin, le déficit de l'État, la dette de l'État qui s'est accru au moment du quoi qu'il en coûte, il a aussi permis aux collectivités locales d'avoir moins de dépenses à effectuer quand on fait le quoi qu'il en coûte, on évite à des centaines de milliers d'entreprises de se casser la figure et donc il y a des dépenses sociales pour les collectivités locales, si on avait retrouvé des millions de Français plonger là dans la précarité, des dépenses sociales qui aurait explosé pour les collectivités locales, donc l'investissement du quoi qu'il en coûte oui qui a a alourdi le déficit de l'État et la dette de l'État, ben, c'est aussi un investissement qui a évité des dépenses pour les collectivités locales et on l'assume totalement parce que notre conviction, c'est qu'il ne faut pas opposer l'État et les collectivités locales, comme s'il y avait l'un contre l'autre mais que c'est l'un avec l'autre et qu'on a les mêmes objectifs a priori les mêmes intérêts, les objectifs et désintéressés, quoi, c'est de permettre à notre pays de continuer à investir, on a besoin d'investir, face à la transition écologique, on a besoin d'investir, face à la transition démographique, si on veut avoir les marges de manoeuvre pour investir et ce qu'il faut laisser filer les dépenses se retrouver avec des taux d'intérêt qui explose et donc un État privé de marge de manoeuvre et des collectivités locales, elles-mêmes, privé de marge de manoeuvre pour investir, si vous avez des taux d'intérêt qui explose, non, on a plutôt intérêt, État et collectivités locales à affronter le défi de la transition écologique de la transition énergétique de la transition démographique numérique en investissant massivement et pour investir, il faut qu'on ait des marges de manoeuvre et pour avoir des marges de manoeuvre, il faut maîtriser suffisamment nos dépenses de fonctionnement, État et collectivités locales pour avoir des taux d'intérêt soutenable pour être capable d'emprunter pour investir, c'est ça la logique comporte, ça n'est rien d'autre que ça, c'est de main dans la main avec les collectivités locales de. Capable de bénéficier des marges de manoeuvre suffisante, enfin je voulais répondre à Monsieur Bakhit sur la question des investissements sociaux et notamment pour un certain nombre de professions que vous avez salué qui sont très engagés dans d'autres pays, vous avez cité, notamment les enseignants et les aides-soignants en disant qu'ils sont méprisés. Moi, je veux quand même rappeler que le séjour de la santé dans son volet revalorisation, c'est l'augmentation salariale la plus forte qu'a connu l'hôpital public dans son histoire sur un temps aussi court. C'est près de 200 euros Net en plus par mois pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital, ces 10 milliards d'euros d'investissement pérenniser pour la revalorisation des salaires pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital, vous avez cité les enseignants dans le projet de loi de finances pour 2023, on prévoit une augmentation de 10 % pour tous les enseignants à la rentrée de septembre 2023 j'ai pas souvenir dans un passé récent ou lointain qu'il y a eu une telle augmentation de 10 % sur une année et on prévoit même 25 %, en plus, ça sera dans les années qui viennent pour des enseignants qui accepteront de s'engager dans des missions supplémentaires qui sont en train d'être défini en concertation avec les représentants des enseignants par le ministre de l'Éducation nationale, je, encore une fois, il y a beaucoup de Français qui sont en difficulté, oui il faut continuer, il faut soutenir davantage nos enseignants, mais dire qu'ils sont maîtrisés mépriser quand on a 6 milliards d'euros de revalorisation salariale pour nos enseignants 10 pour 100 dès l'année prochaine, encore une fois, ça me semble aussi pas totalement adaptées à la réalité des faits mais tout ça, nous aurons l'occasion d'en débattre aussi, à l'occasion du PLF. Merci, nous allons commencer la discussion du texte. Je vous rappelle que je suspendrai à 20 heures et que nous avons 74 amendement monsieur Savoldelli, vous avez demandé la parole sur l'article 1er.

On va au sénat débattre avec l'entrée du 49 3 qui clôture complètement le débat sur la loi de finances à l'Assemblée nationale. Ah, mais ça peut soulevé un enthousiasme de de certains ici et vous savez ce que ça veut dire, Roger Karoutchi, ça veut dire que l'exécutif va choisir et déconstruire des amendements qui ont été votées, y compris dans vos rangs, y compris dans vos rangs, donc on s'est quand même une situation un peu ubuesque, on va débattre ici au Sénat de la loi de programmation de finances, qui est la trajectoire pour les années à venir et on utilise le 49 3 pour clôturer définitivement le débat à l'Assemblée nationale et des tricoter, détricoter des amendements venant de différentes sensibilités à l'Assemblée nationale, ça c'est des conditions alors qu'on nous a dit tout à l'heure et des nous et il y a l'esprit de responsabilité, on nous a parlé de courage politique. Enfin, vous êtes des incompris ou si vous étiez s'y compris que ça Monsieur le Ministre, vous utilisez pas la batterie des 49 3 donc on trouve nous, notre groupe qu'on débat dans des conditions extrêmement précaires et que il y a des questions de sincérité politique qui sont posées, je le dis c'est dit et entendu. Merci de nous passons à l'amendement numéro 26 Monsieur Savoldelli. C'est une suppression d'articles, madame la présidente, que le le ministre.

il a déposé 24 amendements qu'signe de travail et de responsabilité néanmoins là je m'adresserais plutôt au rapporteur général qui a décidé de laisser passer cet article, et là je vous avoue un peu notre stupéfaction. Le rapporteur général, nous dit le motif les hypothèses macro-économiques sont trop optimistes, là, je le suis, nous le suivons, il pourrait être justifié de modifier le rapport annexé ainsi que l'ensemble du scénario macroéconomique sous-jacent, le rapporteur ne souhaite pas aller dans cette direction car une telle révision du scénario nuirait à la clarté du débat entre le gouvernement et le Parlement, fin de citation. Je crois, monsieur le rapporteur général et mes chers collègues de la majorité sénatoriale que vous avez, par cette position, empêcher un débat libre et éclairé ou modifier les trajectoires des sols, des administrations publiques à l'article de mais vous le positionnez pas sur les agrégats économiques qui vous paraissent infondées, d'ailleurs, j'espère que vous allez nous l'expliquer, j'aimerais savoir si la droite sénatoriale, soutient l'ensemble des réformes dites structurelles du gouvernement si c'est le cas, dont acte, respect, pas de problème, la seule intention qui a été la vôtre en commission a été de durcir les prévisions du solde structurel pour le ramener à un virgule 7 en 2027 contre 2 9 dans le projet initial du gouvernement et pour que tous et touche puis suivent ce que ça implique, j'avance une définition le sol budgétaire structurel ou sous-jacent, et la différence entre les recettes et les dépenses publiques, corrigé des effets imputables aux cycles économiques aux événements ponctuels, cet indicateur faire ressortir les tendances structurelles afin de déterminer si la politique budgétaire d'un pays est expansionniste neutre ou restrictive pour une période donnée, c'est un indicateur qui est controversée, mes chers collègues, et vous le savez, il a été controversée, nombre de fois le déficit structurel est estimé à 2 8 % du PIB par la Commission européenne et de de par le gouvernement, nous nous demandons la suppression de cet article. Merci, monsieur le rapporteur pour avis. mais si on veut également l'idée, c'est de dire : on part de cette copie, elle est finalement le point d'entrée et de référence qui nous permet, au fur et à mesure d'ailleurs des débats et des articles d'apporter notre éclairage et surtout la position avec une nouvelle trajectoire, donc ça n'est pas approuvé la copie, c'est s'en servir de base dans la discussion, tout au long de cette loi de programmation des finances publiques et je confirme donc l'avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre défavorable. Oui : avis défavorable également cet article, hein, il ne prévoit que la ratification du rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques, sa suppression entraînerait de facto l'inconstitutionnalité de la loi de programmation des finances publiques, ce qui est je pense souhaitée par très peu de monde ici mais vous avez proposé une question préalable, donc ça va aussi dans cette, dans ce sens-là du rejet du texte que vous portez avec une certaine cohérence, mais évidemment, nous y sommes défavorables, je voulais simplement répondre à votre intervention, la décision de déclencher le 49 3 sur la partie de du PLF à l'Assemblée nationale. Ne remet aucunement en cause la lucidité où la qualité des débats que nous avons ici. Il y a un texte adopté à l'Assemblée nationale, sauf si une motion de censure était votée dans les 48 heures dont vous serez saisis pourquoi est-ce que le 49 3 a été déclenchée, parce qu'hier, les oppositions ou avant-hier, les oppositions se sont réunis pour supprimer au quasi, supprimer le bouclier tarifaire en 2023 qui permet de protéger les Français face à l'envolée des prix. Il n'y a pas de bouclier tarifaire en 2023 la facture d'électricité et de gaz à augmente de 120 % 120 % on met en place un bouclier tarifaire est ce que les oppositions avaient voté, c'est on prend tout l'argent du bouclier tarifaire pour le mette sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur 2023, or on sait très bien qu'on ne pourra pas multiplié par 7 en un an, les rénovations énergétiques, ne serait-ce que pour des capacités opérationnelles pour nos artisans et la filière BTP de le faire et surtout ça veut dire 600 euros d'augmentation de la facture d'électricité pour les Français l'an prochain, donc en responsabilité, oui nous avons réaffirmé notre souhait de vouloir protéger le pouvoir d'achat des Français l'an prochain avec le bouclier tarifaire et déclenché le 49 3 mai nous aurons des débats nourris rapidement sur le PLF ici. Monsieur le Président, Karoutchi pour explication de vote. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, bien entendu, sur l'amendement lui-même je partage pleinement l'avis du rapporteur général, mais je voulais juste en profiter pour dire à monsieur le Ministre, bon évidemment 49 3 on peut toujours dire c'est là tu sais là tu répondais de manière constitutionnelle ne vous cassez pas la tête, c'est comme ça, je veux dire, vous n'avez pas de majorité, vous n'avez pas de majorité, moi j'ai été dans un gouvernement qui, pendant 5 ans, n'a jamais utilisé le 49 3, jamais vous vous n'avez pas de majorité, alors cette fois-ci c'est ça la fois prochaine sera autre chose, mais c'est comme ça, c'est la règle constitutionnelle, je suis désolé pour Nathalie ça lol Savoldelli mais la Constitution prévoit un quart neuf trois on la réduit en 2008 aux textes budgétaires à une fois le reste de la session, c'est comme ça, après le travail du Sénat, heureusement, n'est pas lié en Direct au travail de l'Assemblée nationale, ensuite il y aura des commissions mixtes paritaires, on verra, mais le travail du Sénat, le travail de la commission des finances du Sénat, le travail de l'ensemble des sénateurs, c'est de prendre un texte qu'il plaise ou non, de l'améliorer, de l'amender, de le transformer et de donner une majorité à ce texte qui peut ne pas être une majorité favorable au gouvernement et ce texte peut ne pas plaire au gouvernement il y a pas de 49 3 au Sénat, alors je suis bien d'accord, on sait bien qu'au terme, le dernier mot est à l'Assemblée nationale, mais alors, pardon monsieur ça vol délit, c'est le cas pour tous les textes, c'est le cas depuis 50 ans, 60 ans, et ça n'a pas changé le, le, la manière de fonctionner, on peut faire une réforme constitutionnelle, je suis favorable d'ailleurs à une réforme ou ou sur certains textes, il n'y aurait pas le dernier mot seulement à l'Assemblée nationale, mais en tout état de cause, on lui ait pas aujourd'hui, appliquons la Constitution, on fait notre travail convenablement correctement avec une majorité et sur l'amendement en question, il est évident que si on vous suivez bah, on s'en ira immédiatement parce que s'il y a plus d'articles, hein, il y a plus de débat, il y a plus rien, on pourrait juste aller prendre un thé à la buvette, mais le 49 3 ne nous y a pas obligé tout de suite. Un verre de vin, monsieur le Président, Karoutchi, monsieur le rapporteur. Oui, pardon je voulais finalement dans le droit fil des des propos de du président Karoutchi ça peut être à cet instant redire au ministre, moi j'entends alors le 49 3 la la manière dont le gouvernement intègre tous les réformes de retraites très honnêtement j'ai du mal à voir ce que le gouvernement intègre parce que de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la réforme des retraites, je suis pas sûr que les éléments chiffrés soit vraiment aussi précis que ça simplement et puisque on a, on est dans un régime bicamérisme, je voudrais dire que le Sénat notamment la majorité sénatoriale a fait le choix d'examiner le texte. J'entends les bonnes intentions en tous les cas dans les déclarations des 2 ministres, ce qui sera important c'est la copie qui sortira du Sénat et le sort qui sera réservé, ensuite, donc je pense qu'ici on est dans un temps de travail d'élaboration de la loi et du dialogue parlementaire républicain, mais je crois que le gouvernement a aussi finalement l'ardente obligation d'entendre ce qui peut se dire sur l'ensemble de ces bancs de notre assemblée parce que la démocratie française ne peut pas se permettre des situations, j'ai l'ai déjà dit, je crois, de blocage, notre pays doit avancer, vous avez évoqué la question de la réduction finalement des déficits quand d'autres pays se fixe un objectif d'être sous les 3 % en 2025 faire 2 ans de trop ou deux ans de plus ces 2 ans de trop, ben j'ai pas retenu votre formule magique parce que vous aimez un peu oui plus tard, c'est trop tard et bien écoutez, on verra, je sais pas si ce sera trop tard, mais enfin je nous alerte et j'alerte le gouvernement sur l'ardente obligation qui a d'entendre ce que les travaux du Sénat et les débats qui ont lieu à cette heure-ci. Monsieur Bruillet pour explication de vote. Merci madame la présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, juste pour dire notre groupe s'abstiendra sur cet amendement, on souhaite que les débats s'ouvrent aux gens s'ouvrent à l'instant sur ce projet de programmation mais j'en profite Monsieur le Ministre, pour faire 2 rectifications même trois la première, c'est que je m'appelle Breuiller et pas Breuiller ni voilà donc je, je le dis étant nouveau sénateur j'admets et ça me permet de faire une annonce publique Breuiller R qui se conjugue comme manger et caetera le la 2ème plus importante et et plus sérieuse, ça concerne ce que vous venez de dire sur le vote de la NUPES monsieur le midi, je pense qu'il faut dans cette enceinte que les choses soient dites non, la NUPES a demandé d'augmenter de façon considérable les aides à la rénovation thermique et je le dis parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les sénateurs et sur lequel j'espère même qu'il y ait un consensus très large au Sénat pour pousser, puisque tout le monde admet que MaPrimeRénov'dans ces petites rénovation n'est pas suffisant et donc il ne faut pas reprocher de vouloir supprimer un bouclier énergétique Kant il y a une obligation de gage en fait la demande était simplement de mettre des moyens, et comme c'était impossible d'aller chercher des recettes puisque il ne faut pas rétablir la CVAE, il ne faut pas enfin voilà, à chaque fois qu'il y a des recettes, vous dites non, je voulais juste rétablir ça et puis vous dire aussi comme vous étiez bien placés que les écologistes en 2014 tu sorti de la majorité de François Hollande au moment où il y a eu les baisses de dotations aux collectivités, ce qui me permet comme maire à l'époque d'avoir la conscience très tranquille sur ce sujet. Merci le président rénale.

on n'est pas devant la presse, pas devant le grand public, donc je crois qu'on ne peut pas effectivement. Devant nous, ici, nous faire le coup voilà vous savez parfaitement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale vais pas défendre hein mais effectivement il y a eu une volonté d'afficher 12 milliards je crois en faveur de l'isolation thermique, il fallait gager puisque c'est l'obligation et si je prends la parole, c'est que je suis responsable ici de l'article 40 et et dans l'article quarante s'applique aussi à l'Assemblée, il fallait gager et tout en indiquant d'ailleurs qu'on ne voulait pas toucher à ces crédits et donc la question, c'était juste de dire voilà, messieurs les Ministres, prenez en compte cette demande de 12 milliards et créer le budget, le budget nécessaire, vous le savez parfaitement, je ne vous apprends rien, Monsieur le Ministre, donc, de grâce, évitons ces effets de manche, non, personne n'a voulu supprimer le bouclier tarifaire voilà. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 à. Monsieur Savoldelli pour explication de vote. mais merci madame la présidence du juste un élément de de de clarification. Mon, mon propos était pas de mettre en cause la la possibilité d'activer le 49 3 pour le gouvernement, c'est tout à fait constitutionnelle il y a pas de problème. a, c'est, c'est une pratique politique, c'est une volonté politique, c'est un choix. Moi ce que j'ai entendu qu'est quand même limite. C'est justifié, hein, 49 froid par un amendement, d'où qu'ils viennent d'où qu'ils viennent. ça, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. On limite pas le débat parlementaire par un 49 3 parce que, il y aurait tels ou tels amendements qui met en difficulté l'exécutif et ce que j'ai entendu votre part Monsieur Attal. C'est, vous avez parlé des oppositions. Je vous le dis avec beaucoup de, de, de respect et très apaisé. Vous n'avez pas à choisir les oppositions. Elles ont une légitimité, elles ont une pluralité. Donc vous amusez pas trop à ça. Parce qu'avec le 49 3 on va quand même avoir un texte avec des amendements qui vont être sous la loupe. De l'exécutif et qui va revenir ici, c'est pour ça que je vous dis qu'on a une forme de 49 3 qui arrive, je suis moi aussi j'ai bien compris qu'on aurait pas le 49 3 ici, mais on va avoir un texte arbitré par le gouvernement au regard de majorité qu'il n'a pas et d'opposition qui veut choisir, alors qu'il cherche une majorité faut savoir laquelle il veut par contre attention on choisit pas ses oppositions, des fois, on peut se tromper d'où on regarde. Oui merci madame la présidente, cette aussi une suppression, c'est la suppression de l'alinéa 10 du rapport annexé. Bon, là, franchement, je ne vais pas plus long mais on a là un sujet sur lequel. Nous sommes en total désaccord dans le groupe. C'est l'analyse sur la question de la réforme des retraites. Voilà, faut faut se le dire, bon, voilà, et là il y a un positionnement où il y a une trajectoire qui est proposée avec des arbitrages qui viendront au dollar de nos débats de ce soir, j'en ai bien conscience : mais écoutez, moi je suis comme tous les citoyens français, j'écoute le président de la République, j'écoute les ministres voilà et je vois bien la trajectoire qui va être celle de de la retraite avec des des arguments sur le vieillissement sur l'indexation des prestations de retraite à l'inflation, et cetera, enfin, franchement, on a un problème de vue de viabilité de ce point de vue là et on a un système de retraite ou quand je regarde le PIB, il augmente de 0 5 point à l'horizon 2035 pour ensuite tomber à 1 point de moins que le coût des retraites actuelles en 2070 non mais vous voyez où on va donc la la trajectoire, nous nous y opposons fermement et nous demandons qu'on ait le débat, le débat vraiment le débat sur la question des retraites, un débat sur des vérités argumenter et là on prendra nos décisions, mais pas dans la condition de cet article dans le cas de la loi de programmation merci. Merci, monsieur le rapporteur pour avis. C'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées à l'amendement précédent. Monsieur le Ministre. Oui : avis défavorable également je saisis l'occasion pour répondre à certains points qui ont été évoqués avant je n'avais pas repris la parole pour pas allonger les débats, monsieur le rapporteur général Husson m'a interrogé sur les économies prévues dans la trajectoire lié à la réforme des retraites, je peux vous répondre très concrètement ce qui est intégré dans la trajectoire, c'est l'engagement de campagne du président de la République, c'est-à-dire un recul de l'âge légal de départ de 4 mois par an à compter de l'été 2023 ce qui produit une économie budgétaire brut de 8 milliards d'euros à horizon 2027. Voilà, ensuite il y a des recettes supplémentaires induites grâce à cette réforme et à l'amélioration du taux d'emploi qui en résulte, la dernière estimation de la direction générale du Trésor estime que : il pourrait y avoir des recettes fiscales et sociales supplémentaires entre 15 et 20 milliards d'euros raison 2027 liée à l'amélioration du taux d'emploi produite par la réforme des retraites, ça permet de répondre également aux sénateurs, ça vole des qui a interrogé aussi sur la réforme des retraites, donc c'est ça, en toute transparence, qui a intégré dans notre trajectoire pardon, hein, de l'amendement et du gaz, oui, je sais ce que c'est qu'un gage, enfin, un gage, c'est pas la part cosmétique et vous le savez parfaitement, ça montre qu'il faut faire des choix. Et la réalité, la réalité c'est que c'est pas un amendement qui produit le 49 3 et c'est pas un amusement, évidemment, monsieur le sénateur, mais quand le débat budgétaire dérive à coup de quinzaine de milliards d'euros non financé, pour reprendre les mots qu'il emploie et la première ministre tout à l'heure à l'Assemblée nationale sur le 49 3 les conditions d'un dialogue serein ne sont plus réunies, ne sont plus réunies. Voilà, c'est les mots qu'il emploie la première ministre dans lesquels je m'inscris. Monsieur Savary pour explication de vote. Oui, merci, monsieur le ministre a répondu par anticipation la question que je les lui poser, à savoir, justement, j'ai cru comprendre que dans la trajectoire, il y avait une économie de 8 milliards et je voulais savoir comment elle avait été calculé par contre, merci de ces précisions, puisqu'on a travaillé sur sur ces thèmes-là, c'est tout à fait exact en décalage, ça génère effectivement notamment des cotisations supplémentaires des cotisations fiscales également parce qu'il y a du travail supplémentaire qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, mais où c'est qu'figure derrière dans la trajectoire. Ces milliards d'euros, moi je ne suis pas un spécialiste mais pourquoi vous ne l'affichait pas clairement, il m'a pas semblé que ce que vous venez nous dire était clairement dans les propositions qui a été faite sur cette trajectoire budgétaire, j'ai pas tout lu, hein, mais il me semble que parce que plusieurs de mes collègues ont déjà posé cette question là, donc vous voyez, la transparence, vous êtes amené à l'affaire, pourquoi, pour la faire aussitôt dès le départ, ça donnerait un peu plus confiance par rapport aux chiffres qui sont annoncés sur ce type de document. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient, il n'est pas, z'adopté l'amendement 42 monsieur Savoldelli.

Combien coûte la baisse des impôts de production 2023. Bon, nous on pensait que c'était 10 milliards d'euros comme depuis 2 ans et baignant. Dans le tableau annexé. La baisse va rapporter 100 millions donc on veut bien savoir mais c'est c'est dans le tableau, hein, il faut le lire. Fournis par vous, donc on veut savoir comment une baisse de 10 milliards nous rapporte 100 millions la 2ème chose c'est: combien coûte la baisse du taux d'IS de 33 à 25 %. Vous l'estimé à 400 millions dans le tableau, on a fait un petit calcul. Comme c'est ça aux alentours de 54 milliards nous on pense que c'est plutôt. 4 4 milliards. Et pas 400 millions donc il y a certainement un problème, vous avez le pouvoir nous l'expliquer, et enfin sur le retour d'impôt sur les sociétés de la suppression des impôts de production. Au lieu de nous rapporter. ça va nous coûter 600 millions d'euros, donc je vous dis ça, parce que voilà, sur ce tableau indexé. Il y a, à mon avis, à notre avis, 3 erreurs qui quand même fausse le résultat, vous en conviendrez, si c'est bien le bon tableau que nous avons eu. Merci, vais je je propose une un avis de retrait et je voulais quand même revenir sur ce tableau, qui présente finalement la synthèse du coup des mesures nouvelles en prélèvement obligatoire et qui est dans le rapport annexé positif, il s'explique en fait par le ligne par l'effet de la ligne traitement en recettes des gains sur charges de service public de l'électricité pour rappel, l'État verse des subventions aux producteurs d'énergies renouvelables, elles sont calculées par la différence entre le prix contractuel elle prix de marché actuellement ses prix de marché sont et vous le savez, c'est la première fois depuis longtemps supérieur au prix contractuel en conséquence, l'État ne verse plus de subventions, mais en fait il perçoit des recettes et en comptabilité nationale, ça va tout de même s'élever à 9 6 milliards d'euros en 2023 et c'est des montants qui sont traités comme des mesures nouvelles en prélèvement obligatoire et qui compense donc sur le plan comptable, les pertes de recettes liées aux autres réformes je pense notamment à l'audiovisuel mais également à la la taxe d'habitation. Oui, j'ai été plongé dans le rapport annexé en réponse à monsieur, et surtout, j'ai découvert, j'ai fait la remarque à mes équipes que les pages ne sont pas numérotés, ce qui est objectivement compliqué, donc je je ne peux pas vous demander à quelle page, vous faites référence, je pense que c'est au tableau principal mesure nouvelle en prélèvement obligatoire en 2023, c'est ça : montrez-moi juste la page.

Donc, je vous confirme que la suppression de la CVAE c'est bien 4 milliards d'euros, même 4 virgule 1 milliards d'euros de coût, vous parlez de la baisse des impôts, de production, le zéro, un en réalité, ça c'est un impact des précédentes baisses d'impôts de production ces dernières années une forme de queue de comète de ces mesures, vous savez qu'il y a toujours un petit ajustement à la fin avec des acomptes qui sont versées idem sur la baisse du taux d'IS de 33 à 25 %, ça nous coûte évidemment pas sur l'ensemble de la baisse, 400 millions d'euros, ça serait faible, c'est là aussi l'achèvement de la baisse qui a démarré en 2017 qui s'est fait progressivement sur les années ça en l'occurrence, c'est à la queue de comète en tout cas la fin de la baisse qui concerne désormais à tout le monde en 2023, ça a un impact de 400 millions donc non, la baisse des impôts de production oui elle nous coûte budgétairement dans un 1er temps mais elle nous rapportera en terme d'activité économique sur du moyen et sur du long terme, c'est quand même ça la logique. On a, on avait avant d'engager la baisse des impôts de production des impôts de production en France cette fois supérieurs à ceux de l'Allemagne cette fois supérieur en, vous êtes un investisseur que vous voulez vous implanter dans un pays européen, vous comparez, de pays, vous voyez que les impôts de production sont cette fois supérieur d'un côté ou de l'autre de la frontière ben vous choisissez plutôt d'aller là où les impôts de production sont plus faibles et je peux vous dire Bruno Lemaire le dirait mieux que moi, s'il était ici puisqu'il était avec STMicro à Crolles, en Isère, qui a annoncé un investissement massif ils l'ont, ils ont dit d'ailleurs, quand ils ont annoncé leur investissement massif de plusieurs milliards d'euros dans les années qui viennent, ils le font, notamment en sachant que les impôts de production vont continuer à baisser dans les années à venir, donc oui, c'est ce qui permet d'attirer une activité sur notre sol et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, Bruno Lemaire il faisait référence dans son intervention avec une flèche acte avec vraiment du dumping qui a organisé, qui est un vrai risque aussi pour notre industrie en France et en Europe, on a raison, je pense 2 à baisser la pression fiscale sur les entreprises pour qu'elles installent des activités industrielles dans notre pays. Retrait ou défavorables, c'est cela. Monsieur le Ministre, oui : avis défavorable très bien monsieur Guey pour explication de vote. Je ne veux pas faire durer le débat merci madame la présidente, donc Monsieur le Ministre, vous confirmez parce que on a revérifié le tableau de l'an dernier nous parler de, de, de, de queue de comète, sauf que l'an dernier il y avait 10 milliards d'inscrits et là cette année c'est quoi. C'est encore dix milliards, donc ce n'est pas inscrit dans le dans le tableau, non mais on peut, je sais que vous êtes très habile et je vois bien qu'on ne s'affairent autour de vous, mais le tableau n'est pas bon pareil vous confirmez donc c'est bien 4 milliards IV, donc notre chiffre et le bon et il a inscrit au tableau 400 millions. Mais à la fin. Sur le tableau général mais du coup, je voulais donner, je ne peux pas la récupérer, c'est pas grave, je vous laisse, mais le chiffre à la fin il est pas bon, donc j'entends bien l'avis défavorable de la demande de retrait, mais comme le tableau présenté. il y a 3 erreurs pour nous fondamental, donc on va le maintenir et on va le voter et sachant que si on ne voit pas d'autres amendement, il faut que l'hémicycle Szasz bat le tableau qui est présenté n'est pas bon. Merci monsieur le maintenant enfin je je pas rallonger mais honnêtement je veux quand même que, que l'assemblée soit éclairée sur ce sujet-là, il y a pas d'erreur dans le tableau, le tableau, il présente le sol par rapport à l'année précédente. Donc, par définition, l'impact de la baisse d'impôts de production de 10 milliards qui a été réalisé en 2021 ben, il a été comptabilisés en 2022, et là 2023 par rapport à 2022, c'est ce qui reste donc la baisse, elle a eu lieu avant, or vous voyez bien qu'il y a les quatre, un milliard de suppression de la CVAE puisqu'on propose désormais de le faire en deux fois donc non ce tableau et tout à fait exhaustifs et donc je vous appelle à rejeter cet amendement qui, là aussi, entraînerait des difficultés constitutionnelles pour le texte. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas adopté, j'ai mes aux voix, l'article 1er qui vote pour, contre, abstention il était adopté article de l'amendement 27 monsieur Savoldelli. C'est directement le débat sur le traité de stabilité ça, vous en conviendrez, et là ce qu'on appelle la coordination de gouvernance, le TSCG, le fameux pacte budgétaire européen. Le rapporteur général avait estimé en commission qu'il fallait s'inscrire dans ces règles, plutôt que de les réformer, bon ton tact, c'est un choix politique, mais je voudrais éclairer ici les conséquences que ça. L'article 2 du TSG prévoit que l'objectif de moyen terme, lorsqu'on a une dette publique qui ne dépasse pas 60 % du PIB ne peut pas être inférieur à moins 1 % du PIB potentiel et de façon plus drastiques à moins 0 5 lorsque celle-ci dépasse les 60 %. Une fois qu'on suit ces chiffres là. On en arrive quand même au quotidien des Français, puisque lorsque l'objectif de moyen terme n'est pas atteint, les États doivent déterminer une trajectoire de solde structurel assurant, je cite, une convergence rapide vers cet objectif, donc le gouvernement prévoyant 12 ans il y a plus rapide, en effet, vous voyez, avec 8 années maintenant. Et là je je vous interroge là, Monsieur le Ministre, mais de quoi parle-t-on. En 2021, plus de la moitié des États membres de rester ne respectait pas le ratio d'endettement sur le PIB à 60 %. Quelle finances publiques de quels États pourront assurer la protection des peuples. La transition énergétique en Europe. Avec le carcan de ces règles budgétaires et comme l'article colle en partenariat avec le traité, évidemment, c'est pourquoi nous demandons sa suppression merci. Merci, monsieur le rapporteur. je pense que chacun a bien compris qu'il convenait de proposer une nouvelle évolution du solde structurel plutôt que de supprimer purement et simplement, c'est du gouvernement c'est l'objet même de la loi de programmation et ensuite le le principe d'améliorer le solde structurel est le seul de public, nous pensons que ça ne va pas assez vite, raison pour laquelle il faudrait, il ne faut pas supprimer cet article donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre, même avis défavorable. Oui : avis défavorable, ce qu'on construit en ce moment, c'est être capable à moyen terme, de respecter les règles européennes, tout en réduisant maîtrisant mieux notre dépense publique sans casser la croissance, c'est vrai que c'est complexe, que c'est un équipe qui est complexe à trouver je crois que dans la copie présentée par le gouvernement, on est sur cet équilibre, on peut trouver un meilleur équilibre dans la discussion qu'on aura sur la question des 60 % que vous avez évoquées pour le coup, ça fait vraiment partie des discussions qu'on a en ce moment au niveau européen pour donner plus de flexibilité sur ce sujet-là, c'est Bruno Lemaire qui porte pour le gouvernement, cette négociation au niveau européen et donc ça fait partie des sujets effectivement sur lesquels on travaille dans la réforme du pacte de stabilité. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui votent pour, contre, abstention, il n'est pas adopté. Amendement 61 présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, c'est un amendement que je présente au nom du gouvernement qui vise à rétablir la trajectoire, il était à présenté dans le cadre du projet de loi qui vous a été soumis, soumis, avec donc le retour sous les 3 % de déficit à un seul de 2 virgule huit très exactement à horizon 2027 on a eu le débat tout à l'heure dans la discussion générale, vous avez proposé une trajectoire qui implique d'être à un virgule 7 pour 100 de déficit en 2027 et de revenir sous les 3 % à horizon 2025 on souhaite tous faire des économies rétablir nos finances publiques, la question c'est le rythme vous proposer un rythme beaucoup plus soutenu, ce qui est aussi un appel à ce que nous fassions plus et moi je suis très ouvert, Bruno Lemaire, aussi, il l'a dit, mais faire plus, il faut le faire dans des conditions qui sont crédibles et soutenables trouver 25 milliards d'euros d'économies en plus dans 2 ans à horizon 2025, objectivement, pour nous, ça n'est pas crédible et soutenable et encore une fois, il faut dire où est-ce qu'on prendra ses 25 milliards d'euros, ce qu'on baissera le budget de la défense de l'éducation nationale, de la transition écologique c'est c'est très concret, puisque à l'article 12 de ce texte, il y a la programmation sur 3 ans à horizon 2025 de toutes les missions budgétaires de l'État, donc il faut dire dans quelle mission on prend les les 25 milliards d'euros, nous, on a construit une trajectoire qui impose. Une maîtrise des dépenses, d'ailleurs, on entend souvent les groupes de la gauche de cet hémicycle, ou de celui de l'Assemblée nationale, nous dire qu'on fait de l'austérité, on entend de l'autre côté, souvent sur les bancs de la droite, qu'on ne maîtrise pas assez, peut être que ça veut dire que, on a trouvé un équilibre encore une fois, on a dit qu'on était prêt à trouver une trajectoire qui permettrait de faire un peu plus même sensiblement plus d'économie, en passant d'une baisse en volume de 0 4 à une baisse en volume à zéro cinq pour les dépenses de l'État sur les 5 années qui viennent, mais la trajectoire qu'on présente, elle implique déjà un effort qui est en terme de dépenses publiques pour l'État, l'effort le plus soutenu depuis 20 ans. Voilà, depuis 20 ans, il y a jamais eu dans la une telle maîtrise de la progression des dépenses de l'État, donc l'amendement du gouvernement vise à rétablir l'Arctique tels qu'il figurait dans le projet de loi. Merci, monsieur le rapporteur. Et l'avis du rapporteur et de rester sur la proposition, on le fait par le Sénat je ai entendu tout à l'heure et à plusieurs reprises, on a, j'ai entendu le mot austérité, vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que de gérer avec attention, sérieux et de manière rigoureuse, un budget c'est pas non plus un gros mot, vous avez parlé de politique brutale d'austérité budgétaire mais personne nous a parlé de ici de brutalité, donc vous êtes en train de nous dire que vous entendez la demande d'effort supplémentaire que le ministre Bruno Lemaire adhère sur le principe, bah écoutez, vous êtes à mon avis sur la bonne voie, j'je j'ose même plus dire que vous êtes en marche parce que c'est déjà has been Old School, c'est comme on veut, et vous avez bien compris que la majorité sénatoriale souhaité que l'on consente des efforts supplémentaires pour que les efforts financiers soient ciblées, partout où la dépense doit être encouragée et que des économies et il nous appartiendra évidemment de le faire ensemble, soit également trouvé pour répondre à ce besoin que les Français attendent aussi de notre part de faire des économies sur la dépense publique et quand on invite l'État à faire le même effort proportionnellement que celui que vous demandez, pour pas dire que vous que l'État impose aux collectivités, je le redis ici, c'est déjà de la part du sénat un choix relativement audacieux et courageux, donc maintenant il appartient à l'État de faire ce pas, d'où l'avis défavorable. Merci Monsieur le Président, Patriat pour explication de vote. Oui, la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, moi je salue d'ailleurs la façon dont le Sénat attaque les discussions budgétaires, il le fait avec un esprit complètement différent de celui de l'Assemblée nationale constructif que que nous saluons mais il doit le faire sous le signe de la lucidité, de la responsabilité et de la sincérité. sincérité. Ni je disais qu'philosopher avec un marteau, j'ai l'impression qu'on demandant de 37 milliards et demi d'efforts supplémentaires, vous demandez aux pouvoirs publics de traiter et cela à coups de marteau alors vous dites on va prendre dans les Budgets non régaliens va le faire comme telle, on va peut être des leçons n'ont pas d'austérité mais de bonne gestion vous tracer une trajectoire dont vous savez très bien que la France, ça aura eu du mal à tenir, je vous rappelle quand même que c'est cette majorité qui, au cours du quinquennat précédent avait ramené le budget la difficile budgétaire en dessous des 3 % ce qui n'était jamais arrivé avant, donc elle s'inscrit dans la responsabilité, on en voulant le faire au bout demander aujourd'hui des efforts mais se demande d'effort, elle va voler en éclats dès qu'on parlera des collectivités locales, il serait plus question d'articles 23 et cetera on dépensera sans compter, on reviendra en arrière,

c'est que la gestion des finances publiques et je crois que le mixte a très bien rappelé tout à l'heure en cas de difficultés en cas de crise avec la crise qui a eu il y a eu sur le sanitaire avec, aujourd'hui, la crise financière due à l'inflation, par ailleurs, on peut, on peut le traiter les finances que globalement qu'on a tout, donc nous soutiendrons le gouvernement dans le rétablissement sa trajectoire qui à la fois lucides, responsable et puis on espère que, au bout du compte, à la fin de ces débats Sénat ayant fait preuve, j'allais dire de de de respectabilité, mais aussi de responsabilité nous arrive bourré nous aboutirons à la CMP, avec un accord qui permettra de satisfaire tout le monde, voilà merci. Oui merci madame la présidente, monsieur le Ministre, moi j'entends souvent parler d'austérité, je suis un peu comme le rapporteur général, on en parle, on en parle quand est-ce qu'elle a été appliquée en France, j'avais demandé à Pierre Moscovici quand il est arrivé à la tête de la Cour des comptes, je vais demander puisqu'il avait dit : il faut arrêter la logique austéritaire, je lui dis : c'est quoi la logique austéritaire et quand est-ce que ça a été appliqué quand on augmente les dépenses publiques de 20 30 50 milliards par an et à un moment donné où c'est pas possible, on peut pas parler d'austérité quand est-ce que ça a été menée, donc moi je suis pour une politique sérieuse et rigoureuse, voilà et je ne sais pas si ce qu'on appelle ça de l'austérité, mais on fait attention : un Euro est un euro et on fait attention à tout ce qu'on dépense et on n'a pas du tout l'impression que c'est le cas au niveau du budget de l'État Monsieur le Ministre, quand je vous entends parler de trajectoire, j'aimerais bien que vous se distinguer les dépenses courantes, des dépenses exceptionnelles ce c'est un peu facile de partir d'une référence où on a des dépenses exceptionnelles importantes et on dit : ah ben on va vous baisser ça progressivement vous inquiétez pas, ça va faire moins 04 ou moins 0 5 non, c'est les dépenses courantes qui doivent faire moins 0 5 c'est pas les dépenses courantes plus ces dépenses exceptionnelles, donc il faut faire très attention au point de départ. Monsieur Féraud pour explications de vote. Merci madame la présidente, avec cet amendement du gouvernement qui fait suite à l'amendement adopté en commission à l'initiative du rapporteur général, je crois qu'on est au coeur du débat que nous avons presque tripartite où il y a largement une position commune sur l'essentiel entre le gouvernement et la majorité sénatoriale, vous avez tous les 2 raison. D'abord le gouvernement quand il dit le ministre-quand il dit que de passer d'une trajectoire d'austérité à une trajectoire d'austérité brutal, ça n'est pas raisonnable, vous avez raison, mais la majorité sénatoriale et le rapporteur général a raison quand il dit que le gouvernement n'adapte pas sa politique de dépenses à sa politique de recettes en réalité de notre point de vue, vous avez tous les deux tort et c'est l'intérêt aussi de notre débat, c'est de ne pas. pas. Avoir une politique de recettes qui correspond à la nécessité, en terme de dépenses publiques et Monsieur le Ministre, c'est un peu sur cette question des taux d'imposition et de la recette fiscale la même histoire que celle que vous nous racontiez sur le gage tout à l'heure si, plus on baisse les taux, plus les recettes fiscales augmentent, alors pourquoi ne les baissez-vous pas davantage et plus vite pourquoi mettez-vous 2 ans a supprimé la CVAE et Nadine qui supprimé vous pas tout de suite puisque ça rapporterait encore davantage, donc tout cela n'est pas sérieux, nous ne nous prononçons pas entre les 2 trajectoire de dépenses, parce que les deux sont mauvaises, due à une trajectoire des recettes qui n'est pas réaliste. Merci Monsieur Bruillet pour explications de vote. Même vote une abstention : nous ne voulons pas participer au concours de Mister austérité pour notre part et nous comprenons les logiques, mais dès lors qu'on se prive des recettes évidemment ensuite il ne reste plus qu'à se demander comment ira le plus possible dans les dépenses, ça n'est pas notre choix, et donc pas de vote sur ces, sur ces 2 propositions, l'amendement et la proposition du rapporteur général. peut-être, j'ai la mauvaise définition de l'austérité en tout cas des fois. Je je cherche à à chercher où elle époux, elle est pas alors, s'il y a bien quelque part, ou elle est pas. C'est dans les dividendes des plus grands groupes hein. Non mais là cherchait pas mes, mes chers collègues. 160 milliards c'est 160 milliards il y a un rapport puisqu'on discute de l'austérité ou pas l'austérité au moins ça je suis sûr que pour les entreprises du CAC 40 il y a pas eu d'austérité, ça c'est la première chose la 2ème chose on va s'abstenir, mais c'était un peu le débat qu'on avait tout à l'heure parce qu'il va être où le compromis, le président Patriat nous dit on va aboutir à la commission mixte. Ah ben d'accord. Mais là, le compromis Les ou un peu plus un peu moins sur le sol structurelles pour arriver, dépenses publiques. Donc, ne croyait pas qu'on va arbitrer ça. Voilà, le gouvernement revient à l'initiale parce que la majorité sénatoriale durcit encore plus sur les dépenses publiques pensait pas qu'on va alimenter ça, donc c'est vrai qu'on va s'abstenir parce que pas participé au vote, bon. Mais moi j'aurais tendance à penser qu'on ne devrait pas participer au vote, quand c'est comme ça. Plutôt que même s'abstenir parce qu'on arbitre quoi. On arbitre voilà une une communauté de point de vue sur l'objectif unique étant la baisse, la baisse, la baisse, la baisse des dépenses publiques et puis après, ici ou là, on va dire : il manque des infirmières, il manque des enseignants, il manque des policiers, il manque des mais, bon, allez, dont taxe, ce que j'ai appelé tout à l'heure là la propension à être interventionniste sur les besoins et puis quand on parle des finances, là

Merci madame la présidente, peut être juste pour réagir à différentes interventions qui ont eu lieu, d'abord peut-être pour répondre au rapporteur général à nouveau ce que vous avez adopté en commission des finances ne revient pas, de notre point de vue à dire on demande le même effort à l'État qu'aux collectivités locales. Vous avez effectivement aligner l'effort, c'est-à-dire la baisse des dépenses en volume, l'objectif pour l'État sur celui des collectivités locales, moins 0 5 vous avez dit pour l'État, on compte pas les dépenses de crise et de relance dans la baisse des dépenses, or elles sont comptées pour les collectivités locales dans les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, vous avez des dépenses qualifiées de dépenses de crise qui seront donc comptabilisés. De sorte que, avec ce que vous avez adopté les dépenses de l'État en valeur progresserait dans les 5 ans qui viennent de un virgule 5 % là où elle progresserait de 10 pour 100 pour les collectivités locales, donc il y a pas du tout de parité sur la trajectoire qui est dans cette LPFP moi je veux recontextualiser et peut-être prendre un peu de recul sur ce qui s'est fait dans ces derniers quinquennats. La dépense publique, toutes administrations publiques a progressé en volume de 1 virgule 4 % dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Augmentation de 1,4 % dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle a augmenté de 1 % dans le quinquennat de François Hollande. Elle a augmenté de 0,9 % dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et dont la trajectoire que nous présentons dans cette loi de programmation des finances publiques, elle augmenterait de 0 6 % c'est donc l'effort de maîtrise de dépenses déjà le plus fort depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs décennies 4 % d'augmentation de dépenses sous Sarkozy un % sous François Hollande 09 dans le premier quinquennat Macron 0 6 % dans le quinquennat qui s'ouvre avec ce que vous avez adoptée, elle ne serait que de 0 1 % 0 2 % ça ne nous semble pas soutenable, sauf encore une fois, à faire des coupes massives dans nos services publics dans les toutes prochaines années 25 milliards à trouver en 2025 ou à casser la dynamique de croissance économique, je voulais simplement répondre aussi à Monsieur Féraud, ce que vous appelez. Une politique de recettes, enfin il faut dire les choses très clairement ce que vous proposez, c'est d'augmenter massivement les impôts. Politique de recettes, c'est augmenter les impôts, nous, pour le coup, on assume de ne pas vouloir augmenter les impôts qui pèsent sur les Français et même de les baisser et en réalité, si il fallait à couvrir l'intégralité des dépenses que vous proposez, ce serait pas simplement une taxe sur les dix super profits qui permettrait de le couvrir, ça devrait être une augmentation massive des impôts qui concernerait beaucoup de Français, y compris les classes moyennes, c'est vrai que ça n'est pas notre projet. Je mets donc aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui vote pour. Qui vote contre.

qui a pour pour objectifs la baisse des dépenses publiques. De l'État et des collectivités territoriales, nous, nous pensons que la aussi je sais que ça ne va pas plaire à l'hémicycle. Il avait été reconnu. Mais il y a une compétition austérité a entre la droite sénatoriale et le gouvernement. Et il va falloir nous dire pour la baisse des dépenses publiques où c'est qu'on les prend par exemple de l'État, moins de fonctionnaires ou. Dans la police, dans la justice dans l'Éducation nationale dans les hôpitaux, non mais il faut nous expliquer ou parce que comme ça il y a de l'humour, l'urgence partout et des besoins criants partout. Il va falloir nous expliquer où c'est qu'on fait l'austérité et comme il y a un petit débat. Sur la caution austérité aujourd'hui le 1er budget de dépenses. C'est l'aide publique aux entreprises hors Covid. 160 milliards d'euros donnés au Capitole. C'est 2 fois le budget de l'Éducation nationale, vous voyez ça. Ce le Ministre, vous êtes en charge des comptes publics hors Covid ce chiffre de 2019 ça voilà, ça c'est une politique qui donne beaucoup au capital sans contrepartie, jamais de contrepartie et par contre pour tout à ne pas d'autres dépenses publiques, il va falloir serrer la ceinture, donc je vous demande où c'est qu'on va chercher les postes de dépenses. Où et si c'est par les fonctionnaires, donc c'est aussi la question de l'investissement : 25 milliards a été prévu, dont 9 milliards pour la rénovation des logements si on doit baisser, ça veut dire moins d'investissements, notamment pour la rénovation des bâtiments en pleine crise énergétique, donc il faut nous expliquer comment vous allez boucler tout ça, je vous remercie. est de supprimer de l'amendement, qui est de supprimer l'article qui présente la trajectoire d'évolution des finances publiques, donc, comme pour l'article 2 je rends évidemment un avis défavorable et je donne tout de suite mon temps restant de parole au ministre qui doit pas en abuser pour qu'il apporte ses réponses aux sénateurs gay. Monsieur le Ministre. Oui : avis défavorable également cet article 3 il y a tous les chiffres hein dans cet article 3 si les supprimer, là aussi, constitutionnalité de la loi, mais encore une fois, il y a une cohérence, vous vouliez rejeté le texte avec une question préalable, ce qui n'est pas évidemment notre projet, donc avis défavorable. Je voulais revenir sur ce que vous avez indiqué sur les aides aux entreprises, on entend beaucoup cet argument utilisé 160 milliards d'aides aux entreprises, comme si ces 160 milliards c'était une forme de cadeau que l'État faisait chaque année aux entreprises, en grande majorité dans ces 160 milliards d'euros il y a quoi, il y a les allégements de cotisations. Qui ont permis aux entreprises de recruter qui ont permis au coût du travail de baisser dans notre pays et qui permettent aujourd'hui à notre pays d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, taux de chômage des jeunes, le plus bas depuis 40 ans, le taux d'emploi au plus haut depuis qu'il est mesuré, pas encore assez haut, hein, pour reprendre les débats qu'on avait tout à l'heure donc majoritairement ce qu'on appelle des aides aux entreprises, c'est tout simplement des allégements de cotisations qui permettent à des millions de Français aujourd'hui de travailler ou d'avoir retrouvé un emploi. Je mets donc au monsieur Guy. sur les aides aux entreprises, on peut avoir un un un long débat, moi je m'en rappelle, c'était la baisse de TVA et baisse de cotisations pour les restaurants, nous a dit : vous allez voir les prix vont baisser. Et ça va recruter, et les salaires vont augmenter, bon je ne suis pas sûr que les prix et baisser franchement non, mais, et ça a été calculé les prix n'ont pas baissé les salaires, allez demander aux serveurs ou serveuses aux plongeurs ou au cuistot si leur salaire augmenter et, par contre, bon, la baisse a été pris par les restaurateurs non mais voilà, vous voyez, là on ne parle pas des grandes entreprises, parce que souvent on nous reproche ou parler que des grandes entreprises sur une question sur la restauration, ça a pas marché, donc il faut essayer autre chose et on pourrait vous donner beaucoup d'exemples sur les grandes entreprises, où l'argent a pas servi à recruter pas servi sur la recherche et développement pas servi à augmenter les salaires mais plutôt à à continuer à engraisser un certain nombre d'actionnaires. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Compte. Abstention : il n'est pas adopté, mes chers collègues, je vais suspendre la séance de vous informer que, compte tenu du nombre d'amendements restant examiner sur ce texte soixante-huit nous ne commencerons pas ce soir l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables mais nous finirons la programmation des finances publiques, la séance sera donc reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'Ordre du jour, la séance est suspendue, bon appétit.